La séance est ouverte, le compte rendu intégral de la séance du 13 juillet 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Je n'ai pas reçu d'observation. Je n'en vois points en séance le procès-verbal est donc adopté.

Patrick Masclet nous a quittés le 4 juin dernier. Il s'est éteint à l'hôpital Percy de Clamart. Oui, lutter avec un courage exceptionnel contre la maladie. Et pourtant. Nous avions avec lui un peu tous repris espoir. C'est au nom du Sénat. Que je l'ai accompagné le 9 juin. En l'église Saint-Nicolas le sa commune. Nous étions autour de sa famille. Autour de ses amis. Nous lui avons rendu hommage en votre présence, monsieur le ministre, Gérald armada en présence. J'plusieurs. Le président Bruno Retailleau. Un grand nombre de nos collègues du département du Nord et du Pas-de-Calais et de Jean-René Lecerf. Cette belle cérémonie.

Sa maladie, sa lutte. Patrick Masclet en parler avec beaucoup de lucidité. Malgré une plusieurs naturel. Son combat ne l'a jamais empêchée de continuer à suivre jusqu'à ces derniers jours la vie de son département et les travaux du Sénat. Je souhaite exprimer une nouvelle fois à Madame inscrire leurs enfants Stéphanie Pierre-Antoine. à toute sa famille à tous les proches, nos pensées au nom de tout le Sénat. Avec Patrick Masclet, c'est une figure majeure de la Russie et l'un des élus les plus respectés du département du Nord qui s'en est allé. Il était amer. Un président. De l'association des maires du Nord. Un parlementaire, un humaniste à la fois pondéré, chaleureux, un serviteur de la République constamment dévoués à l'intérêt général a défenseur des communes rurales de son département. Bon. Il aimait les gens. Il était attentif. à l'écoute de chacun. Calme. Il était aussi volontaire, énergique dans l'action. Homme de terrain comme 2 dossiers au fond il ne laissait place ni à la résignation, ni au scepticisme serviteurs de la République, il a toujours été porteur des valeurs qu'il avait fait sienne celle du gaullisme, lui qui aimait profondément l'Irlande peut-elle a-t-il arpenter dans la baie de Cacharel. Dans le Connemara cette même plage qui vit le général de Gaulle. Un temps s'en aller. C'est dans le combat que se révèlent les hommes que notre peuple jugera digne et capable de diriger ses actions. C'est ce qu'écrivait Charles-de-Gaulle. Au fond, Patrick Masclet dans sa simplicité était de ces hommes là. Mais dans le Nord, Asier il aimait raconter qu'enfant il accompagnait son père à la pêche dans les marais d'Arles. Une passion qui ne l'a jamais quittée. le. Une commune dont il deviendra le 1er magistrat durant 22 ans. Patrick Masclet. C'est aussi une longue carrière d'enseignant après un diplôme universitaire de technologie de génie électrique à diplôme d'études approfondies d'automatismes, l'École Normale de Lille l'École normale nationale d'apprentissage en électronique. Il est agrégé de génie électrique, sa carrière de professeur agrégé le conduisit successivement à Valenciennes, à Cambrai, à Douai. Avant d'être chargé de la formation des professeurs de génie électrique à l'institut universitaire de formation des maîtres, à Villeneuve d'Ascq et d'être ensuite professeurs de BTS ou lycée Pasteur à Hénin-Beaumont. Patrick Masclet s'investit très tôt dans le milieu associatif, toujours soucieux de se mettre au service de ses concitoyens et animé par le désir de justice. Son engagement associatif. Le conduisit bientôt à s'engager dans les responsabilités locales, je l'évoquais commet vers le alors là, vous savez, c'est à la croisée du canal du Nord et du canal de la. Il en fut le maire, mai 1995 est réélu sans cesse en 2014, avec un score de 78 pourcent des des voix dans sa commune. Il fut aussi conseiller régional durant 17 ans et un président attentif. L'ensemble des maires du Nord. Il le fit aussi comment du bureau et vice-président de l'Association des maires de France et comme un homme du Nord naturellement attachés à la cohésion sociale. Au sein du bureau des maires de France. J'étais amer heureux et comblé, nous a-t-il écrit, il y a quelques mois je n'étaient que locataires mais j'de garder la maison, dans le meilleur état que je pouvais. J'ai même essayé de l'embellir. Le service public ont été améliorés, diversifier les services marchands ont été étoffés, la ligne politique de tous les mandats, ils étaient à son conseil municipal, c'était de bien vivre et vieillir au village. Le 1er mars dernier c'est ça d'être maire. Et il dit à ce moment-là, c'est un déchirement est un Crèvecoeur, la fonction de maire est une mission exaltante et passionnante qui humainement m'a beaucoup apporté. Le choix de ce recul, le fini à la fois pour se mettre en adéquation avec le texte qui va s'appliquer dans quelques semaines, mais aussi par raison. J'ai encore l'envie. Mais il faut être raisonnables. Et ce mot Molière meurt en scène et après, point d'interrogation. 3ème si on la liste conduite par Valérie Létard, c'était en 2011. Et Jean-René Lecerf. Nous rejoint ici, c'était le 22 avril 2015 si on les bancs du Palais du Luxembourg, il y représente le département du Nord. Quand Jean-René Lecerf nous quitte, nous dit je veux pas être un sénateur TGV et me consacrer pleinement à ce département à ce département, il y a la fois des souffrances et et désespérant.

quelle est cette commission un peu le coeur du réacteur du Sénat, je le cite encore. Durant les 25 mois qui passa parmi nous, il fut un défenseur inlassable des collectivités locales notamment, et j'y reviens. il rapporte ainsi on n'avril 2016 devant le Sénat au nom de la commission des lois, avec conviction, avec succès, la proposition de loi de Jacques Mézard, devenu ministre et modifiant la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Souvenez-vous frictions par pragmatisme et par bon sens rallongée d'un an le délai d'entrée en vigueur des nouvelles intercommunalités. Malgré les contraintes du traitement qu'il subissait Patrick Masclet suivie jusqu'à ces derniers jours avec une attention constante, les travaux du Sénat, comment ne pas évoquer un café que nous avons partagé quelques jours avant dans mon bureau mais quelques extraits de l'une de ses dernières interventions dans cette émission, c'était le 15 mars dernier nous examinions le rapport d'information de la mission de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre des dernières lois de réforme. Et il disait : c'est pour moi un plaisir de vous retrouver après quelques mois d'absence, et je veux vous apporter mon témoignage d'élus du Nord. Patrick Masclet, c'est plus d'un quart de siècle d'engagement politique. Je crois qu'on n'oubliera pas, même s'il est resté trop peu de temps, son sourire, son calme, sa simplicité le revoit moi dans l'hémicycle, Médicis, tout près de l'endroit où nous entrons. Et c'est toujours un bonheur. échanger avec lui.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs. Chère madame chargeant René Lasserre. C'est une lourde charge qui me revient, Monsieur le Président de prononcer quelques mots au nom du président de la République et du gouvernement pour avoir une pensée. Que vous permettrez très amical envers Patrick masqués qui était un homme que personne ne pouvait détester. Lors de son enterrement, vous l'avez dit, monsieur le président, a foule innombrable des élus locaux, des personnalités mais les citoyens de sa commune et d'ailleurs ont rendu un hommage. Tout assez mérité. Un homme dont Jean-René Lecerf, a dit dans son oraison qui ne lisait jamais de mal de personne. Et il est vrai que Patrick Masclet ne disait jamais de mal de personne. Je veux dire, hein. à l'ensemble ses collègues pas je partage la peine et je partage appelle surtout de le voir absent, même si il s'affiche parmi nous.

nous nous adressons au nom du gouvernement et à tous les sénateurs nos sincères condoléances. Personnellement, je regrette de ne pas voir Patrick Masclet continuer son combat politique, il était un militant, vous l'avez dit avant tout un militant du Nord, un militant des villes, un militant de notre région, un militant du gaullisme. Ce qui pousse sans doute avoir. Vis-à-vis de chacune et chacun beaucoup d'empathie, parce qu'il était très attaché, vous l'avez dit, Monsieur le Président. à la cohésion sociale et à l'attention des plus faibles. Il était maire d'une ville symbolique dans le Nord, et c'est peut-être un moment d'autant plus délicat que de regrets ça. Sa perte que savoir commode juillet au mois d'août, il était souvent en Irlande pour pêcher avec sa femme, avec ses enfants et que je sais de. Tout la bas le bonheur et la tendresse qu'il avait, pour sa famille. où nous allons terminer cet hommage, il nous revient sans doute de dire à Patrick masqué à sa famille, bien sûr, qu'seront toujours dans le coeur de la République, lui qui était un parlementaire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, très assidus, notamment en commission des lois très attentif vis-à-vis du gouvernement, peut-être pointilleux mais c'est exactement ce que nous attendions et lui qui était si gaulliste revient au moment de dire ces quelques mots ici. Qui n'avait un jour compléter la fresque, général de Gaulle avait cité à la fin de ses Mémoires de guerre, soyons fermes juste et fidèle, car à la fin et il y a plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont passé. Je remercie. Je vous invite maintenant. Communion avec la mémoire de Patrick Masclet à partager un moment de recueillement.

de recueillement. Conformément. à notre tradition en signe d'hommage à Patrick Masclet nous allons. Sport nos travaux, la séance est suspendue, elle sera reprise à 15.

La séance est reprise. Par lettre en date de ce jour, et conformément à l'article 20 de terre du règlement, monsieur Philippe Bas, président de la commission des lois, a indiqué à monsieur le président du Sénat, que la commission des lois, demande au Sénat, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires de lui conférer le mais pirogues hâtives attribuées aux commissions d'enquête pour le suivi de la loi du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence pour une durée de 4 mois sur la proposition donc de monsieur le président du Sénat, nous pourrions examiner cette demande jeudi 20 juillet 2017 il y a un sur à 9 heures 30. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y en a pas, donc il en est ainsi décidé. Monsieur le ministre, mais, chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la procédure accélérée a été engagée sur ce texte dans la discussion générale, la parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur,

Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur de la commission des lois, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères de la Défense des forces armées, mesdames et messieurs les sénateurs. J'étais vendredi dernier à Nice. Pour la cérémonie de commémoration de l'attentat du 14 juillet. Toute seule, et tous ceux qui étaient présents ce jour-là. J'avais le coeur serré. Parce que c'était toute une vie. Qui était touché. Chacune et chacun ayant parmi ses proches, ses amis dans l'école de ses enfants sur son lieu de travail. Une personne qui avait été ce jour-là. Oui. Ou gravement blessée, oui, il y a un peu plus d'un an. Ils étaient des dizaines de milliers sur la promenade des Anglais à regarder le feu d'artifice. Il faut imaginer le sourire des enfants. La joie des parents ou les grands-parents qui pensait leur avoir apporté un moment de bonheur en les amenant ici. Et puis soudain. L'horreur absolue. Des centaines de blessés 80 6 personnes arrachés à la vie, tout simplement. Parce qu'un individu fanatisés par la propagande terroriste avait décidé de passer à l'acte On aurait pu être beaucoup plus lourd. Si des civils, des policiers n'avait pas au péril de leur vie, intercepté le camion. Alors qu'il allait entrer dans la zone où la foule était la plus dense. Dans les rues de Nice aujourd'hui. On ne croissent pas une personne. Il n'a été profondément touchée par ce drame. On ne croissent pas une personne qui ne se souviennent de ce qu'elle faisait, où elle se trouvait en cet instant tragique. Non, plus jamais les 14 juillet niçois n'auront la même saveur. Et c'est en ayant ce souvenir-là. Gravé dans les que cet après-midi, je viens vous présenter le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Pour sortir de l'état d'urgence. Mais en même temps. Afin que soit mis en oeuvre tout pour que de tels drames abominable ne se reproduise pas. C'est là ma responsabilité de ministre de l'Intérieur. Et je ne l'oublierai jamais je n'oublierai jamais. Ce que, au cours de ces années, nous avons tous ensemble, vécu. Oui, nous voulons sortir de l'état d'urgence. Mais nous ne pouvons le faire sans adapter notre dispose. Ce type de lutte contre le terrorisme. Certes. Celui-ci, vous l'avez indiqué largement en commission. C'est déjà beaucoup renforcé dans les dernières années sous l'impulsion du Sénat. Et votre rapport l'indique très largement 8 ex-sont venus renforcer les moyens de l'État pour lutter contre ce fléau. Mais il nous reste encore à prendre. Des mesures qui sont pour nous essentielles. C'est là l'objet du projet de loi dont nous allons débattre cet après-midi. Car. Nous le savons. La menace terroriste est toujours là, braillant. Et si certains peuvent croire qu'avec la prise de Mossoul avec la progression des forces antijihadistes, à Raqa, le risque d'attentat est désormais moins fort, il se trompe. Car Daech reste toujours présent là où les États faillite. Les attentats de Manchester ou de Londres ont montré que ceux qui commettent des attentats terroristes en son nom, sont capables de frapper partout et à tout moment. Quant à des organisations comme Al-Qaïda. Elles ressurgissent. ça développe un nouveau Yémen au Sahel sans que l'on puisse exclure qu'elle fera demain en France. Il y a cette menace-là. Télécommandé. Et celle, plus diffuses et donc plus difficiles à prévenir de ce que la propagande a fait ou peut faire basculer. Cela peuvent passer à l'action en étant de plus en plus courts avec des instruments de plus en plus rudimentaire. La menace. Et donc plus complexe à détecter. Il faut pouvoir agir plus rapidement protéger davantage, c'est c'est ce que vise ce projet de loi. Il ne s'agit donc pas, vous l'aurez compris. D'un texte comme les autres, de ce que l'on peut décaler au gré d'un calendrier parlementaire, il s'agit d'une loi urgente. Crucial. Une loi essentielle parce qu'elle touche à la sécurité immédiate de nos compatriotes. Mesdames et messieurs les sénateurs. Avant d'emmener au détail des mesures présente dans ce projet de loi, permettez-moi de souligner que notre constante volonté. Et, malgré le danger que je viens de l'écrire. A toujours été dans ce texte de concilier efficacité de la lutte antiterroriste et préservation des libertés individuelles et que c'est à l'aune de cet équilibre qu'il convient d'analyser les mesures que nous vous proposons. Le 1er article traite, vous le savez, de la question des périmètres de protection pourront après ce texte de loi être instauré par les préfets pour sécuriser les grands événements culturels, sportifs. Depuis le 14 novembre 2015, cette disposition a été utilisé 71 fois. Sans elle, l'Euro 2016. Des événements comme le Tour de France n'aurait sans doute pas pu se tenir. Si l'on s'en tient à la seule période correspondant à la 5ème prorogation de l'état d'urgence, c'est-à-dire depuis décembre 2016 19 zones de protection ont été établis par les préfets. Par les fouilles, les mesures de sécurité qu'elles autorisent. Ce sont elles qui ont rendu possible récemment. La sécurisation du festival de Cannes des FrancoFolies à La Rochelle, et bien sûr celle du défilé des. ChampsElysées le 14 juillet dernier. Cette mesure ne restreint donc pas les libertés non elle est garantie, elle les rend possible. Parce que ce sont ces zones de protection. Ils permettront aux Français de continuer à se divertir à se cultiver, là où les terroristes voudraient nous voir renoncer à notre mode de vie. Elle protège nos libertés collectives. Mais elles sont aussi respectueuses des libertés individuelles. Parce que. Telle que nous proposons cette mesure. Elle sera respectueuse du choix de chaque individu, et s'il le souhaite, pourra se soustraire aux fouilles et sera accompagné hors du périmètre par des policiers ou des gendarmes parce que la définition du périmètre sera sous contrôle du juge adaptée et proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances enfin parce que nous avons pourrait, vu que les règles d'accès au périmètre devront être adaptés aux impératifs de la vie privée, familiale et professionnelle. La commission des lois a souhaité que l'établissement de telles zones soit conditionné par l'existence d'un risque actuel et sérieux. Je le dis d'emblée, nous ne partageons pas cette option, parce que nous pensons qu'en ce moment, le risque est toujours actuel est sérieux, c'est que tout rassemblement d'ampleur. Vote aujourd'hui faire l'objet d'une attaque. Aurait-on par exemple évoqué il y a un an à risque actuel est sérieux à propos du feu d'artifice de la promenade des Anglais. De même, la volonté émise par la commission d'exempter de fouiller les riverains nous semble porteuse risque important. On ne peut jamais exclure en effet qu'un individu radicalisé et su secret opportunément déjà tâche au sein de la zone contrôlée. profits cette année pour la Fête des Lumières qui prend un vaste périmètre de la ville. Et qui évidemment. Prévue à l'avance, autour du 8 décembre et donc parfaitement identifiables. Tout individu peut se louer un appartement, dire qu'il habite ici et donc se dire exemptée de toute fouille et demain commettre un attentat. Nous avons dans les rues. 2 millions, 3 millions de personnes en 3 jours. Imagine-t-on ce que pourrait donner un attentat dans une telle folie. Je pourrais citer d'autres exemples. Si nous voulons tenir la grande braderie de Lille ou le marché de Noël à Strasbourg vous exemptant de. L'ensemble des habitants, alors je crains que nous ne puissions pas tenir de tels événements. C'est pourquoi, sur ces 2 aspects de l'article 1er je proposerai que nous nous en tenions à la version initiale du texte, il me semblent plus opérationnels, le second article de notre projet, traite de la possibilité donnée au préfet d'ordonner la fermeture administrative de lieux de culte L à encore, cette mesure répond à un enjeu majeur et médias. Pour lutter efficacement contre le terrorisme. Depuis la mise en place. De la 5ème phase de l'état d'urgence, ce sont 5 lieux de culte qui ont été fermés. évitant en ce moment même. Que plusieurs dans une dizaine d'individus ne suivent prêches fanatisés. Il est donc important de pouvoir laisser cette possibilité, encore une fois dans le texte que nous vous proposons, nous avons pas. Prévu un ciblage serré et un contrôle plus important que sous le régime de l'état d'urgence ainsi l'exécution de ces mesures sera-t-il très encadrée, puisque la durée de fermeture ne pourra excéder 6 mois et que les responsables des lieux de culte. Pour en demander la suspension en référé. Devant le tribunal administratif, ce recours en pêchant à la main, à mesure de prendre son caractère exécutoire. Je me réjouis que cette disposition ait pu faire l'objet d'un vaste consensus en commission. Les mesures de surveillance dont il est question dans l'article 3 du projet de loi. Ont-elles conduit à ne plus vive discussion. Je tiens donc à rassurer toutes celles et tous ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes en soulignant d'abord que le projet de loi met fin à la possibilité existant dans l'état d'urgence d'astreinte à résidence, un certain nombre de personnes. Nous avons souhaité cependant. Le ministre de l'Intérieur se trouve en capacité de prononcer les mesures de surveillance individuelle. Parce qu'il laisse agit sans doute de la technique la plus efficace pour détecter l'imminence du passage à l'acte d'un individu sur lequel pèsent de lourds soupçons, encore fallait-il que cette mesure plus très exceptionnel. Son utilisation sera donc très encadrée, puisque la surveillance ne pourra concerner, je cite, que les personnes à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qui soit entré en relations de manière habituelle avec des organisations terroristes soit ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes, c'est un texte très ciblée parce que nous n'avons pas voulu que cette mesure puisse être étendue à tous et en particulier ne puisse concerner l'ordre public, par ailleurs, les mesures de surveillance devront être compatibles. Avec la vie privée et professionnelle des personnes. Ce qui implique qu'elles autoriseront des déplacements dans un périmètre au moins équivalent. à celui de la commune. Au moins équivalent pas la petite commune, monsieur le rapporteur, il existe aussi de grandes communes, et donc c'est au moins cela pourra être plus en août. Conformément aux analyses et recommandations formulées par le Conseil d'État, en décembre 2015, elles ne permettront pas d'astreindre la personne à demeurer à son domicile la nuit. La commission des lois a souhaité revenir sur l'obligation pour les personnes surveillées de pointer une fois par jour. Au commissariat, nous ne pouvons accepter cette proposition, la rédaction proposée par la Commission. Pourrait en effet permettre à un individu de passer 3 jours sans le moindre signalement. 3 jours c'est un délai largement suffisant. Pour échapper à la vigilance des services et passer à l'acte. Je me refuse donc apprendre à untel risque et propose d'en revenir au texte initial. De même, le gouvernement estime nécessaire de rétablir l'obligation supprimée par la commission de communiquer à l'autorité administrative, les numéros d'abonnement identifiant technique de tout moyen de communication électronique pour faciliter la surveillance des personnes concernées. Et je tiens à redire à cette tribune que cette obligation ne portera pas sur les mots de passe et ne permettra donc pas à l'administration d'avoir accès au contenu. Nous aurons à débattre également des mécanismes retenus pour autoriser la prorogation de la mesure que la commission propose de conditionner à l'intervention du juge des libertés et de la détention, mais je pense que nous arriverons à trouver un accord, nous considérons que l'intervention du juge judiciaire n'est pas nécessaire et même qu'elle n'est conforme ni au principe de séparation des pouvoirs, ni à la tradition juridique française, mais le gouvernement est malgré tout sensible à la préoccupation exprimée par la commission, j'aurai donc l'occasion de défendre un amendement qui prenne en compte l'impact que pourrait avoir le renouvellement des mesures de surveillance de la personne concernée. Enfin, le 4ème article du projet de loi aborde la question des visites domiciliaires et saisi dans le cadre de l'état d'urgence, il s'agissait de perquisitions qui pouvaient être menés à la discrétion de l'autorité administrative pour prévenir tout trouble à l'ordre public. Cet outil s'est avéré profondément utile. Puisque je rappelais devant votre commission des lois, ces perquisitions avaient permis de saisir 600 armes dont plus de 78 armes de guerre.

Eh bien non, depuis le 5ème, prolongement de l'état d'urgence le 22 décembre 2016, ce sont 2 préparations d'attentats que les perquisitions nous ont directement permis de prévenir 2 préparations d'attentats alors que les éléments alors en notre possession ne nous aurait pas permis de procéder à une perquisition judiciaire. Il serait donc peu responsable de se priver d'une telle disposition. En même temps nous avons conscience de ce qu'une visite au domicile d'un individu avec la possibilité de retenir ce dernier durant un laps de temps peut comporter d'atteinte aux libertés, c'est pourquoi ce régime des visites domiciliaires et saisi sera là encore extrêmement ciblés, puisque, comme les mesures de surveillance, il ne pourra concerner qu'une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qu'qui soit entrent en relation, de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant facilitant ou participant à des actes de terrorisme soit soutien ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant apologie de tels actes. Je rappelle que dans l'état d'urgence, les perquisitions pouvait être appliqué à tout individu constituant une menace pour la sécurité et l'ordre public. C'était extrêmement large et là, nous avons voulu que ce ne soit que pour des actions qui soient en rapport avec le terrorisme. C'est pourquoi, surtout en raison de la violation du domicile qui l'autorise, nous avons souhaité que ce régime soit soumis à un double contrôle de l'autorité judiciaire d'abord celui du procureur de Paris qui, du fait de sa spécialisation dans la lutte contre le terrorisme se verra informés de toute visite effectuée sur le territoire national et pourra ainsi s'il le juge nécessaire judiciariser le renseignement et reprendre l'enquête à son compte ensuite et c'est la principe. L'innovation de ce texte. Le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris devra autoriser la visite et contrôler l'exploitation qui sera faite du matériel saisi sous son autorisation. La commission des lois reconnu se réserve d'une information du procureur territorialement compétent. Cette rédaction, permettant une meilleure coordination entre autorités administratives et autorité judiciaire confortant cette dernière dans son rôle de gardienne de la liberté individuelle, au sens de l'article 66 de la Constitution. Je veux en remercier le rapporteur et le président pour l'esprit constructif qu'ils peuvent avoir. Dans cette commission vous incompris compris, mesdames et messieurs, notre obsession avec ce texte est de concilier la protection face aux ce terrorisme et cette préservation absolue des libertés qui constitue évidemment le socle de notre démocratie. Si je parlais en introduction de l'attentat de Nice, c'est parce qu'. Je souhaite durant nos débats, nous ne perdons jamais de vue que les décisions que nous allons prendre durant cette séance. On vont avoir des impacts très concrets. Quand nous évoquerons les zones de protection, c'est en effet de la possibilité pour les Français de se cultiver, de se divertir en sécurité dont nous parlerons. Quand nous statueront. Sur la possibilité de fermer administrativement des lieux de culte. C'est de la manière d'éviter la radicalisation de nombreuses personnes dont nous débattrons. Quand nous traiterons des sujets, des mesures de surveillance individuelle des visites et saisi, c'est les moyens que nous nous donnerons pour démanteler des réseaux terroristes. Invité : les attentats dont il sera question oui, toutes les mesures. Sûr que contient cette loi sont là pour que nous évitions d'avoir demain des morts, des blessés. On nous dit parfois. Que le droit pénal suffit mais je vous rappelle qu'ici nous sommes en amont du droit pénal dans la lutte contre le terrorisme et coeur. Dès que les indices sont graves et concordants, nos services se tournent immédiatement vers l'institution judiciaire. Mesdames et messieurs les sénateurs. Quelqu'un mot enfin pour évoquer 3 points qui ont été moins présent dans le débat public mais non. Demeurent pas moins essentiel d'abord la question des systèmes de centralisation des données, qui correspondent à la transposition dans la droite. Français de la directive européenne, PNR, ou à la création d'un fichier issu des. Dossier des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France, si le gouvernement sous. Inscrits aux améliorations juridiques apportées par la commission des lois, il émet néanmoins une réserve sur une modification qui tendrait à figer dans la loi, l'organisation des modalités de consultation des données relatives au PNR maritime mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Autre point : l'établissement d'un cadre juridique pour les opérations de surveillance des communications RCN cette mesure tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016 par laquelle ont été censurées avec un différé au 31 décembre 2017 des dispositions du code de la sécurité intérieure défini. Sans les règles applicables aux opérations de surveillance de ses communications électroniques empruntant la voie exclusivement air tiède. Sur ce point également, le gouvernement a souhaité bien distinguer les techniques qui porte atteinte au secret des correspondances qui seront soumises au cadre de la loi du 24 juillet 2015 et donc contrôlé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de celles qui empruntent la voie hertzienne publique pour lesquelles de telles atteintes n'existe pas, enfin. C'est un point qui a fait débat en commission, nous prévoyons dans l'article 10 le renforcement des possibilités de contrôle aux frontières aux abords des points de passage frontaliers. L'idée de ce dispositif est conforme à la philosophie de l'ensemble du projet de loi. Et il s'agit sans remettre en cause la libre circulation des biens et des personnes, de renforcer nos marges de manoeuvre face à une menace terroriste durant. La commission invoquant jurisprudence européenne a souhaité encadrer davantage ces contrôles dans la durée et dans l'espace, le gouvernement estime toutefois qu'il convient de veiller à ce que ces restrictions ne rendent pas les dispositions prévues inopérant, alors même qu'il est envisagé de lever les contrôles aux frontières intérieures de la France en novembre prochain. Mesdames et messieurs les sénateurs. Un grand conscient qui siégeait sur ces bancs, Victor Hugo écrivait que. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. avec ce projet de loi. Nous augmentons les libertés. Par rapport à l'état d'urgence mais nous assumons pleinement notre responsabilité durant les discussions que nous allons avoir, ne cessant jamais d'avoir à l'esprit et l'une et l'autre de ses préoccupations, les questions dont nous traitons avec cette loi exige en effet un grand sérieux d'infinies précautions, a un sens aigu de ses responsabilités, c'est l'état d'un esprit dans lequel j'dans ces des. c'est l'état d'esprit et je ne doute pas régnera sur vos bancs merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Michel Mercier, rapporteur de la commission des lois. ça rapporte. monsieur Ministre d'État, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission des lois, monsieur le rapporteur de la commission des Affaires étrangères et de la défense nationale, chers collègues, le texte sur lequel le gouvernement nous appelle aujourd'hui à débattre et vous avez eu raison de le dire Monsieur distraire d'État un texte fondamental important comme nous en avons rarement d'aussi important puisqu'il s'agit de faire entrer dans notre droit commun dans d'autres endroits de tous les jours des mesures qui n'ont jamais été. elle était là avec l'état d'urgence, car l'état d'urgence, ces mesures ne peut plus exister, elles n'ont plus de base légale, vous nous proposer de mettre en place un droit qui n'est pas celui de l'état d'urgence et je veux le dire dès le départ, pour que les choses soient claires dans la discussion que nous aurons entre le texte de souvenirs, c'est pas l'état d'urgence qui entrent dans le droit commun. L'état d'urgence permet de prendre des mesures, dont le Champ d'application, notamment, est beaucoup plus large que les 4 mesures essentielles que contient le projet gouvernemental, qui sont ces 4 premières mesures celle de création, le périmètre de protection de fermeture des lieux de culte et je vais changer les noms exprès pour montrer que c'est pas la même chose d'obligation de demeurer dans une commune et de visites domiciliaires ces 4 mesures ne sont pas des mesures qui s'apparente à l'état d'urgence, elles n'ont qu'un seul, l'objectif c'est de prévenir des actions de terrorisme, elles sont donc c'est vrai, des mesures de police administrative et avec ce texte on arrive en quelque sorte à parfaire le droit du terrorisme, que l'on a construit et construction dans laquelle le Sénat a pris toute sa part à droite spécial du terrorisme qui est à la fois droit pénal et un droit administratif du terrorisme, d'ailleurs, si on avait le temps, on pourrait regarder les choses de plus près, on verrait que la force du terrorisme, nous a obligés à dépasser nos catégories juridiques traditionnelles est à rapprocher des notions pénale et des notions administratives plus souvent, peut-être qu'on aurait voulu mais en recherchant l'efficacité

Ils veulent vivre les Français en sécurité et Hugo vie libre et en sécurité, vous êtes dans votre rôle, Monsieur le Ministre d'État lorsque vous nous parlez de la sécurité, le Sénat est dans son rôle lorsqu'il parle de liberté que garantit la constitution le dialogue que nous allons avoir de dialogue franc ou à la loyale, et dans lequel nous allons essayer, si vous le voulez bien de bâtir un vrai équilibre qui est pas seulement valable pour aujourd'hui, mais qui est valable pour la durée entre ces 2 grandes exigences qui sont parfaitement perçus par les Français, même si les exprime pas en termes juridiques, avoir la sécurité nécessaire et disposer des libertés fondamentales, notamment celle d'aller et de venir d'habiter où l'on veut, etc, vous avez rappelé les premières mesures qui elles ont le but prévention du terrorisme, les autres celles qui étaient du PNR et des communications hertziennes et des contrôles aux frontières sont d'application générale, elles ont donc un but un peu différent sur les mesures nouvelles qui vise à prévenir les réactions de terrorisme, je vais passer assez rapidement mais peut-être parfois avec vous parce que votre dans les grands pour démontrer le bien-fondé de vos intentions peut-être parfois aller un peu loin et vous avez peut-être oublié complètement de présenter l'économie de la pensée et de la commission des lois, et vous permettrez que je le fasse pour rétablir l'équilibre qu'à la fin, nous souhaitons trouver. Donc, la première mesure, ce sont des périmètres de sécurité. C'est une mesure que je considère comme tout à fait important au jour dans le droit commun, elle n'existe pas, elle existe par voie judiciaire n'existe peut-être d'urgence mais l'autorité administrative n'a pas ce pouvoir de police administrative. Nous sommes prêts à reconnaître ce pouvoir, l'autorité administrative. Je rappelle que ce périmètre de sécurité permet à l'autorité administrative de sécuriser des événements mais aussi des lieux et j'aurais aimé que dans votre texte vous distinguez mieux événements et lieux, on peut en effet penser que, par exemple, un périmètre de protection permanent autour des 4 piliers de la Tour Eiffel ne pose pas de vrais problèmes, pour ce qui est ailleurs question domicile mais s'il s'agit d'une manifestation place Bellecour, grâce à la politique avançait que vous n'avez en matière de logement social, il y a encore beaucoup de gens qui habitent place Bellecour à Lyon, Monsieur le Ministre n'pas donc il faut qu'ils puissent rentrer chez eux et vous en conviendrez, également, où il y a pas de soldats je mens social place Bellecour pour ceux qui connaissent, mais enfin ça viendra un jour ou l'autre, donc on ne va pas, on ne va pas chicaner sur Suippes, moi je veux donc vous dire que sur ce point, sur ce point très important, nous sommes d'accord pour dire que même si on rentre chez soi. On peut ouvrir son sac. ça ne pose pas de problème, mais on doit pas être empêchés de rentrer chez soi, soi, non, mais je tiens elle dire et qu'il faut trouver un système pour que on puisse rentrer chez soi tous les soirs, voilà.

sur l'est, obligation de résider dans une commune. Je dis pas assignation parce une vraie différence entre l'assignation du droit d'urgence qui est l'obligation de rester dans un appartement et ne pas enfin je dis respect un certain nombre de leur patron pour ne pas être dans une mesure privative de liberté, mais suffisamment pour être dans une mesure restrictive de liberté, il s'agit pas de cela, il s'agit d'obligation de demeurer sur au minimum le territoire d'une commune, c'est un peu la question qui se pose à nous, c'est la question du renouvellement. Il peut pas il y avoir des décisions. Trop longue, sans remise en cause sans rendez-vous de ses obligations de résider aujourd'hui l'obligation de résider à la commune est une mesure de police administrative si nous regardons l'avis du Conseil d'État de 2015. Alors c'est un avis, c'est que le Conseil d'État, certes, mais quand même. Odile Conseil d'État, il dit que la prolongation dans le temps de l'assignation à résidence peu pourrait transformer la mesure restrictive de liberté à mesure privative de liberté, c'est ce qu'il a écrit clairement l'avis du Conseil d'État, et puis si on regarde les décisions je vous communiquerai la vie tout à l'heure monsieur Ministre d'État vois qu'on vous l'a caché, mais je vais il y a ce que vous l'ayez d'un joueur descendrait de La Tribune, je vous signale également que le Conseil constitutionnel dans une décision de 2017 a lui- même pris une position qui n'est pas tout à fait la même mais guère différente puisque le Conseil constitutionnel dispose. S'agissant d'une assignation à résidence, si la prolongation dans le temps ne constitue pas une transformation de la mesure en peine privative de liberté, c'est parce que nous sommes en état d'urgence, il commence sa phrase comme je viens de le dire, or si vous après interprétons cette décision du Conseil constitutionnel, selon la règle de l'effet utile et puis y a aussi le Conseil constitutionnel a pris la peine de préciser que c'est en période d'état d'urgence, il n'y a pas changement de nature de la mesure d'assignation à tout le moins, et se reposerait la question : si nous ne sommes pas dans l'état d'urgence, ce qui sera le cas avec la mesure d'obligation de demeurer il y a donc là un vrai problème pour nous, nous avons pensé qu'il fallait peut-être pas aller au bout de la question : avec ce texte mais qu'il y avait une limite ce qu'il fallait qu'à moment donné, le juge intervienne, nous avions choisi le juge judiciaire pourquoi parce que il nous a pas échappé monsieur le Ministre d'État, Madame la ministre, quelle dans le texte que vous avez magnifiquement rédigé, vous avez un article de et un article IV étant à l'article 2 l'article IV il y a l'article 3 alors dans l'article 2 vous avez décidé que c'était le juge administratif qui décidait de la prolongation au-delà de l'exécution de la mesure contentieux administratif et dans l'article IV, vous avez décidé que c'était le juge judiciaire qui était compétent pour décider de la visite domiciliaire alors dans un 1er temps on s'est aligné sur l'article IV, vous nous dites : c'est pas possible, ça va pas du tout alors. Comme nous, notre but c'est pas choisir juge c'est de mettre un juge pour qu'il y a un équilibre entre la mesure de sécurité et le respect de la liberté, et nous pensons que le meilleur garant de l'équilibre, c'est le juge, hé bien, nous avons choisi de vous proposer de mettre le juge administratif et de copier et de copier le système de l'article 2, c'est-à-dire que, après la première prolongation si l'autorité administrative, continuer à prolonger, il devra avertir, 5 jours avant la personne concernée, qui aura 72 heures pour saisir le juge des référés administratifs que tant que le juge des référés ne se sera pas prononcée, il y aura pas d'exécution d'office et puis ensuite ce sera à chaque fois, le juge ne se prononcera, voilà l'économie et que nous avons choisi, oui à la mesure de sécurité, oui à la protection des libertés avec le s'agissant des identifiants électroniques je suis pas grand spécialiste de la question, je sais, 2 choses, première chose, c'est que vous n'avez pas besoin de ce texte, je vais terminer très vite vous n'avait pas besoin de ce texte, puisque la loi sur le renseignement vous permet de faire cela et que, deuxièmement s'agissant de. identifiant personnel, le Conseil constitutionnel a déclaré : Ce ne stupidité à ce que l'on puisse donner à la. Une distraction de tels renseignements, c'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans la loi de 2016, s'agissant des visites domiciliaires nous aurons l'occasion de revenir sur ce point avec la discussion des amendements sur ce qui concerne les communications hertziennes je laisserai mon collègue, représentant de la commission de la défense s'exprimer sur cette question la connaît mieux que moi sur la question des contrôles aux frontières qui se font en dehors des frontières nous trouverons certainement un accord, je veux redire pour conclure et je vous remercie, Monsieur le Président, mais elle la question que nous traitons sont quand même très importante, je voulais vous dire pour conclure que nous pensons que le texte revu par la commission des lois du Sénat réalise, lui, un vrai équilibre entre la nécessité de protéger les Français et la nécessité d'assurer leur liberté monsieur Ministre d'État, madame la ministre, la commission des lois, dans cette affaire, s'est livré à un vrai travail de responsabilité républicaine, c'est ce même travail déjà le Sénat à faire maintenant. Merci, monsieur le rapporteur de la commission des lois. La parole est à monsieur Michel Boutant, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, madame la ministre. Mesdames, messieurs, chers collègues, la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Ces saisies donc pour avis des articles relatifs aux dispositions touchant au PNR, d'une part, et à ce que l'on nommait l'exception hertzienne, d'autre part, le PNR Passenger Name Record est issu de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, qui proposait son expérimentation jusqu'à la fin de l'année 2017 cet instrument appréciable dans la lutte contre le terrorisme, a enfin été dotés d'un cadre juridique européen via une directive adoptée le 21 avril 2016 tous les États-membres doivent à présent dotés les bases de données PNR existantes ou nouvelles devront impérativement être mises en relation, pour offrir à chaque autorité nationale la capacité de sonder l'ensemble des renseignements collectés, c'est le principal but du passage par le cadre européen quant au système simplifié de PNR maritime proposé par le texte, il sera également fort utile pour lutter contre les formes les plus graves de criminalité à condition une fois encore qu'une coopération efficace entre pays membres permettent de partager les renseignements recueillis, il s'agit pour le moment d'une initiative française la directive européenne PNR se cantonnant au Direct ou donner des circulations aériennes, par ailleurs, je souhaite rappeler que lors du conseil des ministres Justice affaires intérieures informel du 26 janvier dernier la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne avait formé le voeu que les déplacements ferroviaires internationaux soient également enregistrés. La commission approuve en tous les cas, le texte du gouvernement sur le PNR sur l'exception : le le projet de loi de fait assimile Nombre de communication à des techniques existantes dans le droit commun et créent un une 5ème techniques de renseignement pour les communications. Allusivement hertziennes ou ne transitant pas par un par un opérateur au sein d'un réseau privatif ou d'un groupe fermé d'utilisateurs, tels que les. L'échange entre l'talkie-walkie numérique, les transferts de photos d'un portable vers un ordinateur les communications entre une montre connectée et un téléphone mobile ou encore entre Tél d'intérieur, ainsi donc, la grande majorité des interceptions réalisées sur les communications hertziennes seront désormais soumises au régime de droit commun et donc notamment autorisé par le 1er ministre après avis de la scène CTR, ce qui compte aussi. Tu as un Net renforcement du contrôle. à titre résiduel. Il demeure un régime spécifique pour les communications exclusivement RCN sans opérateur et qui sont transmises de façon ouverte, c'est-à-dire qui peuvent être captées et enregistrées par n'importe quel appareil de réception en vente libre, pour peu qu'on soit calé sur la bonne fréquence. C'est ce que font les radioamateurs les cibistes les utilisateurs de tôle qui volcanologique mais aussi des communications radio et moyens tactiques utilisées par les militaires pour ses communications, le projet de loi confirment leur légalité car cette surveillance demeure indispensable dans le cadre en particulier de la défense militaire de la contrat gérance et de la lutte antiterroriste, ils les soumettent à un certain nombre de règles, respect des finalités de la loi sur le renseignement : d'une part et des missions liées à la différence à la défense militaire d'autre part, mais aussi la durée de conservation des données, la destruction des extractions et des transcriptions. Le projet de loi donne à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mission de veiller au respect des champs d'application respectif des techniques de droit commun et du régime spécifique, c'est sur les modalités de son contrôle que portera entre autres la discussion. à l'article 9, car dans l'ensemble, le texte du gouvernement nous convient depuis plusieurs années maintenant, le législateur a effectué de nombreuses années. Ces juridique concernant le contrôle de nos services de renseignements pour nous hisser aux meilleurs standards en termes d'encadrement légal de ses activités au sein des grandes démocraties. Nos partenaires européens nous offre la possibilité de mener à nouveaux frais. Un dialogue exigeant sur la nécessité de trouver le bon équilibre entre les exigences de sécurité publique et les libertés individuelles, le vote de la directive sur le PNR aérien démontre l'efficacité de suite logs et nous encourageons le gouvernement à poursuivre les discussions pour mettre la dernière main à un maillage élargie et complétée du système PNR. Sur le dispositif de surveillance hertzienne, j'insiste sur le fait que la CNC l'organe de contrôle primordial créé par la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015 et qu'il ne s'agit que que de confirmer son rôle à s'assurant de l'effectivité et de l'efficience de l'exécution de ces missions, celle-ci demeure parfaitement proportionnée aux contraintes opérationnelles qui peuvent exister et il ne s'agit il ne s'agit que de garder cohérent son Champ de contrôle pour toutes ces raisons concernant le PNR comme la surveillance des communications hertziennes, la commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi. Merci monsieur Michel Boutant, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères. Eh bien, mes chers collègues, nous allons passer maintenant à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable Madame Éliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ont déposé une motion distribuée sous le numéro 13 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion Madame Assassi pour la motion.

Pour qui est très forte et très émue pour l'ensemble des familles et l'ensemble des victimes qui ont été meurtries. Lors des attentats qui ont frappé notre pays ces dernières années, ces derniers mois. Vous communiste républicain et citoyen. Il a souhaité déposer cette motion tendant à opposer la question préalable afin que soit rejeté l'ensemble de ce projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, le 9 c'est. En 86 il y a 30 ans, donc, la France se doter de sa première législation en matière de lutte antiterroriste, cette loi instituait un régime dérogatoire au droit commun et créer un corps spécialisé de magistrats depuis lors de nombreuses réformes au conduit à la mise en oeuvre d'un régime procédural dérogatoire en matière d'enquête qu'à la création de nouvelles infractions terroristes suite au terrible attentat du 13 novembre 2015 le Conseil des ministres a adopté un décret déclarant l'état d'urgence en à peine 2 ans, l'état d'urgence a été prorogée 6 fois 2 de ces lois de prorogation ayant largement renforcé ces dispositions en parallèle ont été promulguées le 24 juillet 2015 la loi sur le renseignement et le 3 juin 2016 la loi renforçant la lutte contre le Crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité des garanties de la procédure pénale, nous nous sommes opposés à l'ensemble de ces textes constituant un arsenal non seulement dangereuse pour l'équilibre de notre démocratie, mais surtout inefficace pour en forcer notre sécurité publique comme on témoigne hélas le terrible attentat qui a meurtri la ville de Nice il y a un an, la présente réforme s'inscrit dans la même Villiers digne et illustrent des choix politiques de ces 15 dernières années, des événements, donc de nature exceptionnelle sont utilisés pour justifier la construction d'un droit d'exception, à ceci près que ce projet de loi portant lui le coup d'après, prétendant conditionné la levée de l'état d'urgence à l'adoption de ce texte, le gouvernement introduit en réalité les mesures même de l'état d'urgence dans notre droit commun dans une version prétendument en édulcoré, mais sans la moindre garantie valable aux personnalités du réseau, état d'urgence anti-terrorisme qu'il recevait le 3 juillet dernier, le chef de l'État a affirmé tranquillement qu'il s'agissait de la première et de la dernière loi antiterroriste de son quinquennat. évidemment, évidemment, puisque à inscrire l'état d'urgence dans notre droit commun mettra effectivement enfin au renouvellement incessant de l'état d'urgence, je vous l'ai déjà dit lors de mon intervention concernant la 6ème prorogation de l'état d'urgence, il y a 15 jours, ici même, des voix de plus en plus forte s'élève contre son contenu renoncer à l'état d'urgence nécessaire mais n'autorise certainement pas en faire notre droit commun comme l'écrit Mireille Delmas-Marty dans une lettre ouverte au président de la République et comment ne pas citer ici ce texte signé par plus de 500 universités et universitaires, chercheurs, juristes, Politis, sociologue, qui affirme que les mesures contenues dans ce projet de loi sont dangereuses et font peser des menaces sur notre état de droit, lors de son intervention devant le Parlement réuni en Congrès le 3 juillet dernier, Emmanuel Macron, affirmait le code pénal, telle qu'il ait les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonnée, bien organisés, nous permettent d'anéantir nos adversaires, donnés en revanche à l'administration des pouvoirs limités sur la vie des personnes sans aucune discrimination n'a aucun sens ni en termes de principes, ni en terme d'efficacité, voudrais dire que nous sommes d'accord avec lui et là tout ce qu'il nous propose aujourd'hui avec untel texte est l'exact opposé de ce qu'il semblait dénoncer il y a quelques jours, jours, monsieur ou légitimer l'accroissement des pouvoirs de l'administratif par un soi-disant manque d'anticipation judiciaire, pourtant il est faux de prétendre que seul l'état d'urgence sous l'action de police administrative serait en capacité d'intervenir pour prévenir un attentat et nous les outils relevant du judiciaire, tous les jours, les procureurs et juges d'instruction antiterroristes dirige des enquêtes visant des personnes pour les projets qu'elles élaborent et non qu'elles ont commis à titre des clans, les perquisitions administratives menées en nombre n'ont abouti qu'à l'ouverture de 30 procédures en matière antiterroriste alors qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait pu intervenir dans un CAT intégralement judiciaire sachant qu'entre novembre 2015 et novembre 2016 2016 que seuls 20 enquête étaient imputables à l'état d'urgence 170 procédures d'information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Paris dans un cadre normal, monsieur Macron écrivait dans son livre de campagne révolution pourquoi il souhaitait sortir de l'état d'urgence, pourquoi alors proposer un untel texte si cela n'est pas pure démagogie, serait-ce pour utiliser la peur légitime de nos concitoyens, peut-être que la raison est plus profonde, je le crains, ce texte est idéologique, au-delà de son pragmatisme apparent, il porte en lui de nombreuses questions, celle des répressions administrative et des pouvoirs grandissants des forces de leur toujours plus exempt du contrôle judiciaire, celle des migrations et des contrôles aux frontières et enfin celle des inégalités grandissantes entre les citoyens face à des jeunes qui sont tangents si vous défoncer leur porte à 4 heures du matin que vous les assigne à résidence ou ici à commune pendant 3 mois, ce qui a pour conséquence que certains perdent leur boulot, expliquez-moi en quoi ils sont moins dangereux, ensuite tout homme sensé comprend qu'on attise le feu avec de telles méthodes ont à n'importe qui n'apporte que comment ce n'est pas moi qui dit cela, c'est le désormais très médiatique, Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste face à ces dérives qui ne sont plus à prouver, il faut désormais avoir le courage de passer d'une logique de peur irrationnelle qui justifie une logique de guerre à une logique de paix pour lutter contre le terrorisme, il y a certainement pas de loi instaurant un risque 0, mais peut-être qu'il faudrait sérieusement commencer à amorcer une réflexion qui est double : d'abord sur le plan international pour combattre ses ennemis, il faut les connaître, il faut expliquer, contrairement à ce que certains ont pu dire remonter aux origines géopolitique rappeler les responsabilités bien réelle des puissances occidentales cette guerre destructrice en Irak et en Afghanistan, le non-sens de l'intervention en Libye, il faut enfin dénoncé le rôle trouble des puissances régionales comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar le terrorisme se nourrit de la guerre du pétrole et du trafic d'armes, nous le répétons depuis le congrès de Versailles du 16 novembre 2015 la coalition internationale est au coeur du problème, il faut rapidement repenser les choses et cesser d'agir en ordre dispersé une large coalition internationale sous mandat de l'ONU doit être mis en place avec la nécessité au-delà du combat contre Daech l'ambition de reconstruire ces régions permettent d'établir une paix durable et ainsi le retour de milliers de réfugiés sans cette perspective pas d'issue au terrorisme, deuxièmement, sur le plan national, il faut refonder le vivre-ensemble en bannissant le culte de l'argent, si chère au chef de l'État, qui instaure en vertu, le statut de milliardaires faire miroiter la fortune à ceux qui ne pourront latin fenêtre la colère, désespoir pouvant aller jusqu'à des dérives extrêmes, la culture et l'éducation sont d'abord le fruit d'un échange de Liens, de partage, de social d'homme, cela n'en quelque sorte, pas de prix, si ce n'est celui des politiques publiques et des moyens alloués pour rémunérer nos acteurs sociaux orienter les Budgets vers ce qui n'est pas visible tout de suite mais indispensable pour l'avenir, ces éducateurs ses assistantes sociales, conseillers en insertion et probation tous ces métiers essentiels : l'emploi doit être l'objectif primordial, les missions de service public de l'État elles-mêmes sont aujourd'hui parfois dévoyée au service de la lutte contre le terrorisme, comme en témoigne la tribune parue dans Mediapart de plusieurs agents publics, fonctionnaires de l'État, au quotidien, nous accomplissons d'ambition respective du mieux possible, malgré des moyens suffisants, des conditions de plus en plus dégradé, écrivent-t-ils, alors même qu'elle nous semble essentiel et complémentaire, l'éducation, la culture, l'insertion, la justice, la prévention et la sécurité, la recherche, la santé, la douane sont toujours dévoyé pour raisons de sécurité, il y a des fins de renseignements pour la lutte contre le terrorisme les policiers subissent la politique du chiffre exacerbée avec l'état d'urgence une politique axée sur le tout sécuritaire, or, leur rôle est aussi d'être au plus près de la population pour prévenir et lutter contre les crimes, les délits mais aussi toute forme de radicalisation en récupérant les renseignements à la source comme nous réclamons en urgence un débat public sur les politiques à mener pour lutter contre le terrorisme, car après cet ancrage de l'état d'urgence dans notre droit commun, quelle sera la prochaine étape, l'état de siège, a déclaré la guerre matériel viendra-t-elle prendre nos rues, notre responsabilité est donc grande a jeté en pâture, nos libertés publiques, notre pays n'en sortira pas grandie et notre sécurité collective de s'verra aucunement renforcer ce que veulent nos ennemis obscurantiste, c'est le recul de nos démocraties, c'est mettre à mal nos droits et libertés publiques pour revenir à cet état primitif de la loi du plus fort, la France doit se ressaisir et non pas et ne pas tomber dans, dans, dans un despotisme fugitive d'où elle doit être fidèle aux idéaux qu'elle porte depuis le siècle des Lumières en renonçant au chemin de la surenchère sécuritaire qui n'aura pour seul fruit que la fracturation de notre société, merci. Merci madame la présidente. Je n'ai pas d'intervenants contre la monsieur donc je vais donner la parole pour l'avis de la Commission et ensuite monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, monsieur le rapporteur de la commission des lois. Merci beaucoup monsieur le président, madame la présidente, je collègues la motion que vient soutenir Madame Assassi me semble inadapté au texte que nous avons préparé en effet comme nous savons tous la menace terroriste perdure à haut niveau dans notre pays, le texte qui nous est présentée aujourd'hui nous semble tenir compte de cette. Menaces nous faisons crédit au gouvernement du fait qu'il a les moyens d'apprécier l'importance de cette menace, grâce aux services de renseignement et que s'il présente ce texte ce qu'il y a un risque certain pour nous, notre rôle est de concilier. La protection qui est dû aux Français en fonction de ce risque avec les libertés traditionnelles auxquelles nous sommes attachés, la commission a travaillé dans ce sens, pense être arrivé à d'équilibre qui est bon et si le Sénat, on pourra encore l'améliorer. Au cours des discussions qui sont, qui vont qui vont avoir lieu, non pour lequel je ne peux donner que l'avis défavorable à la motion présentée par Madame la Présidente, assassiné et je le regrette. Merci, monsieur le rapporteur de la commission, monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement. Quelques mots de de réponse à madame la présidente du groupe communiste, qui s'est tout de même un peu éloigné du sujet. Si l'on regarde les rapports entre ce qu'est l'état d'urgence et ce qu'est le texte que nous vous proposons, on s'aperçoit que le cadre juridique des mesures que nous vous proposons évidemment beaucoup plus protecteur d'abord 1ère différence. Il vise simplement le terrorisme et non pas le maintien de l'ordre public, ce qui je pense pour vous fera une différence relativement appréciable, ensuite il est beaucoup plus encadré de manière juridique en permettant de garantir les droits individuels, le seuil de déclenchement de la mesure est lui aussi beaucoup plus élevé, puisque j'ai lu tout à l'heure, un certain nombre de textes, il s'agit d'une menace d'une particulière gravité et donc nous n'utiliserons pas ce texte et préfet, le ministre de l'Intérieur qui peuvent être concernés n'utiliseront évidemment pas ce texte, de manière comment dirais je sortis des problématiques qui nous concerne, aujourd'hui, je vous rappelle d'ailleurs que même avec l'état d'urgence, un certain nombre de mesures avaient été avec beaucoup de précaution, parce que nous sommes dans un état d'droit et si la mesure avait été importante au départ parce que peut-être pas vous, madame la présidente, mais nous, nous avions été je parlais d'effet de sidération pour les terroristes, mais les faits avaient été réciproque, nous avions été sidéré que sur notre territoire sur le sol français des attentats comme celui de Charlie-Hebdo, comme celui du Bataclan puisse avoir lieu, chaque fois qu'un n'attentat à nouveau se produisait, nous disions non ce n'est pas possible sur notre sol nous avons pris beaucoup de mesures, c'est parce qu'à chaque fois, nous étions précédé d'une certaine manière, par des terroristes qui chaque fois monté d'un cran et c'est pour cela qu'il y a eu autant de nécessité de prendre des législations et de pouvoir riposter si aujourd'hui, nous avons réussi à maîtriser ce risque qui reste important, tous les jours, c'est largement parce que depuis ces années à la fois le gouvernement et le Parlement ont pris de telles mesures et nous ont donné les moyens légaux de pouvoir riposter aux terroristes sur la suite, nul ne vous dit que nous considérons que la société est parfaite. Et que tout va bien dans notre pays, nous voyons comme vous les 3 millions 500 1000 chômeurs peut-être simplement n'apportons-nous pas la même réponse exactement et peut-être ne faisons-nous pas la même analyse de ce qui a provoqué dans notre pays, ce chômage de masse, mais comme vous le savez, c'est un autre débat sur le fait qu'un certain nombre de quartiers de communes soit aujourd'hui paupérisé ait tendance à se ghettoïser je vais vous dire, je partage avec vous la même analyse et donc dans mon agglomération nous essayons de faire lorsque j'étais maire et président de faire en sorte que nous remettions de la mixité sociale dans la ville, et lorsque je vois quelquefois la banlieue parisienne, je me dis qu'effectivement avoir une séparation totale entre des communes qui sont effectivement très et d'autres qui ont une puissance certaine cela ne favorise pas la compréhension entre les uns et les autres, donc oui, nous comprenons les maux dont souffre la société française, le fait que notre fracture sociale est aujourd'hui largement une fracture spatiale et donc il convient de la résorber, mais c'est évidemment d'autre politique que celle menée par le ministre de l'Intérieur et c'est donc dans un ensemble qu'il faut voir l'action du gouvernement mais dire que nous n'aurions pas besoin actuellement et, connaissant ce qu'un ministre de l'Intérieur peut connaître des mesures que nous vous proposons non madame, je me permettrai de ne pas être d'accord avec vous et si vous voulez bien avec la Commission, nous allons justement chercher cet équilibre entre sécurité est liberté.

la question préalable, on peut en comprendre le sens, le texte effectivement nous inquiète par certaines mesures, et on s'en expliquera tout à l'heure et on l'a déjà dit à propos du renouvellement de l'état d'urgence, néanmoins, nous souhaitons d'abord que le débat puisse avoir lieu et d'autre part, nous pensons que dans ce texte il y a des mesures nécessaires, celle notamment car rappeler le rapporteur pour avis Michel Boutant, qui sont des adaptations d'une part, une directive européenne, d'autre part à des décisions du Conseil constitutionnel et puis il y a aussi dans l'article 1er des choses qui nous intéressent, notre groupe votera contre la question préalable. tendant à opposer la question préalable, bien sûr, je rappelle que cette motion entraînerait le rejet que l'adoption pardon entraînerait le rejet du projet de loi. Alors qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur François-Noël Buffet. Pour le groupe, les républicains et pour 10 minutes.

Merci à mes yeux, nous avons créé les conditions qui rendent possible une sortie de l'état d'urgence sans nous affaiblir ni demeurer impuissants face à la menace du terrorisme, tels étaient les mots de Jean-Jacques Urvoas devant les représentants des juridictions administratives en mars dernier. Qui est-ce qui a changé depuis mars dernier pour que vous nous proposez un nouveau, ou plutôt devrais-je dit oh, devrait-on dire à un énième texte pour renforcer la sécurité intérieure et lutter contre le terrorisme, la réponse la plus évidente serait l'élection d'un nouveau président de la République, malgré ses écrits de novembre 2016, expliquant que nous avons tous l'appareil législatif permettant de répondant dans la durée à la situation qui est la nôtre, certes, l'élection du président de la République est un élément structurant de nos institutions, mais insuffisant pour justifier à lui seul une nouvelle législation de droit commun intégrant des dispositions que certains ont dénommé la pilule empoisonnée. Nous trompons pas de cibles, mes chers collègues, la pilule empoisonnée le terrorisme qui sévit sur notre territoire en Europe et au-delà, au nom de valeurs atroce et d'expédition sanglante, la situation est grave et la menace élevé, vous nous l'avez rappelé monsieur le Ministre d'État à la nature de l'intimidation a évolué, la menace n'est plus seulement exogènes, elle est aussi en 2 semaines, voilà ce qui a changé depuis le mois de mars dernier, notamment une alternative s'offrent aujourd'hui à nous après avoir posé pour la 6ème fois l'état d'urgence qu'au 1er novembre prochain, soit il faut choisir de légiférer sur des dispositions que notre commission des lois a rendu exceptionnel au sens lexical de termes évitant toute dérive pernicieuse ou bien envisager de proroger de nouveau l'état d'urgence dans 3 mois, mais il n'est pas question pour nous de nous accoutumer à l'état d'urgence ce régime exceptionnel relevant de l'autorité administrative, même si l'extrémisme islamiste continue d'exister dans notre environnement quotidien, nous tenons ardemment à maintenir l'équilibre précieux de nos institutions démocrate démocratique issu des Lumières, fondée sur la pensée de Montesquieu, qui écrivait que pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut. Pour qu'on ne puisse habile pouvoir pardon, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir, nous tenons à ce que le pouvoir législatif que nous incarnons puissent exercer la plénitude de ses compétences constitutionnelles et que l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, jouent un rôle protecteur, comme le rappelle notre collègue François Pilet dans un, dans l'ouvrage qu'il vient de publier notre rapporteur nous a très récemment très justement interrogé, pardon, sur la nécessité de rechercher l'existence d'autres moyens pour atteindre les objectifs assignés en assurant le respect des garanties de notre état de droit, comme l'aime d'ailleurs à le rappeler notre président du Sénat, la mission historique de notre assemblée et d'être le protecteur des libertés publiques le rôle fondamental du Sénat et plus largement celui du Parlement dans la défense et le contrôle des libertés devait retrouver une réalité efficace que le Sénat avait su imposer dans l'état d'urgence, il faut donc remercier le président de la Commission et le rapporteur d'avoir habilement imposer l'expérimentation de 2 mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles que sont la surveillance individuelle et la visite du domicile erronément appelé assignation et perquisitions alors oui, la situation est ambivalente : le gouvernement a imaginé qu'il suffirait d'inscrire dans le droit commun, un certain nombre de pouvoirs supplémentaires qui seraient exercées par l'autorité administrative avec l'autorisation du juge des libertés et pourtant, comme vous en avait averti le président bas dès la semaine dernière, je le cite, ces dispositions ne constitue pas par rapport à l'ensemble des dispositions déjà prises un saut décisif permettant d'améliorer notre arsenal juridique, vous ne l'avez exprimé lors de votre audition, Monsieur le Ministre, le gouvernement souhaite apporter des garanties à la sécurité des Français, hé bien, nous aussi, nous avons au cours des 2 dernières années déjà inscrit dans le droit commun de très nombreuses mesures permettant de répondre au manque manifeste de moyens et de procédures, le Sénat et d'ailleurs à l'origine d'un certain nombre d'entre elles, je pense notamment à l'élargissement des facultés de recours aux perquisitions nocturnes à la meilleure prise en charge de la radicalisation par les juges en étendant la possibilité de prescrire des actions de prise en charge d'indications de la radicalisation dans le cas d'un sursis avec mise à l'épreuve, comme nous l'a rappelé notre collègue Catherine Tremblay en présentant ce rapport d'information sur les 2 2 des embrigadement je pense aussi à la création de 2 nouveaux délits terroristes que sont le délit d'entrave au blocage des sites incitant à la commission d'actes de terrorisme, le délit de consultation habituelle de tels sites mais aussi à la possibilité de rendre applicable la période de sûreté incompressible de 30 ans au lieu de 22 ans actuellement pour les criminels terroristes condamnés à la perpétuité et je dirais enfin que nous avons réussi à obtenir un régime procédural spécifique permettant d'empêcher l'accès des personnes condamnées pour terrorisme à la libération conditionnelle, ces mesures, personne ne peut le négliger sont efficace judiciairement, comme nous l'a d'ailleurs expliqué le président de la République lors du congrès de Versailles, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui extrêmement vigilants aux propositions que le gouvernement nous formule il n'est pas question d'accepter un état d'urgence dégradé qui serait introduit dans le droit commun, je voudrais donc de saluer notre rapporteur Michel merci pour, à son habitude, détecter toute mesure attentatoire aux libertés fondamentales qui ne seraient pas conformes à notre constitution les Français demandent aux pouvoirs publics de les protéger de leur apporter la sécurité nécessaire pour vivre en liberté, il est de notre devoir de leur répondre en les éclairant vous nous avez rassurés sur un certain nombre d'interrogations, ce qui me permet de dire que plusieurs dispositions de votre texte ne soulève pas de difficultés particulières pour notre groupe, qu'il s'agisse du renforcement du contrôle aux frontières, des opérations de surveillance des communications hertziennes de la transposition de la directive européenne sur le PNR que nous appelons de nos voeux depuis des années, ou encore de la fermeture des lieux de culte aux seules fins de prévenir des actes terroristes, car le coeur de notre débat porte bien sur la prévention des actes terroristes comme finalité de chacune des mesures envisagées. L'analyse des procédures en matière de terrorisme montre d'ailleurs que cette matière fonctionne de manière optimale lorsque les actions sont engagées en coopération entre les services de la entretien le meilleur exemple étant celui, selon lui, celui de Paris, où le préfet et le procureur coopèrent de manière permanente, permettant de judiciariser, une grande partie des dossiers, c'est pourquoi il est fondamental pour nous que toutes ces nouvelles procédures administratives de droit commun implique la justice judiciaire garante des libertés individuelles, nous nous satisfaisons donc pleinement des avancées proposées par la commission des lois, en la matière, essentiellement dans le dispositif des mesures de surveillance individuelle en imposant que celle-ci ne puisse être prononcée que pour une durée limitée et renouvelé sur autorisation d'un juge afin qu'elles ne puissent devenir des mesures privatives de liberté, ce qui les détourneraient de leur objet, une garantie supplémentaire au dispositif des visites de domiciles et saisi a été importé en prévoyant l'accord Express du juge pour retenir pendant le temps des opérations toute personne à l'égard de laquelle la visite a été autorisé cette implication de l'autorité judiciaire peut rassurer nos concitoyens et démontre que nous sortons réellement du régime juridique de l'état d'urgence à caractère purement administratif, il n'est donc pas question pour nous de faire perdurer comme j'ai pu le lire, le régime d'exception que l'état d'urgence, il n'est pas non plus question de marginaliser l'autorité judiciaire au profit de l'autorité administrative, au détriment des droits du justiciable, notre démarche s'inscrit en faux par rapport à ses présupposés qui laissent penser à nos concitoyens que nous ferions reculer les libertés par le glissement d'un contrôle des mesures contraignantes attentatoire à ses libertés, effectuée par le juge judiciaire vers un contrôle la postériori effectuée par le juge administratif pour conclure je souhaiterai ajouter que nous devons nous ne devons pas oublier mes chers collègues, je me tourne particulièrement vers Alain Marc et Philippe Dominati, nos 2 rapporteurs budgétaires en charge du programme de sécurité que les dispositifs que nous allons voter aujourd'hui nécessiteront encore plus d'efforts de la part de l'État pour que chaque maillon de la chaîne de sécurité puis judiciaire puisse assumer nos décisions le soupçon ne constitue pas pour nous un motif légitime d'application des mesures restrictives de liberté mais la lutte contre le terrorisme est en revanche un motif suffisant pour nous battre collectivement pour la sécurité de nos concitoyens et la liberté de notre pays, merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur David Rachline pour 3 minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, pourquoi une telle logorrhée législative sur le sujet du terrorisme, la menace a-t-elle si profondément changé en seulement 4 années pour que nous ayons dû voter 8 textes non, en réalité, je crois que les gouvernements ont pris la mauvaise habitude de faire voter des textes pour fuir leurs responsabilités, de faire voter des textes pour faire croire aux Français qu'ils agissent de faire voter des textes plutôt que de mettre en oeuvre une politique de sécurité fermes et courageuses, il faut dire que les gouvernements successifs sont largement responsables de la difficile situation sécuritaire que nous vivons, responsable d'avoir laissé se développer le communautarisme en particulier le communautarisme islamiste responsable d'avoir laissé les portes de la maison France, grande ouverte avec les accords de Schengen responsable d'avoir permis quand ce n'est pas encourager une immigration de masse s'installer en France y compris illégalement d'ailleurs responsable d'avoir suivi des politiques étrangères désastreuse, par exemple, en intervenant en Libye ou en saluant avec des pays soutenant les islamistes radicaux responsables d'avoir mené une politique pénale des plus laxiste, faisant naître un sentiment d'impunité, bref, responsable d'avoir laissé terreau antifrançais prospérer sur notre sol dans lequel l'islamisme radical racines du terrorisme, a pu se développer alors à défaut de mener réellement le combat, vous nous faites voter des textes, permettez-moi de croire qu'un contrôle strict à la frontière franco-belge des terroristes qui ont lâchement attaqué la France un soir du 13 novembre aurait été plus efficace que d'ajouter quelques pages au code pénal, cela fait presque 2 ans que nous sommes sous le régime de l'état d'urgence, et bon nombre de mesures permises par cet état d'exception n'ont pas été pris, je pense par exemple à la fermeture immédiate de la centaine de mosquées radicales en outre un certain nombre de mesures efficaces pour limiter le risque terroriste ne sont pas mises en oeuvre et pourtant vous n'êtes nullement limitée par le droit existant, expulsion des étrangers fichés S condamnation des Français Coupat d'Intelligence avec l'ennemi, plan de désarmement des banlieues mais aussi renforcement des moyens humains et techniques des forces de sécurité, mesure qui, si j'ai bien suivi l'actualité ne sont pas vraiment d'actualité précisément c'est ainsi d'ailleurs qu'à Fréjus comme je crois dans beaucoup d'autres villes, la police ne pourra plus faire appel à ces réservistes, il faut dire que pour vous, la sécurité des Français passe après le respect de la règle des 3 pourcent imposés imposés par l'Union européenne, alors oui, nous pensons que l'arsenal législatif est déjà bien suffisant pour commencer vraiment à mener une véritable lutte contre le terrorisme islamiste qui menace notre pays mais pour ça il faut du courage politique qui ne se limite pas à dire je suis le chef, faites-moi confiance, la confiance, ça se mérite, et pour cela, plutôt que des paroles, on attend des actes et si j'en crois le grand nombre d'actes délictueux commis à l'occasion du 14 juillet le faible nombre d'interpellations, les délinquants de en tout genre ont de beaux jours devant eux, or l'histoire tragique de ces dernières années, nous apprend que certains d'entre eux seront les terroristes de demain, nous ne voterons donc pas ce texte pour 3 raisons : le droit actuel permet déjà de lutter contre le terrorisme, encore faudrait-il avoir le courage et la volonté de l'utiliser, ce texte ne supprime pas le principe de l'état d'urgence que le gouvernement peut donc à tout moment rétablir en cas de menace imminente et de mettre à l'heure à Laurent, 9 des mesures d'exception et enfin de femmes trop attachés à la liberté pour voir cette valeur, une nouvelle fois grignoter alors, mes chers collègues, faisons plutôt notre cette belle devise du lieutenant Tom Morel, le héros des Glières vive vivre libre ou mourir.

Monsieur le président. Monsieur et madame le ministre et chers collègues, nous allons à nouveau légiférer, nous allons faire la loi et donc au-delà des attitudes et une formule d'éloquence, regardons de près pourquoi il faut de nouveau légiférer et sur quoi nous allons nous prononcer pourquoi. Le péril. La menace pour la sécurité de nos concitoyens, du fait de mouvement terroristes persistant. Va se poursuivre. Sans entrer dans un. Paysage trop large, nous savons bien. Que le changement de situation au Proche-Orient, la réduction progressive du capacités opérationnelles. De Daech n'est pas à court terme en tout cas un facteur d'allégement de la menace sur notre sol sur notre population. Donc, voilà pourquoi il faut légiférer, le chef de l'État a indiqué, ce que nous souhaitions tous et déjà avant le 14 juillet 2016. 2 présidents a donc souhaité que l'on mette fin à l'état d'exception que constitue l'état d'urgence, de ce fait, il faut regarder de façon précise. Texte à la main, quelles sont les mesures de limitation du risque de prévention du risque dont nous avons besoin, en réalité, si nous voulons être précis, factuel Respectons le contenu de la loi sur laquelle nous allons légiférer, il y a 4 dispositions de sont des dispositions de police administrative que nous connaissons en permanence, c'est d'une part, les zones de sécurité écoutez au cours de la semaine passée dans combien de nos communes, avons-nous dû organiser le 14 juillet avec des contrôles accrus par rapport à ceux des périodes antérieures avec un support légal un peu fragile, organiser des limitations d'accès aux zones de spectacles et des fouilles de sacs. Sur instruction de nos préfets avec un petit risque d'irrégularités qui peut prétendre que c'est une atteinte aux libertés. Qui ne voit que c'est en réalité le moyen de concilier la liberté et l'initiative culturelle festives, la vie sociale avec l'exigence de la prévention du terrorisme, de même la fermeture des lieux de culte. Je rappelle pour ceux qui ont quelques appétence historique que la loi de 1905. Prévoit depuis son origine, dans son article 35 des sanctions pénales contre l'atteinte à l'ordre public, prononcée dans le dans l'exercice du culte en revanche la sanction administrative, la possibilité d'interrompre, elle existe dans la jurisprudence du Conseil d'État depuis l'arrêt Benjamin de 1933 simplement par rapport au droit commun de la police administrative, le dispositif qui est proposé ici présente l'Avantage d'agir dans un moment dans un pas de temps le plus réduit possible et en même temps d'assurer les droits de la défense par rapport à l'association culturelle ou à l'officiant qui serait mise en cause. En réalité, il y a 2 mesures et 2 seulement, qui porte une limitation aux libertés individuelles et une imitation et organisé, c'est d'une part, la possibilité de visite avec saisie par décision administrative et d'autre part, ce que j'appellerais une limitation individuelle de mouvements et de contact qui sont l'une et l'autre différente dans la substance de la perquisition administrative d'une part et de l'assignation à résidence, d'autres pas, dans les 2 cas. Nous voyons bien que ce sont des outils indispensables à la poursuite d'une activité de renseignement qui est, je dirais, le carburant qui est l'énergie nécessaire à la lutte effective contre le terrorisme, la visite est saisie, elle est nécessaire, comme l'a dit le ministre pour repérer des situations dans lesquelles il n'y a pas la capacité d'engager une poursuite judiciaire, parce qu'elle souhaite infructueuse et que l'intéressé serait blanchi. Et pourtant, de mener une action de prévention en temps utile pour empêcher la constitution d'un véritable préparatifs terroristes ceci : c'est une mesure qui a un caractère intrusif et donc le gouvernement et la commission sont d'accord pour prévoir que cette mesure soit précédé l'autorisation d'un magistrat judiciaire du juge de la liberté et des détentions où est donc l'atteinte à la liberté individuelle, on est bien dans une procédure qui assure la protection, la vérification de l'adéquation de la mesure avec la nécessité de la sécurité du public. Et quant à la limitation du mouvement là c'est typiquement une mesure certes nouvelle de police administrative mais qui représente bien une mesure restrictive de liberté au sens où l'entend le Conseil constitutionnel, donc il doivent être prises par l'administration qui ne peut pas être prise par un juge, puisque par définition, cela supposerait qu'une procédure judiciaire complète est eu lieu alors qu'il y a éventuellement urgence donc cette limitation de mouvement et de contact, elle est organisée dans le projet de loi et là encore il y a après le dialogue qui s'est poursuivi ces derniers jours : accord entre le gouvernement et la commission pour que des conditions d'encadrement légal et procédurales strictes accompagnent cette mesure donc évite qu'elle ne soit détournée qu'elles ne soient trop généraliser et parmi ceux qui font des proclamations hostiles à ce projet de loi, je n'en vois aucun qui conteste sur le fond, les mesures.

donc quand on regarde ce que sont les critères de l'État de droit, ce projet de loi les remplit et satisfait, c'est un projet conforme à l'état droit et d'ailleurs forcément ceux qui le contestent le porteront devant le Conseil constitutionnel, sous une forme ou sous une autre, et ce sera vérifié mais je constate que les critiques qui portent que sont contre ce projet de loi sont décrits tire sont des critiques d'attitude d'expression et qui ne porte pas sur le contenu de ce projet de loi, il me semble que le Sénat fait son travail, répondant au gouvernement sur les objectifs de ce projet de loi et en fixant un cadre mais en menant notre travail de législateur, c'est toujours un peu la discussion d'Antigone, nous prions et rappelons-nous que quand Créon prenait la responsabilité que raconte que Nahr ce Sophocle la cité était menacée, donc je crois que nous sommes toujours dans cette situation et que nous pouvons nous placer dans la position de crayon et respecter la philosophie des Lumières. Merci monsieur Alain Richard, la parole est à monsieur Christian Favier.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est N-ième Projet de loi renforçant la lutte antiterroriste, Marc, vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre d'État, un tournant important, il propose d'inscrire dans notre droit commun Les principales mesures autorisées à titre exceptionnel dans le cadre de l'état d'urgence au détriment d'autres équilibres démocratique entre sécurité et liberté en présentant notre motion de procédure ma collègue, il y a là ça si vous a déjà énoncé le point de vue de notre groupe sur les problématiques que soulève ce texte et je vais pour ma part donc me concentrer davantage sur les mesures proposées en elle-même et sur les modifications apportées par la commission des lois, en assistant aux débats en commission des lois, la semaine dernière, j'ai d'abord été assez étonné des remarques de mes collègues et notamment chez les républicains, qui ont apporté plusieurs nuances à leur propos, d'ordinaire plus tranché plus guerrier au sujet de la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, monsieur nous a même enjoint de réfléchir au mode Benjamin Franklin, je cite, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les 2 quelle lucidité, mon cher collègue, par les réflexions de nos collègues socialistes qui semble découvrir un texte jugé aujourd'hui particulièrement dangereuse, estime opportun par exemple de supprimer les articles 3 et 4 de la commission et en allant jusqu'à invoquer la Cour européenne des droits de l'homme qui s'opposera sûrement à cette instauration de l'état d'urgence dans le droit commun, il faut pourtant rappeler que l'entaille dans le droit commun a été ouverte par le gouvernement de Manuel Valls avec sa loi du 3 juin 2016, que le président Macron donc aujourd'hui se contente de parachever comme à son habitude, la commission des lois, elle s'est ainsi posé en défenseur des libertés publiques, certes toutes les mises en garde, soulevée par notre rapporteur sont bien légitimes et ne peuvent que recueillir notre assentiment mais là où le bât blesse, c'est que le rapporteur, comme le président et la majorité d'entre commission en reste aux considérations de mise en garde. Oh prévention aux prétendues garanties comme si les mesures qui nous était proposé était inédite, jamais mises en oeuvre et comme et, comme si aucune dérive n'avait jamais été noté, c'est là notre rapporteur a amendé le texte afin de, je cite : rechercher un meilleur équilibre entre la nécessité d'assurer la sécurité et l'ordre public et celle de protéger les droits et libertés constitutionnellement garanti ainsi sur l'article 1er, la Commission a admis l'instauration de périmètres de protection sur arrêté préfectoral mais on a timidement circonscrit le l'usage pourtant il reste toujours à craindre que les mesures proposées permettent une application discriminatoire dès lors que les fouilles rocker aucune base objective, les agents identifiés comme pouvant intervenir pour mettre en oeuvre ces mesures sur ce suscite notre plus vive opposition je pense en particulier l'usage d'agents de sécurité privées nous y reviendront sûrement dans la discussion, enfin il est à craindre que ce type de mesure laisse place à une utilisation autre que celles définies initialement tels que l'étouffement ou la répression de contestation politique sur la voie publique, hélas, nous en avons d'ailleurs déjà eu plusieurs fois l'exemple ces derniers mois, concernant les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance contenue à l'article 3, certes, la commission des lois, aligner les conditions de pointage sur celle prévue par le contrôle administratif, de retour sur le territoire et a placé le renouvellement de ces mesures sous contrôle total de l'autorité judiciaire, elle a également supprimer l'obligation de déclaration des numéros d'abonnement et identifiant de communications électroniques mais il n'empêche que cet article n'en croit pas moins dangereux droit commun les mesures d'assignation administrative l'article IV transcrit le régime des perquisitions de l'état d'urgence en mettant en place un régime juridique visites domiciliaires et de et dessaisi la différence réside pour le gouvernement, dans l'introduction d'une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de Paris communiqué au parquet de Paris, hélas, cela ne constitue en rien une garantie soumis à la pression et contraint de travailler dans l'urgence et en petit nombre, ces magistrats seront difficilement évidemment refusé ce genre d'intervention, en outre, le texte ne prévoit pas quelles pièces seront versés au dossier qui lui sera soumis et l'appréciation de l'autorité administrative résultera donc des éléments fournis par les services de renseignement pour ces 2 articles du projet de loi qui reprennent dans notre roi commun de dispositions emblématiques de l'état d'urgence, la commission des lois à l'initiative de son rapporteur a limité dans le temps, donc jusqu'au 31 décembre 2021, leur application dans une sorte de clause, on pourrait dire d'autodestruction,

pour notre part, nous ne pouvons accepter pour quelques période que ce soit que ce genre de mesures viennent contaminer notre droit et remettre en cause nos libertés publiques, c'est la raison qui nous conduira à vous proposer plusieurs amendements de suppression, ce qui est à l'oeuvre, on le voit, c'est donc un glissement très dangereux entre la police judiciaire, police administrative on accorde aujourd'hui à l'autorité administrative des pouvoirs permanent alors qu'elle ne les avait que dans un cas que dans le cadre d'un état d'urgence certes reconduit 6 fois, mais dans un cadre a priori border ce que chacun pouvait craindre avec ses prorogation incessantes finit donc par se produire, nous voilà avec ce texte à l'aube, donc dans l'état d'urgence pourrait dire permanent et les quelques garanties apportées n'y changeront rien ce qui vous est désormais désormais proposée, c'est d'avoir, en parallèle, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire qui pourront être compétente en même temps et ainsi créer un système hybride, incarnée par le juge des libertés et de la détention, à un moment ou, au contraire, nous avons plutôt besoin de clarification, quoi qu'il en soit, la sécurité collective et la lutte contre le terrorisme ne résidera que dans un travail de plus long terme, des services de renseignement également alimentée par une police de proximité rénové une police judiciaire et des magistrats en charge de ces contentieux complexe selon des règles procédurales clairement définie, en référence à des infractions pénales, ce que ce texte semble ignorer et ce que nous continuons donc de vous proposer tout en nous opposant donc à ce type de dérives ainsi, vous l'aurez compris donc les membres du groupe communiste républicain et citoyen refuseront cette banalisation de l'état d'urgence permanent, véritable menace pour nos libertés publiques et voteront donc unanimement contre ça. La parole est à monsieur Philippe Bohn

il met notamment en évidence qu'une des premières qualités des sociétés qui résiste dans le temps, face aux aléas réside dans leur capacité à prendre conscience des mots qui les traversent au pouvoir ensuite formuler des des solutions de sociétés qui au contraire tarderait à regarder la réalité en face, accélérerait quant à elle, leur effondrement. En adossant à une 6ème loi de prorogation de l'état d'urgence votée la semaine dernière, ce projet de loi renforçant la sécurité intérieure, le gouvernement manifeste clairement sa volonté d'ériger la lutte contre le terrorisme, en priorité, c'est alors que nous venons de commémorer l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 86 innocents qui n'avait d'autre tort que de vouloir admirer le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet une preuve est plutôt rassurante : je trouve qu'il a pris la mesure de la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays je dis tit insistant car je sais que ce test : ce texte ne laisse pas indifférent, voire même inquiète et que des tentations existent dès lors que pas moins de 5 lois relatives à la lutte contre le terrorisme ont été adoptées ces dernières années, de porter un coup d'arrêt à ce que l'on qualifie de logique sécuritaire sans balayé d'un revers de la main les arguments avancés par les tenants d'une telle position, ma conviction, mes chers collègues, que nous avons besoin, plus que jamais de faire la preuve de réalisme et d'efficacité pour maintenir en vie, notre société. Cela étant, je souscris comme la majorité d'entre vous, elle n'de sortir de l'état d'urgence pour lui redonner son caractère exceptionnel, dès lors que la menace terroriste est devenue permanente. Dans les Yvelines, mon département, marquée par l'attentat de Magnanville comique contre un couple de pop policiers assassinés dans leur maison et sous les yeux, leurs enfants, comme ailleurs, l'état d'urgence a été conduit avec un grand professionnalisme par les autorités préfectorales sous le contrôle attentif des juges administratif et constitutionnel depuis novembre 2015 des forces de l'ordre ont fait preuve d'un dévouement exemplaire pour mettre en oeuvre ces mesures exceptionnelles dans des circonstances particulièrement dangereuse, mais il faut bien admettre que le régime d'état d'urgence désormais ces sous son efficacité décroît et sa seule évocation est devenue un signal paradoxal pour les Français qui exige à la fois que soit maintenu un niveau de vigilance maximale et Aspire aussi à tourner la page des attentats meurtriers. Face à ce constat, monsieur mise, vous proposez de créer de nouveaux outils administratifs permanents tirées du bilan de l'application prolongée de l'état d'urgence après un retour d'expérience ainsi certaines mesures sont montrés particulièrement efficace et il apparaît donc pertinent de faire en sorte de pouvoir profiter de leurs bénéfices sur le long terme, sans avoir à passer par là lors procédure de l'état d'urgence, et je pense notamment aux perquisitions administratives vous propose également de nouveaux dispositifs tels que la protection des lieux événements souligne menace particulière ou encore la fermeture administrative des lieux de culte ces mesures répondent à des voeux évolution concrète de la menace terroriste, les lieux accueillant des événements culturels ont en effet montré leur vulnérabilité que l'on pense à l'attentat du bord Bataclan ou encore à celui plus récent qui a endeuillé Manchester, de même la nouvelle procédure de fermeture des lieux de culture, décision du préfet constitue pour endiguer le phénomène de radicalisation un outil intéressant et complémentaire de la possibilité qui leur est déjà offerte de recourir à l'explosion de prédicateur radicaliser étrangers ou d'interdire des réunions, il s'agit également d'un message fort de responsabilisation adressée au propriétaire des lieux de culte qui ne peuvent tout simplement pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans leurs murs, nous légiférons pas ex nihilo et depuis la baisse corpus, entre autres, de nombreux textes de loi, on construit une architecture institutionnelle équilibrée destinée à assurer notre sécurité, tout en protégeant nos libertés, c'est la raison pour laquelle, dans une démarche de cons construction avec le gouvernement, les membres du groupe RDSE ont proposé d'introduire quelques modifications dans le but de garantir cet équilibre le texte il y a, ont été ainsi dotée de garde-fous destinés notamment à ce que des dispositions ne puissent pas être utilisé à des fins détournées, le groupe RDSE ne souhaite dès lors pas priver l'état des outils qu'il instaure même si l'alerte, le fait qu'ils seront seuls insuffisant, c'est pourquoi nous voulons dans le même temps réaffirmé que lutter efficacement contre le terrorisme, c'est aussi donner des moyens à la justice, et surtout peut-être au services de renseignement. Enfin, permettez-nous simplement de regretter que, s'agissant d'une loi aussi importante pour notre régime démocratique était à nouveau fait le choix de la procédure. Merci, merci Monsieur Philippe Aisne. La parole est à monsieur Philippe Bohn Carrère.

Monsieur le président, Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre mais, chers collègues, vous avez adopté le 4 juillet la 6ème progression de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale l'a fait le 6 juillet et la promulgation et du 11 juillet de sa déclaration le 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017, date de fin programmée, notre pays aura vécu pratiquement 2 ans, mais sous le régime de l'état d'urgence sur les 4 dernières emmené 8 lois ont été adoptées afin de lutter contre le terrorisme 18 décembre 2013 13 novembre 2014 24 juillet 2015 30 novembre 2015 22 mars 2016, 3 juin 2016, 21 juillet 2016, 28 février 2017, notre pays a pu compter sur l'engagement sans faille du Parlement dans la lutte contre le terrorisme, l'exécutif et le législatif ont conjointement doter notre nation de l'arsenal juridique le plus comblé le plus complet de combat contre le terrorisme, tout en restant une démocratie protectrice des libertés publiques, il reste à sortir de l'état d'urgence, régime d'exception, comme chacun le sait, dont chacun s'accorde à admettre qu'il ne peut devenir permanent, c'est l'objet du projet de loi qui nous est soumis, après une réécriture à l'issue de l'avis du Conseil d'État du 15 juin et une 2ème réécriture justifiée par notre commission des lois, sous l'impulsion de son rapporteur, Michel Mercier, disons-le tout Net, je ne vais pas reprendre le détail des articles, des amendements adoptés en commission, le rapporteur, mes collègues viennent de le faire, remarquablement je voudrais insister sur 2 éléments: premièrement, le texte dans la version qui vous est proposé rend assimilable au sens politique et juridique, les mesures souhaitées par l'exécutif, deuxièmement l'exercice d'équilibre recherché et réussi, premièrement, assurer l'acceptabilité. L'assimilation politique et ou juridique des dispositions issues de l'état d'urgence dans notre droit commun répond à la commande passée par le président de la République et par le gouvernement à l'issue de l'examen en commission des lois, je prenais connaissance du type suivant d'un article de presse, projet de loi antiterroriste le Sénat ampute les ambitions sécuritaires du gouvernement, je crois que c'est d'une part, excessif et, d'autre part, inexact, le travail réalisé avec par exemple la définition du 4 juridique d'intervention plus précis à l'article de l'autorisation du juge judiciaire la proportionnalité, le contrôle parlementaire la limitation dans le temps, ce travail est bienvenue, ce travail est aussi nécessaire si nous voulons rendre compatible le projet de loi avec le contrôle du Conseil constitutionnel, puis de la CEDEAO en d'autres termes, le travail qui a été réalisé et que vous êtes en train de prolonger en 7 séances et avec l'examen des amendements à suivre et ne consiste pas à raboter le texte mais au contraire on permettra Lamizana effective, deuxièmement l'équilibre ou les différentes formes d'équilibre Janez dénombré IV comme fil rouge du travail du Sénat l'équilibre entre la lutte contre le terrorisme et la protection des libertés individuelles proposées par le Sénat, avec détermination et finesse, mais je sais que pour Monsieur, le président de la commission des lois, ces 2 termes sont en le pléonasme s'agissant du Sénat est suffisamment évident pour me permettre d'aller directement à une 2ème forme d'équilibre dans la proposition soumise à savoir l'équilibre entre les pouvoirs exécutif, judiciaire, mais aussi législatif dans la durée, à travers le maintien que vous avez proposé, monsieur le rapporteur du contrôle par le Parlement une autre modalité d'équilibres porte sur la répartition des rôles entre le judiciaire et le juge administratif, nous n'aurions rien à gagner au maintien de tension entre le judiciaire et le juge administratif et cette question n'est pas le témoignage simplement de susceptibilité, nous avons assisté de texte en texte, ceci a été développée par plusieurs collègues ce que j'appellerais une optimisation une optimisation, extension de la police dite administrative et de la même optimisation en matière de droit pénal, les mesures de police administrative ne porte plus simplement sur la prévention, mais se rapproche de l'objet même du droit pénal, qui est la sanction et le droit pénal, a défini les infractions, notamment en matière de terrorisme, de plus en plus en amont de telle manière qu'il n'arrive lui-même à rejoindre la notion de prévention, ce qui veut dire qu'entre le droit Miss ratissent spéciale de lutte contre le terrorisme et le droit pénal spécial de même objet ce produit ce que Monsieur Michel Mercier, notre collègue Michel Mercier, appelé l'hybridation dans son rapport, à très juste titre et pour que cette hybridation fonctionnent pour que les choses se il y faut une précision, une élégance d'écriture, le dernier équilibres que je souhaiterais abordé en conclusion et celui entre droits communs et droit d'exception, la commande politique était connu, intégrer les dispositions utiles de l'état d'urgence dans le droit commun, nous partageons cette logique monsieur ministre mais l'état d'urgence ne peut pas fonctionner comme une boîte à mails où l'on transfère et d'une adresse à une autre, les messages ou d'une corbeille à une autre, si vous le préféré. Comment l'exception peut devenir le droit commun, quelle place dans notre système institutionnel à l'état d'urgence, si le droit d'exception devient le droit commun, comment garder une réponse progressive et différenciée en démocratie, à des situations de crise l'exercice mais indiscutablement pas aisée, le parlement accepte de le mener puisque il est très conscient de l'État continue de guerre menée par les terroristes, guerre qui s'inscrit dans la durée avec des auteurs agissant soit individuellement soit collectivement, soit par Auto radicalisation soit sur l'émission sinon commander du moins inspiré, auteur pour reprendre la formule de l'un de mes prédécesseurs à la tribune endogènes comme exogènes, nous avons en tête la fermeté nécessaire dans la durée, c'est le sens de la palette des amendements qui ont été adoptés par la commission sous votre impulsion, monsieur le rapporteur, en espérant que le gouvernement voudra bien ont partagé la pertinence pour d'autres objectifs communs de lutte contre le terrorisme, en conclusion, notre groupe est favorable à doter l'État de droit, de moyens lui permettant de se défendre face à une menace terroriste permanente et non ponctuel dans le respect des droits et des libertés, en vous remerciant cher collègue de votre attention. Merci Monsieur, bonne qui la parole est à Jacques Bigot.

Monsieur le président, Monsieur le ministre d'État, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois Monsieur rapporteur monsieur rapporteur pour avis mais chers collègues. Personne ne saurait ici ici l'existence du risque terroriste sa permanence et le côté dramatique de ce que vivent les victimes du terrorisme, et l'angoisse de nos concitoyens face au terrorisme. Et le rappeler, comme vous l'avez fait monsieur le ministre tout à l'heure ne justifie pas forcément l'ampleur des textes et des atteintes à notre système démocratique et judiciaire que vous proposez. D'autant plus que le risque terroriste semble s'amplifier d'une certaine manière, par l'évolution de la nature du terrorisme Charlie-Hebdo le Bataclan, c'était des opérations très organisé, très commandé aujourd'hui, on a de plus en plus et ça a été le cas à Saint-Étienne-du-Rouvray à Nice des récemment sur les Champs-Élysées, des individus isolés qui entend en contact par le biais d'Internet organisent leur propre activité terroriste de manière complètement qu'isolé, et donc effectivement le danger se renforcer précisément par cela et ce n'est pas la chute de Daech au Moyen-Orient qui va limiter les risques, nous en sommes bien conscients et il risque même d'être d'une certaine manière démultipliée. Et pour autant, c'est le souhait du président de la République, il avait exprimé depuis longtemps, on ne peut pas rester dans le cadre d'une loi de 1955 bien qu'elle était modifiée et renforcée par des mesures démocratiques importantes, je pense notamment à l'article 4 qui obliger le gouvernement à tenir informer le Parlement et à rendre compte régulièrement des mesures qui étaient prises, on ne peut pas rester en permanence dans ce système d'état d'urgence, qui en plus inquiète d'une certaine manière, nos concitoyens parce que il est une façon de leur rappeler que le risque existe, je crois qu'il faut effectivement le leur rappeler, ils en sont bien conscients, ils en sont bien conscients, dans ce que nous avons prolongé l'état d'urgence à la veille de l'Euro, ils l'ont compris aussi ce que malgré les convictions que nous avions les uns les autres, notamment après la preuve la la la loi du 3 juin 2016 dernière loi renforçant les moyens donnés aux services de renseignement au procureur de la République au moyens judiciaires, nous pensions que tout avait été fait pour que nous n'ayons plus besoin de l'état d'urgence et pourtant après l'attentat de Nice, le gouvernement nous a demandé de le prolonger encore

Et pourtant, si nous avions écouté, celui qui est aujourd'hui notre président de la République, nous n'aurions pas dû en décembre 2016 votez la progression de l'état d'urgence, puisque lui-même écrivait au mois de novembre dans son livre, qui a déjà été cité que nous devons sortir de l'état d'urgence et que nous avons dans nos textes dans l'arsenal législatif, tous les moyens juridiques nécessaires pour lutter contre le terrorisme, donc nous n'avions plus besoin des mesures de l'état d'urgence dans le texte que vous nous proposez monsieur le ministre, il est des mesures administratives qui effectivement peuvent nous paraître nécessaire, s'agissant de l'article 1er qui est aussi controversé comme comme d'autres s'agissant de nos concitoyens veulent que l'on puisse continuer à organiser des manifestations, vous l'avez remplir rappeler des manifestations d'ampleur. Conçoit pas privé mais qu'en même temps on essaie de rechercher la sécurité maximum de ces manifestations, on est là dans la compétence tout à fait normal de l'autorité administrative, notamment du préfet qui doit pouvoir prendre des mesures telles qu'elles sont décrites à l'article 1er avec sans doute quelques modifications qui était proposé, monsieur le rapporteur par la commission avec des prudences qui sont nécessaires, mais on est tout à fait dans le cadre des mesures administratives et je crois que nos concitoyens cela le comprennent bien. S'agissant de l'article 2 et de la fermeture des lieux de culte, nous sommes effectivement à la limite de la commission d'infraction, c'est l'apologie du terrorisme, qui serait propagée dans ces lieux de culte et qui justifierait à même déjà les poursuites pénales et des mesures qui pourraient être prises Il est utile, avoir la Poste et d'une mesure administrative et on doit souligner que dans le texte qui mérite là aussi quelques modifications, on en parlera tout à l'heure, il était très intéressant de voir que vous ouvrez la possibilité au président de l'association de cet axe cas de lieu de culte de saisir le juge des référés Al-Misrati fait que la mesure ne prendra effet que après que le juge se soit prononcée dans les 48 heures, je pense que là on a une forme de protection des libertés qui est intéressante malgré une mesure qui est le. Les mesures dans notre collègue Michel Boutant a parlé tout à l'heure ne nous pose pas de difficultés particulières, d'autant plus que il est quand même proposé un fort contrôle de Lixus Lisa Sion de prises de renseignements par voie aérienne et de l'interception des communications et je pense que de ce point de vue là nous pouvons soutenir les propositions qui vous sont faites, comme l'a dit à l'instant, notre collègue Alain Richard parlant pour le groupe, la République en marche les mesures les plus décriées sont celles de l'article 3 et de l'article ce sont des mesures très attentatoire aux libertés, dénoncées par le défenseur des droits, ancien garde des Sceaux, dénoncée par la Commission nationale de la scène des Ch dénoncé par toutes un mouvement important de professeurs d'université, des magistrats, 2 organisations syndicales et pas forcément des gens qui souhaitent à l'extrême gauche, je ne crois pas, et donc, très clairement, il nous faut pour accepter ces articles, avoir des explications qui soient claires. On ne peut pas envisager. De prolonger. Dans le droit commun, les mesures de l'état d'urgence, je souligne, monsieur le rapporteur, votre habileté. à avoir réussi à montrer dans la rédaction Nouvelles des articles III et IV que finalement vous souhaitiez adoucir la mesure mais en même temps et on y reviendra tout à l'heure dans les débats, la manière dont vous avez re rédigé les articles 3 et 4 nous prouve si besoin. N'était que l'on peut rester entièrement dans le Champ judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a à côté du pouvoir police voie administrative, le contrôle et l'autorité du procureur et du juge des libertés. Et mettre ces mesures dans ce cadre-là est parfaitement possible, on ne peut pas se contenter de dire que quelqu'un est mis sous surveillance ne parle plus d'assignation à résidence pour des raisons sérieuses quand il y a des raisons sérieuses de penser. Et de penser que son comportement en fait est constitutif d'infractions qui sont déjà sanctionnés par les articles de la loi, vous dites vous-même, monsieur le rapporteur, que ces textes, article 3 comme article 4 suscite des interrogations et à telle enseigne que vous nous proposez en fait d'en faire des mesures d'exception limitée dans le temps alors temps plus long que 6 mois, mais un temps de 4 ans. ans. Sans toutefois, et c'est aussi important, parce que Monsieur, mannequin je crois rappeler l'importance du pouvoir législatif dans l'état d'exception dans l'état d'urgence le Parlement avait ce pouvoir de contrôle, information et contrôle tous les 6 mois au moment de la demande de renouvellement, ici, dans ce que vous proposez, monsieur le rapporteur, pendant 4 ans, le pouvoir exécutif pourra faire ce qu'il veut et ce sera le simple contrôle pour l'essentiel du pouvoir administratif de la juridiction administrative,

la seule différence, c'est que le aime intervient toujours à postériori alors que il contre l'excès de pouvoir alors que. Le juge glissières et celui qui autorise et il peut parfaitement prendre toutes les mesures qui sont prévues à l'article 3 il y a l'article IV mais dans le cadre de débat contradictoire prévu le cas échéant, dans le cadre de mesures d'instruction sous le contrôle judiciaire et c'est ce que nous démontrerons tout à l'heure et il n'y a pas de raison d'en sortir et c'est la raison pour laquelle nous proposerons comme d'autres des amendements de suppression de Ceuta et de ses 2 articles qui ne nous paraissent pas utile. Ou dans la salle, lité mais à ce moment là, Monsieur le Ministre, ce serait grave sur c'est très grave, c'est de laisser croire aux Français et aux Françaises que le président de la République qui est convaincu qu'il faut quitter l'état d'urgence à trouver la bonne solution et qu'il maintient quand même un état d'urgence déguisé pour les rassurer, hé bien non, je crois, comme l'a dit un de nos collègues, c'était François Pillet dans la commission des lois, on est sans doute aller du point du législatif au bout du bout, et il faut effectivement peut-être expliquer aux Français ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible d'apporter une sécurité absolue, par contre, les moyens dont la police a besoin de nous serons toujours à vos côtés pour les apporter, de même que nous espérons que le gouvernement donnera à la justice les moyens dont elle a besoin parce que c'est vrai que donner des pouvoirs, un juge des libertés, un procureur de la République suppose qu'ils aient des moyens, or nous savons que ces moyens ne sont pas au rendez-vous : le rapport que à déposer notre président de la commission des lois auxquelles j'ai parfaitement participer, a prouvé le contraire, et la nécessité d'urgence d'une loi de programmation pour permettre à la justice d'être plus efficace en ayant plus de moyens pour toutes ces raisons, nous attendons ce débat, monsieur le ministre d'État, je n'aurai qu'une demande retirer les articles 3 et 4 et nous serons ravis de voter la loi, si vous n'est retiré pas, nous serons contraints de vous dire et de vous rappeler ce que le président de la République lui-même a dit en novembre 2016. Merci monsieur Jacques Bigot. La parole est à monsieur le ministre. Bien, mesdames et messieurs les sénateurs. Quelques mots pour répondre aux différents orateurs, je crois que Monsieur Buffet a explicité dans son intervention, quelques propos de la commission et nous aurons l'occasion tout auto au cours des articles de pouvoir discuter de cet équilibre que nous souhaitons pouvoir trouver en sang. Monsieur racheter une je n'en parlerai pas sauf pour lui dire : peut-être que le héros du plateau des Glières ne pensait pas être cité comme cela dans cette assemblée, monsieur Richard avec l'esprit de finesse qui au moins égal à celui de monsieur le rapporteur expliciter toutes les subtilités des articles 3 et 4 dont nous aurons évidemment l'occasion de discuter sur lesquels nous préciseront ce qui Pearl peut permettent d'avoir un équilibre toujours difficile à trouver entre protection de la sécurité donc nécessité de prendre un certain nombre de décisions en amont et puis en même temps, garantie des libertés individuelles, monsieur Christian Favier, je crois, par principe, hostile à toutes les mesures, je pense que, depuis qu'un certain nombre de mesures ont été proposées, il n'en a voté aucune donc il continue dans sa logique, permettez-moi simplement de de vous dire que, peut-être, en face de nous, nous avons un certain nombre d'adversaires qui ne sont pas exactement dans les mêmes logiques que nous nous avons hélas à affronter un danger bien réel et que ce que je peux, je peux voir des notes qu'on me donne nous montre l'étendue

je partage totalement c'est et c'est pour cela que nous portons ce projet de loi parce que évidemment nous avons conscience de la difficulté dans laquelle nous sommes, je réponds d'un mot à ce qu'on cite souvent des phrases du président de de la République, permettez-moi de vous dire que lorsque l'on prend connaissance d'un certain nombre de notes et on ne les a pas forcément avant d'être président de la République, on peut prendre conscience de l'ampleur du danger, il avait dit par ailleurs qu'il apprécierait au moment où il serait élu, c'est-à-dire quand il aurait la véritable connaissance de la situation dans laquelle nous sommes sa propre décision en fonction des éléments d'analyse qu'il ferait de la situation

comment il y avait un espèce d'équilibre qui était en train de de se constituer entre police administrative et police judiciaire avec les en prenant plus en amont et les autres, donc ayant le le souci de, de, de pouvoir conserver un certain nombre de prérogatives qui tendaient à rapprocher les 2 institutions Monsieur Bigot mais nous aurons l'occasion de discuter évidemment des articles 3 et 4 je m'aperçois qu'il est d'accord avec l'article 1 il a raison est à être d'accord avec l'article 1 parce que, à Strasbourg, si effectivement l'article 1 n'existait pas, je crains que le marché de Noël ne puisse se tenir, ce qui évidemment serait moyennement apprécié par ses concitoyens par ailleurs entre un certain nombre de dispositions qui avaient été votées précédemment et puis les dispositions que nous proposons aujourd'hui me semble il y avoir comme un air de continuité, je ne sais pas où a pu intervenir exactement le changement, mais je le laisse lui-même juge de sa propre évolution de penser

Merci monsieur le ministre, la discussion générale est Close, je vais suspendent 10 minutes la séance, elle sera reprise à 17 heures 20. Séance est suspendue.

La séance est reprise comme saisie de 2 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune : l'article 1er un amendement numéro 5 qui est défendu par Madame Assassi. Azziman chers collègues. Ce président, monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues, à travers cet amendement de suppression de l'article 1er nous souhaitons alerter sur cette partie qui confie effectivement au préfet la compétence pour instaurer des périmètres de protection, je cite, permettant, assurer la sécurité des lieux ou d'événements, soumis à un risque d'acte de terrorisme, à raison de leur nature ou de l'ampleur de la fréquentation ce périmètre, le périmètre, le préfet pardon peut également réglementer l'accès, la circulation, le stationnement des personnes afin de pouvoir organiser le filtrage des accès à ce périmètre protégé ce filtrage permet de procéder à des palpations de sécurité à l'inspection visuelle, voire à la fouille de bagages, nous sommes inquiets de ces nouvelles dispositions qui sont mises en place par le gouvernement qui, de fait, confère aux préfets des pouvoirs disproportionnés en matière de sécurité publique, les mesures proposées risquons-nous de permettre une application discriminatoire dès lors que les fouilles ne requiert aucune base objective les agents définie comme pouvant intervenir pour mettre en 9, ces mesures suscitent également notre plus vives inquiétudes puisque les agents de police municipale, les agents de sécurité privés ou autres agents de gardiennage ne dispose pas de la formation nécessaire pour appliquer de façon plus égalitaire, j'ai envie de dire ici ce genre de mesures enfin la question de l'usage de ce type de mesures nous inquiète pour parce qu'elle pourrait, à terme, et même si j'ai entendu ce que vous avez dit monsieur le Ministre dans vos réponses tout à l'heure une fois inscrit dans la loi, ces mesures pourraient permettent d'étouffer et de réprimer tout type de contestation politique sur la voie publique, pour toutes ces raisons et bien d'autres, mais que le temps ne laissera pas, nous nous opposons à l'adoption d'une telle mesure et nous proposons donc la suppression de cet article 1er. Merci, ma chère collègue un amendement numéro 25 rectifier d'anticorps numéro 5 Madame Benbassa. Monsieur le président, mes chers collègues, principale innovation par le rapport à l'état d'urgence, l'article 1er du projet de loi confère aux préfets est apparu au préfet de police, le pouvoir d'instituer afin afin d'assurer la sécurité des lieux ou d'événements, soumis à un risque d'acte de terrorisme des périmètres de protection au sein desquelles l'accès et la circulation des personnes seraient réglementées, quelle idée de société transparaît au travers de cette disposition, je vous le demande, une société du soupçon qui permet de contrôler, de fouiller sans motif valable, une société qui favorise la stigmatisation de nos concitoyens musulmans qui, loin de lutter contre les discriminations, les facilite. Notre devoir est de lutter contre les contrôles au faciès, pas de les encourager. De surcroît, dans la période que nous vivons, quels sont les lieux où les événements qui ne soit soumis à aucun risque datent de terreur, soyons sérieux, mes chers collègues, une telle restriction des libertés n'est pas nécessaire pour lutter contre le terrorisme, ce qui est efficace, en revanche, c'est une action coordonnée des services de l'enseignement et des services d'enquête judiciaire et des moyens conséquents alloués à ce service, ce qui est efficace, c'est aussi de réfléchir aux causes et de faire de la prévention, une priorité, nous, nous nous avons débattu ici de nombreux textes visant à renforcer l'arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme, certains d'entre nous ont alors dénoncé c'est inflation législative, basées souvent sur l'émotion et sur la volonté de donner aux réponses à nos concitoyens inquiets. Le président change le 1er mini-change mais rien ne change, et nous voilà, nous voilà à nouveau autour donne texte un peu plus attentatoire aux libertés individuelles que les précédents et une fois de plus, nous sommes bien peu nombreux en débattre aujourd'hui comme si le législateur lui-même était devenu apathiques merci. Merci, ma chère collègue, monsieur le rapporteur pour la vie de la commission. Merci monsieur le président, la commission exprimé tout à l'heure, l'intérêt que présentait cette mesure, c'est une mesure qui est en effet de nouvelles dans notre droit, et c'est celle qui permet le que certains nombre de manifestations culturelles ou autres puisse se réaliser, on a parlé du marché de Strasbourg, on pourrait parler et de l'Euro 2016, ou d'autres manifestations de ce type pense donc qu'elle mérite, cette mesure de préciser d'être encadré, mais elle doit exister, c'est à ce prix là que l'on pourra continuer à voir ces manifestations donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement. Avis défavorable pour les raisons que j'ai évoquée tout à l'heure, voyez pour de grands événements, la Biennale du Design, il peut arriver, par exemple, que nous ayons besoin d'établir ce type de périmètre et donc de procéder pour sécuriser les lieux, un certain nombre de palpations pour Madame Ben ça je lui dirais qu'il n'y aura jamais tant que je serai ministre de l'Intérieur, de discrimination et de contrôles au faciès, il n'est d'ailleurs prévu aucun contrôle d'identité dans ce dans ce texte, c'est simplement de pouvoir faire ouvrir les sacs de pouvoir effectivement vérifié que personne n'a d'armes diverses et variées dans ce type de grandes manifestations avis défavorable. Merci monsieur le ministre, il y a-t-il des explications de vote. Monsieur Assouline. j'ai un avis que j'exprimerai sur les articles 3 et 4 sur l'économie générale de de cette loi qui, à mon sens ne va pas dans le bon sens, mais cette mesure-là est en discussion et nous devons d'ailleurs à travers cet article comme sur le reste, aborder la question que nous essayons, discuté depuis le début d'un marine à qui, comment, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, comment protéger, sécuriser, se défend et en même temps, défendent la liberté et la liberté individuelle et collective, c'est le défi. Nous lancé les terroristes de toute façon, et donc si nous tombions dans la sécurité, comptez liberté ils auraient gagné donc la lutte contre terrorisme passe par le fait que nous soyons attentifs et que nous garantissons à la fin, et pendant cette lutte, les libertés, c'est bien ça qui nous ont lancé comme défi alors là, je vois bien et d'ailleurs, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez à chaque fois évoqué

probablement, c'est d'une situation permanente, encore pour quelques mois, quelques années parce que même quand on dit que sur le terrain sont entrain de perdre, c'est le retour aussi de nombreux d'entre notre pays et donc on a cette menace encore pour longtemps mais vous évoquez pas un aspect qui me tient particulièrement à coeur, c'est les manifestations revendicatives et du mouvement social et nous voyons bien là à ce moment-là, pourquoi.

contrôler l'accès établir un périmètre pour toute manifestation d'ailleurs à Paris le on pourrait évoquer le danger terroriste parce que, une grande manifestation pas la République Bastille etc faudrait l'évoquer ailleurs ça a déjà eu lieu, c'est pour ça que les défenseurs des droits lui est contre et c'est pas un grand gauchiste disons donc là, le leader de la CGT plus dans son rôle et c'est normal, j'interroge le ministre la dessus qu'est-ce qui se passe, comment c'est utilisé pour l'ensemble des manifestations qui importantes qui sont prévus, qui sont courantes, notamment dans la capitale, le contrôle systématique etc et à est de nature à dissuader au moins et donc il y a un problème là de liberté collective à mettre en face du danger réel à chaque fois qu'on va de manifestation, c'est qu'un danger aujourd'hui, mais comment on tranche sur les 2 j'aimerais écouter les esprits. Merci y a-t-il d'autres explications de vote, je n'en vois pas je mets aux voix c'était oui, j'ai mon cher collègue, excusez-moi, je vous ai pas vu. Oui je je voulais aussi donc dans le complément de ce que dit David Assouline exprimer les les mêmes inquiétudes il me semble, et c'est un peu le problème de cette proposition de loi que typiquement, nous sommes là dans de l'état d'urgence dans une situation exceptionnelle, ça ne peut pas devenir une norme habituelle, c'est quand même une décision lourde qui est prise-là parce que, effectivement, la définition est quand même vague, donc quand l'état dure Jeanson prenne des mesures exceptionnelles, c'est la logique de l'état d'urgence en faire en faire la règle habituelle me semble très discutable et donc en complément de la question David Assouline pour pour le ministre, la question est aussi la question du recours, c'est-à-dire où peut-on finalement remettre en cause le fait que le préfet, juge qu'il y a une situation de de risques terroristes parce que on va se retrouver avec des situations assez conflictuelle si les organisateurs de la manifestation conteste même le le classement risque terroriste.

vous m'inquiétez quand vous dites tant que je serai ministre. De l'intérieur, on ne pourra créer de périmètres de protection pour empêcher des manifestations certes voulait ce propriétaire de vos paroles Monsieur Richard de de toute évidence, malheureusement, je ne sais pas comment lire monsieur Collomb ne sera pas ministre de l'Intérieur Habib on peut craindre en tout cas nous nous ferons tout pour qu'il n'en soit pas ainsi, mais imaginons qu'un gouvernement d'extrême droite arrive malheureusement au gouvernement et je répète : nous ferons tout pour qu'il n'en soit pas ainsi, avec cette mesure, qui rentre dans notre droit commun, on pourrait être confronté à des interdictions majeures qui toucherait au coeur même de notre démocratie, donc voilà aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes pour la suppression de cet article 1er. Merci Madame assassiné, Monsieur le Ministre. Je veux dire, madame assassiné bord que si un régime d'extrême droite venait, je pense qu'il pourrait prendre d'autre loi que celle-ci est donc, oui, donc ce ne sera pas celle-ci qui sera appliqué hélas je le craindrais je vous rappelle que nous parlons ici Pau répond. Monsieur Assouline d'événements culturels et sportifs, et non pas donc de défilés de cortège de rassemblement de personnes sur la voie publique, qui elles sont gérées au titre les articles L 211 1 L 214 du code de la sécurité intérieure, donc je lui précise que nous avons affirmé et réaffirmé que ces mesures ne seraient pas utilisées pour maintenir l'ordre public. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets donc on voit ces 2 amendements, l'amendement numéro 5. Qui s'abstient

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, nous abordons l'examen de cet article dans l'état d'esprit suivant nous sommes favorables à la création d'un outil juridique nouveau destiné à former un périmètre de sécurité pour protéger les lieux accueillant ponctuellement des événements nous sommes vigilants à ce que ce nouveau dispositif ne constitue pas une charge supplémentaire pour les communes, c'est le risque, si la police municipale devient certes avec l'accord des maires, la clé de voûte de ces périmètres de sécurité, nous souhaitons également que ces nouveaux périmètres ne constitue pas un obstacle à la vie culturelle normal de nos territoires et ne s'installe pas dans le temps selon les lieux, ceci étant clarifié janvier à l'amendement 53 rectifier, nous considérons que l'article pourrait se passer de la mention de lieux à protéger en ne gardant que celle d'événements, en effet, s'il s'agit de ce 1er mai du risque temporaire liée à l'afflux de la population ou d'un risque anormal pesant sur des lieux lié à un événement insensible la mention d'événements ne suffit elle permettra la protection de ces lieux au seul moment où c'est les événements se dérouleront si en revanche des lieux sont par essence, soumis à un risque particulier pour ce qu'il représente, il nous semble nécessaire de prévoir des dispositifs pérenne pour les protéger, comme cela est déjà le cas pour les centrales nucléaires par exemple, telle est l'état d'esprit de cet amendement. monsieur le rapporteur de la commission des lois. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. L'avis est défavorable, il y a un certain nombre de lieux tout à l'heure monsieur le rapporteur, a évoqué la Tour Eiffel par exemple ou ce genre de mesures doivent pouvoir être prises, donc avec des favoris. Merci monsieur mise état monsieur Assouline pour l'explication de vote. J'en profite pour rebondir parce que la réponse du ministre à ma question et Matterhorn vraiment parce que c'est pas le projet de loi, projet de loi, pas de mesures visant les manifestations culturelles ou sportives, je lis article L de 226. Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement, soumis à un risque d'acte de terrorisme en raison de sa nature ou de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'État dans le département où à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, donc ça c'est le texte de loi peut discuter d'autre chose, vous pouvez proposer un amendement qui disent les manifestations sportives ou culturelles, mais là il s'agit de toute événement manifestation où il y a un risque terroriste il y a le reste terroriste surtout grand rassemblement de personnes à Paris, manifestation revendicative sociale ou autres et spécifié donc peut-être c'est parce que vous vous apprêtez à faire un amendement mais ne me dites pas que dans le texte, c'est circonscrit aux manifestations sportives, culturelles, ce n'est pas le cas, donc j'attend encore une réponse. Merci monsieur Assouline, y a-t-il d'autres explications de vote, je n'en vois pas, je rappelle qu'il y a eu un avis défavorable de la commission d'avis défavorable du gouvernement je m'est amendement 53 rectifier au au vote qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté un amendement et un sous-amendement qui font le c'est l'objet d'une discussion commune toujours article 1er un amendement 67 qui est présenté par le gouvernement, monsieur le ministre d'État. nous souhaitons par cet amendement, revenir à la rédaction initiale proposée par le gouvernement sur plusieurs aspects de l'Artic 1er d'abord, la commission a introduit pour la qualification du risque terroriste, les maux actuels et sérieux, comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, nous pensons qu'aujourd'hui, le risque est malheureusement toujours actuelle et sérieux en 2ème lieu le gouvernement est bien entendu pleinement qu'. Conscient de la nécessité d'adapter les dispositions d'accès et de circulation dans les périmètres concernés aux impératifs de la vie privée familiale aux professionnels, pourtant il lui apparaît tout autant indispensable de préserver la possibilité de soumettre aux vérifications prévues par cet article, inspection des bagages et visite des véhicules, les personnes travaillant dans le périmètre. Devanciers rendent pour un motif familial pour des raisons que là aussi, j'ai précisé dans mon intervention liminaire en disant qu'évidemment on pouvait toujours prendre un faux domicile pour pouvoir commettre un attentat.

on peut en effet se rendre aux arguments du gouvernement sur l'expression actuelle est sérieux, la commission des lois, après en avoir délibéré ce matin serait d'accord pour abandonner et cette condition. Sous la condition que les 2 conditions évoquées dans le texte initial du gouvernement de Vienne cumulative et pas alternative, sous cette réserve là et il nous semble que le le texte serait acceptable et puis on comprend bien que certaines mesures doivent avoir une durée dans le temps plus longue. Mais est néanmoins on peut difficilement accepter la commission ne peut pas accepter qu'il n'y a pas de délai maximum donc, la commission des lois vous propose de sous-amendé le texte du gouvernement, en prévoyant un délai de un mois qui est d'ailleurs renouvelable, le préfet de pouvoir constater que les conditions qui ont conduit à prendre l'arrêté créant périmètre de protection demeure et donc pouvoir renouveler mais de mois en mois, mais pas pour toujours. Sous la condition d'adoption de sous amendements, je pense que pour lui ont donné un avis favorable à l'amendement du gouvernement. Merci Monsieur Mercier, que pense le gouvernement de ce sous-amendement. Le gouvernement est favorable au Suzann Mandement proposé par le rapporteur et par la Commission, je reviens un peu sur donc ce dont nous avons discuté précédemment, donc sur la le caractère de d'abord immédiat, il faudra quand même qu'on a une expertise juridique et technique sur ce que pourrait entraîner le mot immédiat ok, merci. Merci monsieur le ministre d'État, il y a-t-il des explications de vote, je n'en vois pas je vais d'abord faire voter le sous-amendement numéro 83 qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

Monsieur le président Monsieur ministère comment la on l'a souligné auparavant, l'objectif est de maintenir une vie culturelle normale dans tous nos territoires en s'assurant que ces événements se déroulent dans les meilleures conditions sécuritaires possibles, il s'agit ici de clarifier la modalité de définition des mesures de protection déployées dans le périmètre et notamment de mieux associer des organisateurs d'événements à leur définition, en particulier l'amendement vise à ce que les organisateurs soient informés en amont de la tenue des événements du dispositif mis en oeuvre afin de leur permettre d'adapter leur programmation si besoin tout en descente,

Merci monsieur le président, la commission amendement présenté par Monsieur Guérini et nous pensons que, bien entendu, l'autorité. Administratives dialoguer avec les organisateurs de manifestations et que l'arrêté qui créé le périmètre de protection est aussi le résultat d'un dialogue, on va pas créer un périmètre de protection pour organiser, ai pas match un grand match de football, ça j'en parler avec les organisateurs du match donc la formation a eu lieu l'abonnement me semble surabondant, raison pour laquelle la Commission demande le retrait et à défaut : avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Même avis que la Commission et pour les mêmes raisons, monsieur Guérini donc retrait ou bien avis favorable.

L'article 1er du projet de loi prévoit actuellement que les maires seront informés de la mise en oeuvre du périmètre sécurité au moment où le préfet sollicitera leur contribution via la demande d'appui de la police municipale, j'en profite ici pour faire une petite indiscrétion CO2 vous permettez, l'association de la police municipale à ce nouveau dispositif relève évidemment du bon sens, si cette force existe, il est normal qu'elle contribue au périmètre de sécurité, ces dispositions est cependant sujette à une quiétude notamment au risque que la mise en oeuvre des périmètres de sécurité repose essentiellement sur la mobilisation de la police municipale, selon les arbitrages du préfet en d'autres termes, nous redoutons que cela constituait un transfert de charge caché de l'État vers les collectivités territoriales, grand débat Monsieur Mercier, je vous vois très étonné, nous serons particulièrement à ce que d'tas tiennent c'est promesse et que le fonds dédiés à la protection des événements culturels effectif jusqu'en 2018 ne soit pas remis en cause, pour revenir à l'amendement, il paraît important de mentionner dans le test que le maire. Je dis bien que le maire sera toujours informé du périmètre au même titre que le procureur de la République, y compris dans les communes ne disposant pas de police nationale ou lorsque le préfet choisira de ne pas la mobilisés. que le maire soit informé que l'arrêté que par le préfet, créant périmètre sur sa commune, me semble tout à fait normal quand à l'utilisation de la police municipale, je rappelle absolue Guérini qu'elle est soumise à l'autorisation du maire, c'est le maire qui décide, ou non, donc il peut pas y avoir de transfert de charge si cela été acceptée par le maire. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Oui, comme l'a dit le rapporteur je ne pense pas que le préfet puisse ne pas informer le maire de la commune, je rappelle d'ailleurs que sur l'organisation des grands événements, c'est plutôt les maires qui sont demandeurs de ce type de dispositif et donc c'est en général qui appelle le préfet pour lui dire : Monsieur le Préfet voilà nous organisions telle grande manifestation et nous serions extrêmement heureux que vous puissiez mettre en place ce dispositif et en général, ils font appel à la police nationale et gendarmerie je rappelle par exemple que pour les 14 et 15 juillet ces 80 6000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés. Merci, Monsieur le Ministre, alors la vie est favorable, défavorable.

Cet amendement, monsieur le président, vise à faciliter le recours au juge administratif, par voie de référé liberté des personnes, il y a intérêt à agir contre l'instauration d'un périmètre de sécurité, en prévoyant que l'urgence est présumé, ce faisant, elle n'aura pas à être démontrée par le requérant qui pourra se concentrer sur la démonstration des autres moyens de sa requête, l'objectif de cet amendement et donc de faciliter l'accès au juge administratif, un cas d'instauration de périmètre de sécurité.

dans le cadre d'un référé-liberté très bon je pense que il appartient aux demandeurs de démontrer qu'il y a urgence, c'est-à-dire que la mesure prise par le préfet va bouleverser ses conditions de vie et d'exercice et toucher, s'agissant du d'une liberté fondamentale, donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Je partage l'avis du rapporteur, l'appréciation de l'urgence relève évidemment du juge au regard des circonstances particulières de chaque situation sans qu'il soit nécessaire de contraindre son appréciation par la loi, retraits ou un avis défavorable. Merci monsieur le minus Monsieur Richard pour l'explication de vote. Je je crois qu'on devrait ajouter une petite nuance aux propos et du rapporteur et du ministre parce que dans le cas où une liberté est en cause si le juge considère qu'il est saisi d'une contestation d'une mesure administrative qui met en cause une liberté à ce moment-là, le juge considère que si la procédure du référé-liberté qui s'applique et là l'urgence à ce moment-là est présumé le juge peut se prononcer dans les 48 heures, donc il me semble que ce qui est en jeu, c'est de savoir si dans tous les cas, parce que, au fond, ce que propose notre collègue c'est que dès l'instant où il y a une décision de zones de sécurité, la liberté individuelle de quelqu'un et forcément mise en jeu, je pense que c'est à chaque personne de le démontrer, et donc il ne faut peut-être pas qu'on oblige le juge a considéré, dans tous les cas que la liberté d'individuel est en cause. C'est Monsieur Richard. Je le mets au voir je rappelle qu'il a reçu 2 avis défavorables Dans ce genre d'événement, une manifestation qu'on organise dans mon département, auteurs de 100000 personnes, bon effectivement, à certains moments, le préfet peut prendre des mesures excessives, donc ce qui était indiqué, se justifie, c'est peut être tout à fait excessif parce que les préfets et directeurs de cabinet ailleurs qui font ça, ils ont peur

Oui, merci, merci, monsieur le président Monsieur musette, les policiers municipaux sont considérés comme la 3ème force de sécurité dans le pays, si l'on peut se féliciter que ce projet de loi sur la sécurité intérieure n'oublie pas la police municipale, il convient d'aller un petit peu plus loin le filtre à Lévis le filtrage des accès au périmètre de protection palpations de sécurité inspection visuelle fouilles de bagages soit assurée par les policiers et les gendarmes, officiers, agent de police judiciaire après l'accord du maire, ils pourront être assistés par les agents de la poste de police municipale, néanmoins, ces derniers ne pourront les assister pour la fouille des véhicules susceptibles de pénétrer au sein du périmètre de protection, ils l'ont proposé les autorisés à effectuer ces fouilles après accord du maire, ce 8 sous l'autorité de l'OPJ compétents et naturellement le consentement des produits je profite de cette occasion Monsieur le ministre d'État, au moment où on demande à nos collectivités de faire un effort financier extraordinaire pour appeler le poids budgétaire des polices municipales et au fil du temps, j'ai pu mesurer combien il y avait entre les polices municipales et les forces de de lors de l'État, un travail en commun extrêmement important, je rappelle quand même que nos collectivités nos communes mettent à disposition aussi de l'État,

d'une mission qui n'est pas la nôtre, mais que nous assumons quand même pour compléter celle de l'État efficace non merci. Merci monsieur, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup Monsieur Président l'amendement que vient de présenter, monsieur Grand vise endroit à étendre aux agents de police municipale, la possibilité de procéder à des visites de véhicules ça et périmètres de protection instituée par arrêté préfectoral, vous savez que d'autres, droit. Le véhicule fait partie, c'est une sorte de démembrement du domicile pour le juge, en tous les cas, il y a une jurisprudence constante depuis très longtemps dans ce pays accordé aux aux agents de police municipale, le droit de fouiller avec le consentement du propriétaire, bien entendu, sinon il faut entrer dans une procédure judiciaire véhicule me semble quand même quelque chose qui était assez attentatoire au liberté individuelles réserver ce droit aux agents de police, gendarmerie, formés à cet effet, me semble une bonne mesure d'équilibre pour respecter mais liberté individuelle, donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur merci. Monsieur le ministre d'État pour la vie du gouvernement. Bien évidemment, le ministre ne mésestime pas le rôle des polices municipales est évidemment apporte un concours extrêmement important à la sécurité dans nos villes et dans nos communes s'agissant particulièrement des opérations de visite des véhicules c'est vérification comme l'a dit Michel Mercier, qui touche au droit au respect de la vie privée sont actuellement réservées par le code de procédure pénale aux policiers nationaux et aux gendarmes qui peuvent y procéder dans certaines conditions, à l'occasion d'un contrôle d'identité et donc avis des Far Rabat au retrait. Merci monsieur le ministre, monsieur Grand. Oui, si cet amendement n'est pas venu comme ça, il s'inspirer à la lecture des rapports de police nocturne dans dans nos colonnes aux et quand vous avez 2 gendarmes devant 4 ou 5 personnes une voiture etc et que la police municipale et là en présence, il y a une complémentarité d'actions sur le terrain et c'est réclamé effectivement, pardon, parce que le problème, à ce moment-là, c'est de savoir qui tient en respect est-ce que c'est la gendarmerie ou la police municipale, qui a un respect et les autres fouilles ou c'est l'inverse, voilà la vraie question, ça c'est c'est du vécu, c'est du terrain alors naturellement je vais retirer l'amendement mais monsieur le ministre d'État, monsieur mise Aida il faut il faudrait travailler sur ce sur ce cet aspect du code du code pénal, le modifier et je pense que le président de la commission des lois et et le rapporteur devront se pencher là-dessus parce que c'est des réclamée par nos polices municipales,

1 38 rectifier c'est Monsieur Guérini. Monsieur Guérini. Je président le recours croissant à des agents de sécurité privés pour effectuer des missions habituellement assurées par des agents publics, de la police ou la gendarmerie était un autre de nos sujets d'inquiétude dans l'article 1er des dispositions permettant aux agents privés d'assister des proches de l'ordre dans l'exécution du périmètre de sécurité, notamment de pratiquer des palpations de sécurité et des fouilles de bagages, ce qui nous paraît acceptable à condition qu'il soit bien informé, bien formés pour le faire sur le regard vigilant du défenseur des droits, entre autres, nos forces de l'ordre sont soumis à une déontologie de plus en plus élaborés, on peut au contraire s'interroger à ce propos sur la qualité de la formation déontologique de 6 agents privés. Compte tenu de l'importance des recrutements nécessaires avec l'instauration des périmètres de sécurité, pour en revenir à l'amendement l'article prévoit également alinéa 14 de façon un peu crypté, la possibilité pour ces agents de participer à la prévention des éventuels vols, dégradations et effractions et effractions sur le périmètre qui ne concernera pas seulement le lieu de l'événement mais aussi ses abords cette disposition, nous sommes un peu éloigné du test qui vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, c'est pourquoi sauf explications plusieurs profonde dit par le gouvernement de proposant la suppression de cet amendement. Merci Monsieur Guérini, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, donc l'amendement présenté par Monsieur Guérini vise à supprimer l'année la Guinée à 14 de l'article 1er je pense qu'il s'agit là donne alinéa qui opère une coordination avec l'article L. 613 1 du code de la sécurité intérieure afin de prévoir que les agents de sécurité privés puisse intervenir au sein des périmètres de protection. Et il nous semble tout à fait nécessaire de conserver cet alinéa mais je vais laisser comme l'a souhaité Monsieur Guérini le ministre d'État, fournir de plus amples renseignements, et en attendant, je donne un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Monsieur Guérini soulève toujours des questions importantes, mais des questions sur le fond, il est clair aujourd'hui que de plus en plus les agents privés de sécurité prenne une place déterminante dans toute une série de manifestations et donc il conviendra que nous réfléchissions dans l'avenir, alors professionnalisation renforcée à leur formation et donc à faire en sorte que nous puissions avoir dans ses agents de sécurité, une confiance de plus en plus importante, en l'occurrence dans les mesures que nous avons prévu, ils agissent sous le contrôle donc d'un policier ou d'un gendarme et donc ils n'ont pas de rôle majeur je rappelle d'ailleurs que lorsque l'on renvoie quelqu'un hors du périmètre de sécurité s'est toujours donc le policier ou le gendarme qui raccompagne. Merci monsieur le ministre d'État, il y a-t-il des explications de vote, je n'en vois pas je mets aux voix qui est pour. Qui s'abstient, Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je mets on voit donc l'article 1er oui, explications de vote. vote. Je souligne, explications de vote sur l'article 1er oui. Je, je suis désolé je prends au sérieux cet exercice parlementaire. Et j'ai posé une question ma répondu quelque chose le ministre qui n'est pas factuel, puisque j'ai lu et relu l'article de loi, donc je rappelle qu'elle était ma question. Il est nécessaire d'assurer des périmètres de protection n'a parlé de marché Strasbourg, d'autres d'autres événements culturels, sportifs il y avait l'Euro, il y aura 2 événements, je le conçois complètement et je pense que il n'y a aucune raison que l'État, le pouvoir, les pouvoirs publics abuse quand il s'agit de ce type de manifestation. Par contre, nous sommes dans un pays où la liberté de manifester existe et d'ailleurs, le préfet peut interdire une manifestation s'il juge que la situation est telle que pour protéger, on peut interdire mais si elle est autorisée. Et qu'il s'agit de manifestations de contestation par exemple de ce pouvoir, il peut y avoir abus. Avec cet article de loi qui à l'inverse de ce que m'a dit le ministre, ne concerne pas que les manifestations sportives et culturelles, puisque j'ai relu les textes qui parlent. événements soumis à un risque d'acte de terrorisme, a raison de sa nature, de l'ampleur de sa fréquentation. La manifestation dans n'importe quelle grande ville ou à Paris rentre complètement dans cette définition, donc j'aimerais qu'ils me répondent à la question et peut me dire j'assume et c'est quelque chose qu'on doit assumer, mais je ne comprends pas pourquoi on me répond, et c'est les mots du ministre ça ne touche que les manifestations sportives et culturelles, je, je, je demande vraiment qu'on prenne au sérieux notre exercice, je rentre dans ce débat complètement ouvert et comprenant les il s'agit avant tout de protéger les ménages, les, mais là je pointe quelque chose, on me répond à côté, j'aimerais vraiment avoir la réponse est dans le cas contraire, je je ne malgré toute la bienveillante, je ne pourrai voter untel article. Merci monsieur Assouline, y a-t-il d'autres explications de vote sur l'article 1er. Je n'en vois pas.

Qui s'abstient, il est adopté. à l'article 2 un amendement 26 rectifier c'est Madame Ben Bassa Madame Ben ça. Monsieur le président, mes chers collègues, l'article 2 du projet de loi permet au préfet de police à Paris ou au représentant de l'État dans le département aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, d'ordonner la fermeture de lieux de culte dans lequel les propos qui sont tenus les idéaux théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoque à la violence provoque à la commission d'actes de terrorisme au fond l'apologie de tels actes, disons-le clairement : nous sommes ici en présence de l'article, se basant sur l'arbitraire le plus complet, comment définir clairement. Les idées. Ou théorie qui pourrait entraîner une fermeture ce motif imprécis ouvrant en réalité un véritable boulevard aux fermetures vous abusive de lieux de culte, bien sûr, cela ne signifie pas qu'il ne combien pas de fermer des mosquées ou la radicalité de un imam est avérée. Le droit de tout individu a exercé paisiblement son culte que bien sûr, personne dans cette hémicycle n'oserait remettre en question se trouvera profondément bafouée par cette disposition, que penser d'hommes, pays où la pratique du culte est entravée au moindre soupçon. Le commissaire européen aux droits de l'homme ne s'y est pas trompé et s'est récemment inquiété de la portée de cet article 2 susceptibles de limiter considérablement la liberté de culte garantie par l'article 9 de la CEDH enfin. Comment ne pas reconnaître le caractère punitif mais stigmatisant d'une telle mesure pour les communautés religieuses entière concernés, soyons réalistes, cette disposition vise particulièrement les musulmans et l'arbitraire des fermetures ne fera que que raviver un sentiment de stigmatisation et de discrimination à justifie déjà bien installé au sein de cette communauté, cette disposition plus étendues que celles contenues dans la loi sur l'état d'urgence est insuffisamment encadrées menace lourdement la liberté de culte, nous en proposons donc la suppression. Merci Mandanda ça, monsieur le rapporteur de la commission des lois. Merci beaucoup, je le président et Madame Ben Basat propose de supprimer l'article 2 qui institué un pouvoir de police spéciale au profit et du préfère matière de fermeture de Dieu si le

donc c'est un quand même un pouvoir de police générale du maire et qui peut intervenir uniquement pour maintenir l'ordre public, c'est quelque chose qui est quand même un peu daté, en 1905 et s'agissait d'abord de du problème de la séparation des Églises et de l'État et il fallait maintenir l'ordre public, parce qu'il y avait un certain nombre de manifestations il me semble que, ayant relu du histoire locale, le maire de Lyon de l'époque très pratiquant à muscler et déjà interdiction de procession dans sur le territoire de la ville de Lyon a bien changé maintenant, mais à l'époque, c'était assez le choix du gouvernement de créer un pouvoir de police spéciale au profit du préfet ressemblent à la Commission plus adapté et que de se fonder sur la loi de 1905 fermer et des lieux de culte et ce pouvoir est suffisamment encadré, il y aura d'autres amendements qui vont venir en discussion avec le montreront, vous avez raison d'ailleurs de dire qu'il s'agit d'abord de fermer des lieux de culte musulmans de Moscou. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. proposition que nous avons fait donc l'arrêté de fermeture est assortie, je lis le texte d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 48 heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office toutefois sur une personne ayant il y a un intérêt, a saisi le tribunal administratif dans ce délai d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutés d'office avant que le juge des référés mais informer les parties de la tenue ou non d'une audience publique, en application du 2ème alinéa de l'article L. 522 1 du même code si les partis ont été informés d'une telle audience avant que le juge mais statuer sur la demande, c'est-à-dire que il n'y a pas d'arbitraire, mais des des possibilités pour celui qui pense que la mesure justement est arbitraire d'avoir donc un appel au juge en référé.

concernant l'état d'urgence qu'on va faire fi de la loi de 1905 qui autorise la liberté du culte, donc je ne vois pas du tout cette séparation que vous faites,

souvent dans des appartements ou dans des salles dans des toutes petites salles et je crois que il y a un peu de, de personnes qui irait jusqu'à, s'adresser au juge pour mettre en question la fermeture qui a été imposé, donc je, je, je, je suis pas le commissaire de de des droits de l'homme du Conseil de l'Europe n'est pas non plus est quelqu'un qui ne comprendrait pas la loi, donc il y a quand même un problème s'est lui-même également prend

Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre déjà collègues, j'ai le plaisir et le privilège de présider une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes ici plus une mission d'information sur l'organisation de l'Islam, j'ai juste 2 2 observations à faire, la 1ère c'est que la radicalisation en général se fait assez peu déjà dans les dans les mosquées, elle se fait à l'extérieur qui pose problème, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de fermetures de lieux de culte quand il était avéré qu'il avait des problèmes, donc je voudrais que vous me confirmiez que c'était grâce à l'état d'urgence et pas en raison d'une législation particulière et la 3ème qui me pose un léger problème compte tenu d'une histoire partagée, c'est la façon dont les propos seraient rapportés et remonterait jusqu'au préfet qui autoriserait le préfet à prendre des dispositions pour fermer le lieu de culte parce que il faut que quelqu'un les rapporte ces propos, donc là la preuve de de de ses propos pose aussi alléger problème alors je comprends la nécessité absolue de pouvoir fermer des lieux qui prêche contrairement aux vertus de la République et qui prêchent la violence, la question que je me pose, c'est la justification des des éléments qui vont permettre la mais la mise en place de certains articles bien d'être sûr que tout ce qui a été fermé et tous les lieux de culte ont été fermés sous l'ère de Bernard Cazeneuve, l'ont été uniquement dans le cas de l'état d'urgence. Merci madame, il y a-t-il d'autres explications de vote. Monsieur le ministre d'État. Donc, cette mesure a été utilisé même du temps de l'état d'urgence avec beaucoup de, de précaution puisque nous avons eu 17 donc, lieu de culte qui ont été fermés, qu'il y en a 11 qui sont fermés en ce moment, moi j'ai assisté à la fermeture, dans mon département d'un lieu de culte et je dois dire que cela s'est fait en accord avec les autorités musulmanes du département, effectivement, lorsque nous avons mis un délai de 6 mois, c'est pour que le lieu de culte puisse être réouvert avec une autre association cultuelle que celles qui effectivement a valu la dissolution. Merci monsieur le ministre d'État, je mets au voix cette amendement qui est pour. L'amendement de Madame Benbassa. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée.

l'article de vous connaissez l'attachement des membres de leur groupe au principe de laïcité et vous comprendrez donc que nous avons été particulièrement vigilants sur cette partie du texte, il s'agit en l'occurrence de permettent la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos faisant l'apologie d'actes terroristes qui sont proférées, ça n'est pas rien dans la perspective de lutter contre les phénomènes de radicalisation, compte tenu de la diversité des lieux peuvent avoir lieu les pratiques culturelles et non seulement dans des lieux de culte désignés comme tels, nous souhaiterions préciser la rédaction actuelle de l'article, en ajoutant la possibilité d'interdire de se réunir dans un lieu afin d'exercer une pratique culturelle en effet nous sommes important de combattre la tenu de tels propos lors de ce type de réunion religieuse comme ceux tenus dans les lieux de culte identifiés. identifiés. Monsieur le rapporteur. Je comprends parfaitement le souhait des auteurs de l'amendement, qui est de pouvoir fermer tout du culte, la formule qui est contenu dans la loi permet de le faire, donc il y a aucun problème l'abonnement est satisfait et je veux rappeler que cette police spéciale qui écrit au profit du préfet est une police qui est quand même très encadré L'autorité administrative a décidé de fermer halieutique culte, quel qu'il soit avertir personne concernée, il y aura un délai de 72 heures pendant lequel les personnes concernées pourront saisir sur la base de l'article 512 TER, comme l'a dit le ministre d'État, le juge des référés administratifs ça va suspendre il y a pas d'exécution d'office la mesure va suspendre la mesure et c'est lorsque le juge aura rendu sa décision qu'à ce moment-là, si elle est positive décision du juge que la distraction pourra mettre à exécution sa décision, donc c'est un régime très encadrée et qui réalise la bonne bonne exerce équilibre entre la liberté d'être croyant et de manifester son culte et la police, prévention des actes de terrorisme, que l'on met en place, donc je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir retirer leur amendement parce qu'ils ont déjà satisfaction. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Donc, cet amendement, qui se veut de précision vise à inclure dans le Champ de la disposition relative à la fermeture des lieux de culte, ceux des lieux dans lesquels se réunissent les personnes afin d'exercer une partie or il va de soi que telle est bien le cas, les lieux de culte étant ceux dans lesquels est exercée de manière régulière et quelle quelle que soit l'affectation initiale de ce lieu, la notion de lieu de culte au sens des dispositions de cet article et donc plus large que celle des édifices du culte, employé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

Monsieur le président, mes chers collègues, comme nous l'avons vu plutôt l'article 2 du projet de loi permet la fermeture de lieux de culte dans lequel les idéaux théories qui sont diffusés provoqua la violence provoqua à la commission d'actes de terrorisme au fond l'apologie de tels, de la diffusion d'idées aux théories est selon nous un motif de fermeture beaucoup trop large, l'interprétation abusive qui peut être fait de ces 2 tonnes et le flou inhérent qui les entourent sont des facteurs de risques pouvant déboucher sur des dérives et des fermetures de lieux de culte injustifiée Je crois, comme le rappelle le défenseur des droits dans son avis du 7 juillet dernier, je le cite en mettant en place un régime juridique fondée sur la diffusion des idées ou théorie en l'absence de tout acte matériel le texte

que la fermeture ne puisse excéder 6 mois mais il n'est pas fait mention du nombre de renouvellements possibles de la décision de fermeture, l'absence de mention quant au nombre de renouvellements équivaut à de potentiels veut conduction abusive de la sanction, nous estimons également qu'une durée de fermeture de 6 mois constitue une atteinte grave à la liberté de culte, nous proposons donc également sans adhérer à la disposition d'un atténuer les effets en limitant à 4 mois renouvelable une seule fois la durée maximale de la fermeture, je terminerai en reprenant les termes sans appel de la scène CDH, qui rappelle que, je cite, la mise en oeuvre de ces mesures particulièrement attentatoire attentatoire aux libertés obéissent simplement à un principe de précaution, un simple soupçon au rang des motifs légitimes d'intervention confusion des régimes aux disproportion dans les 2 cas, l'état de droit, garante du respect des droits fondamentaux et mise à mal, je vous remercie. Merci madame Van passa le 18 rectifier terre Monsieur le comte.

un article complémentaire au code de sécurité intérieure qui dispose, qui disposerait aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lequel des propos qui sont tenus les idéaux théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoqua la violence provoqua la commission d'actes de terrorisme, au fond, la police de tels actes, la possibilité de prononcer la fermeture du lieu de culte peut découler donc de propos tenus ou d'activités se déroulant dans ce lieu, ce qui est facilement caractérise able néanmoins, comme l'a rappelé, notre rapporteur lors de l'audition au Sénat de monsieur le ministre de l'Intérieur relatives au présent projet de loi les idéaux théories qui sont diffusés sont des notions aux contours très indécis et peu précis, nos lois se doivent d'être claire, précise et intelligible, comme le rappelle également la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce n'est pas le cas en l'espèce de la formule relatives aux idées et théories qui sont diffusés retenue à l'article 2 du présent texte et c'est la raison pour laquelle, nous vous proposons la rédaction suivante dans lequel des propos qui sont tenus les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent je vous remercie. Merci monsieur le comte, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup monsieur président ces 2 amendements aborde il y a 2 questions qui sont abordées dans l'amendement soutenu par Madame Ben Bassa et une question dans l'amendement soutenu par monsieur Leconte

petite mais expérience quand même que l'on a acquis avec la mise en oeuvre de telles mesures dans le cadre de l'état d'urgence, que si on veut rouvrir le lieu de culte, le temps de reconstituer une association cultuelle de trouver des gens qui acceptent de venir alors combien de Sedan sortir d'autres qui tenait avant le lieu de culte, il faut un certain temps et je pense que, 4 mois, c'est trop court, et que 6 mois c'est le Bordelais, d'ailleurs, il suffit de regarder le temps qu'il a fallu pour pouvoir faire des choses donc si vous êtes d'accord de retirer cette partie de l'abonnement après les 2 amendements. Oh pour objet de supprimer l'expression vidéo théories qui sont diffusés dans ces lieux de culte, alors il faut bien sûr pour comprendre le sens de l'avis de de l'avis de la commission, il faut regarder que le mot qu'il y a précédemment, ce sont les propos propos ou idées et théorique, qui sont des fusées et l'a à la commission qu'il y avait quand on dit propos on couvre tous les discours discours et quand on parle, on parle quand on se tait, on se tait, mais que par contre l'abonnement, la position du gouvernement était très insuffisante parce qu'elle couvrait pas les écrits. Et que les propos couvrait idée théorie sans problème, mais qui avait pas l'expression, par écrit, par exemple, les distributions de tracts et et de l'assemblée qu'en recherchant l'intention profonde du gouvernement, il valait mieux mettre propos et écrits plutôt que propos idées ou théorie et que si vous mettiez pas écrit, vous pourriez pas vous fondez sur des distributions de tracts par exemple ou diffusion de de de papier écrit dans ces lieux de culte et que vouloir mettre idée ou théorie après propos et le beau propos général couvre idées et théorie, c'est un discours à propos qui rappelle que des propos c'est une suite de mots qui constitue une phrase que plusieurs phrases constitue un discours que ou côté et et donc qu'à l'aide d'un discours on diffuse des idées et des théories, mais qu'on peut aussi le diffuser à la donne, écrit et vouloir propos et des discours, c'est plus peut-être un peu tautologique, alors que si vous mettez propos écrits vous couvrir la totalité. Voilà la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l'amendement de Madame Ben Basat et Bush ou favorable à l'amendement présenté par Monsieur le comte et ses collègues. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Pour Madame Ben Bassa je ne reprendrai pas l'explication de Michel Mercier pour avoir eu à effectuer dans la pratique ce genre de fermeture, il faut effectivement un certain temps pour retrouver des membres capables de former une association cultuelle de retrouver un imam tout ceci, voyez quand on ferme, ça se passe pas quand même toujours dans la douceur et donc les gens qu'on a fermé son un peu violent par rapport à celles et ceux qui devraient les remplacer et donc ça demande une petite période de transition, lorsque l'on parlait d'idées et de théories, un vous savez que un certain nombre de théoriciens de Daech et de l'action violente, sont visés par la notion que nous avions inscrit dans notre projet de de loi moi si vous voulez. Ajoutez propos et théories écrit en en est parfaitement l'accord mais il faut qu'effectivement la notion de théories parce que vous avez un certain nombre de prédicateurs, je veux dire Dieu qui appellent au Djihad dans leurs théories qui sont, effectivement, j'ai pas sous la main les noms mais je pourrais en donner au Sénat, qui ont une certaine influence sur la radicalisation d'un certain nombre de personnes. Merci monsieur misait à monsieur Richard. Et à la réflexion du ministre que les mesures dont il est question, qui sont des mesures administratives qui vont être prises sous son autorité, ce sont des mesures qui, par construction, seront soumises au contrôle du juge et vous savez bien que le contrôle du juge vise à demander avec insistance administration la justification. De la menace du risque qui sert de base à la mesure, or le texte, il parle des propos points, des points de suspension, qui provoqua la commission d'actes de terrorisme, donc ce qui est la base légale de cette possibilité de mesures c'est que une expression provoque à la commission d'actes de terrorisme et donc, les idéaux théorie ne rentreront dans ce Champ que si votre service localement peut démontrer que ça s'était exprimé d'une façon d'une autre, si ça ne s'est pas exprimée par des propos verbaux ça s'est exprimée par un support écrit, qui peut d'ailleurs être numérique mais la théorie en elle-même si elle n'était exprimée par personne ne pourra pas être retenu comme base légale, donc il me semble vraiment que la formule qui, qui a été dégagé en débat dans la commission,

la question de la liberté de de culture le de religion et bien sûr extrêmement importante et je comprends les éléments de ce débat, je voudrais en même temps souligné que la rédaction qui a été retenu par la commission est assez protectrice et qu'en particulier les dispositions qui peuvent être être liés par exemple à la Convention européenne des droits de l'homme, le sont paradoxalement moins puisque je signale que pour laisser aux DH comme toutes les autres libertés la liberté de religion peut faire l'objet de limitation notamment, je la cite : lorsque le discours religieux ou l'entité religieuse, quelle que soit sa forme, prône la violence et soutiennent des valeurs incompatibles avec la démocratie, c'est un arrêt de la CDH la grande forme du 30 janvier 1998 Réf à participer, donc vous voyez que vous êtes un niveau de rédaction qui êtes même plus exigeante que celle de de la CEDH. Merci Monsieur, bonne Carrère Madame Goulet. Oui, pour soutenir la position de la Commission et l'amendement de monsieur Leconte presque Verba volant, ce qui est permanente, c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir des des écrits Samson. L'aussi évident et juste pour rebondir sur ce qu'a dit le ministre, s'agissant des imams, je pense qu'avec 312 imams formés à l'étranger qui sont dans ce pays, compris, ceux qui viennent de Turquie qui parle pas français, je crois que le dossier de Bernard Cazeneuve concernant la formation des imams en France devient vraiment extrêmement urgente à réouvrir chaud merci.

Un amendement numéro 41. Présenté par monsieur Guérini. Bref, monsieur le président, sur l'amendement 41, nous considérons que la liste des propos susceptibles d'entraîner une fermeture pourrait être étendue aux propos faisant l'apologie du de crimes de guerre, crimes contre l'humanité aux crimes et délits de collaboration avec les

Merci beaucoup monsieur le président, je crois que cet amendement va dans un sens plutôt restrictif parce que, et il s'agit là de fermer des 2 culte parce qu'il y aurait et commission d'infraction pénale, alors que l'autorisation quand même donné à l'abonnement précédent est quand même beaucoup plus large et je dois dire d'ailleurs que cet amendement illustre parfaitement la raison pour laquelle il faut propos écrits, c'est qu'il s'agit du support et et pas de rentrer dans le contenu, d'autres, il appartient au juge de vérifier la proportionnalité donc pour ces raisons et je donne un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Eh bien, comme j'ai dit sagesse pour l'amendement précédent, là je ne vendrai le retrait de cet amendement. Merci monsieur le ministre d'État, Monsieur Guérini.

Oui, Monsieur le président Monsieur, ministre à cet amendement vise cette fois-ci à préciser les éléments pouvant justifier la fermeture des lieux de culte afin d'insister sur la responsabilité de ceux qui les gèrent le bon fonctionnement des cultes repose en 1er lieu sur la capacité de leurs responsables, à faire preuve d'autorité vis-à-vis des membres de leur communauté susceptible de dévier dans les pratiques sectaires ou extrémistes dans la lutte contre la radicalisation, les responsables religieux comme les gestionnaires de lieux de culte doivent donc être au avant poste il constitue un selon crucial pour faire appliquer les lois de la République, cet amendement vise à le rappeler. Merci beaucoup monsieur le président, cet amendement, donc on demande donc précision qui a pour objet d'indiquer que la répétition de propos interdit et justifie la fermeture de lieux de culte, de lieux de culte, ce que je comprends de la lecture de l'abonnement, nous sommes donc si c'est bien le cas, cet amendement est déjà satisfait et quelles conséquences demande aux auteurs de vouloir bien retirer. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Je partage l'avis de Monsieur Mercier, par ailleurs, sur les propos que vous avez pu développer évidemment que l'on essaye de faire en sorte que tous les responsables de culte puisse dénoncer la radicalisation et l'apologie des crimes terroristes et que nous soyons pour un Islam qui soit un Islam républicain respectant effectivement la loi de 1905 tels qu'Aristide Briand la définie comme une loi de liberté de culte, de croire ou de ne pas croire. Merci monsieur le ministre d'État, Monsieur Arnell, vous faites quoi. Il est retiré, merci monsieur Arnell et je mets au voile, article 2 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté

à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, elle met notamment en place la mesure d'assignation à communes la possibilité d'un pointage quotidien et du port de bracelet les chroniques malgré les précautions positive de la commission des lois, qui a notamment supprimé la mesure tendant à obliger la déclaration des numéros d'abonnement ou identifiant de tout moyen de communications extra et qui a surtout organisé un contrôle du Parlement quant à cet article, exigeant notamment à nouveau débat en 2021 sur cette mesure précise ainsi que sur l'article 4 concernant les perquisitions administratives qu'on aille ont été rebaptisée visite évidemment le terme un petit peu différent, nous ne pouvons nous résoudre à faire entrer dans notre droit commun ce genre de mesures individuelles tiré de l'état d'urgence est inspiré, donc d'un dangereux le principe de précaution ces mesures bafouent les droits et libertés des personnes, que ce soit au regard du droit à la sûreté prévue par l'article 2 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, article 7 8 et 66 de la Constitution, c'est pourquoi nous proposons donc la suppression pure et simple de cet article.

tout simplement qu'aux fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser. Des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité dans le public, cette personne peut-être mis sous surveillance, en réalité, assigné à résidence, alors on nous dit : on fait des efforts, on va pourquoi plus loin, on peut l'autoriser à lui à l'à ce que on ne peut pas faire en dehors du périmètre de la commune, on peut même envisager que ce soit tout le département, à la condition que la personne accepte d'être mise sous bracelet électronique, une plus qu'une mesure restrictive de liberté, c'est une atteinte très forte à la liberté, elle est acceptée dans le cas de l'état d'urgence, pourquoi, parce que l'état d'urgence qui n'aurait pas dû durer aussi ont envie la durée, c'était un temps donné pour faire face à un péril imminents.

comportements qui peuvent parfaitement justifié l'ouverture d'une procédure judiciaire, Souad pour apologie du terrorisme, soit pour complicité avec des personnes se préparant à faire des actes de terrorisme dans ce cas-là, la saisine par le procureur de la République d'un juge d'instruction. Le même la mise en place d'un contrôle judiciaire peut parfaitement se mettre en place et on va même plus loin. Lorsque des personnes et nous savons que dans le cas de l'état des gens, c'est des personnes qui ont été assignés à ainsi à résidence pendant une année entière la signifie quoi, la personne est sous contrôle, elle le sait et donc, par définition, elle ne va avoir aucun comportement et donc André alité, ce que les services de renseignement souhaité avoir, c'est-à-dire pouvoir démontrer quelque chose et apporter plus d'éléments, le cas échéant pour permet des poursuites ne se justifiera pas donné untel pouvoir au ministre de l'Intérieur, sans contrôle du juge des libertés, alors je rappelle que le juge des libertés et celui qui, en France, à la compétence, y compris pour les rétention des étrangers, y compris pour les personnes mises en hôpital psychiatrique, ce juge des libertés n'aura pas à contrôler ce que pourra faire le ministre de l'Intérieur, nous donnons la un pouvoir excessif au pouvoir exécutif. Merci Monsieur Migaud Madame Ben Basat, vous défendez le 28 qui est identique aux 2 autres. Monsieur le président, mes chers collègues, l'article 3 concernent les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance issus à la fois des mesures d'assignation à résidence, prévue par la loi sur l'état d'urgence et des dispositions de contrôle administratif des personnes de retour en France d'un théâtre d'opérations terroristes il donne pouvoir au ministre de l'Intérieur, de procéder à la surveille. France 2 personnes répondant à un certain nombre de critères, malgré les quelques améliorations apportées par le rapporteur nous considérons encore et toujours comme dangereuse généralisation excessive des mesures exceptionnelles de police administrative, de surcroît, comme le relève le défenseur des droits dans son avis du 7 juillet 2017 l'imprécision des critères d'application de ces mesures de surveillance constituent une atteinte certaine au principe de l'égalité et de sécurité juridique, faut-il encore le rappeler, cette disposition permet de prendre des mesures de mesure privative restrictive de liberté à l'égard de personnes auxquelles aucune infraction pénale n'est reproché. Cela n'a rien d'anodin. Et en dit long sur la vision de l'État de droit qui semble aujourd'hui dominer, d'autant que le droit pénal antiterroriste a été largement étoffé ces dernières années et de l'ombre infraction de soutien au terrorisme ont été créés, notre arsenal juridique est suffisant, ça n'est d'ailleurs pas qu'une lubie d'écologistes, puisque ce sont aujourd'hui près de 500 personnalités du droit, chercheurs et universitaires, associations, qui dénoncent un projet de loi qui, je cite, hypothèque les libertés de toute de manière absolument inédite en proposant d'inscrire dans le droit ordinaire, les principales mesures autorisées à titre exceptionnel, dans le cas de l'état d'urgence, je vous remercie. Si Madame Ben ça, monsieur le rapporteur de la commission des lois. Oui merci beaucoup monsieur le président, nous sommes saisis de 3 amendements de suppression de l'article 3 du projet de loi il y a là, c'est vrai, une mesure essentielle de ce projet qui est non pas l'assignation à résidence, telle qu'on a connu avec l'état d'urgence, mais qui, qui est une obligation de demeurer dans un territoire qui est au minimum, celui de la commune et qui peut être portée territoire du département si la personne concernée accepte de porter un bracelet électronique, je voudrais dire une chose toute simple, c'est que le terrorisme, c'est pas une action. Contre la société comme les autres. C'est une action qui veut détruire notre société cette le terrorisme est protéiforme, on connaît pas toutes ses formes et il y en a probablement de nouvelles tous les jours, les formes de radicalisation change perpétuellement, les gens sont de plus en plus isolé et décide de de même de commettre des attentats, ensuite il se revendique d'une organisation dont ils connaissent pas grand-chose. Si on ne se dote pas. Dans le droit commun. 2 mesures suffisantes. Pour pouvoir lutter contre nos terrorisme, je crois qu'on aura toutes les difficultés à maintenir notre société alors je sais bien. Il y a pas de liberté. Sans protection, mais qu'il peut pas y avoir de vraies protections sans liberté et et cet équilibre. Qu'on essaye de bâtir, petit à petit dans ce texte, c'est pas facile, c'est pas facile, le plus facile, ce serait de faire un grand discours d'être commissaire à quelque chose quelque part et et de dire aux supprime toutes ces mesures attentatoires aux libertés et on va s'asseoir, Suzanna arbre on regarde et on attend. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que l'État doit agir. Bien sûr se tromper. On peut très bien même avec toutes les tout l'arsenal juridique laisse échapper un terroriste qui est quand même des attentats, il y a eu des attentats sur l'état d'urgence et il y en aura encore, demain, probablement, mais si on a doté l'état des armes efficaces mais aussi des de la liberté. On aura fait notre travail, si on a refusé à des armes pour maintenir la liberté, on aura perdu la liberté. C'est cela, c'est ce dilemme dans lequel nous sommes enfermés, alors c'est un travail très difficile, très délicat, la commission a choisi de ne pas supprimer l'article 3 de ne pas supprimer l'article IV mais nous avons prévu une autre mesure et je ne serai au président le soin d'en parler qui permettra au Parlement de jouer tout son rôle et qui est pour nous essentiel, mais s'agissant spécificité bon de la mesure d'obligation de demeurer de résider dans une commune ou d'autres départements, nous l'avons enserrer. Dans un certain nombre de règles pour réaliser un équilibre entre la le respect de la liberté individuelle et la nécessité la nécessité de protéger ceux qui veulent vivre leur liberté individuelle fait, raison pour laquelle la Commission propose de rejeter les amendements de suppression. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Je crois que nous l'avons rappelé tout au long de ces premiers moments d'examen de ce texte, la menace terroriste est évidemment profonde dans notre pays et qu'elle a comme le disait Alain Richard tout à l'heure, changer d'une certaine manière, de forme. Nous avions une menace terroriste exogène, avec une organisation qui qui pilotait les attentats qui était connu qui était commis, aujourd'hui nous avons une menace beaucoup plus protéiforme où un certain nombre d'individus se radicalise seul. Ou bien lorsque l'on creuse un peu les dossiers avec des réseaux qui ont peut leur apporter à la fois armes soutien logistique et l'on s'aperçoit souvent que le terrorisme et le grand banditisme en quelques fois partie liée,

nous risquons d'arriver toujours après l'attentat. C'est pour cela que nous avons inscrit un certain nombre de mesures, mais en même temps nous avons veillé à ce qu'il y a un texte équilibré, lorsque l'on disait tout à l'heure de manière un peu rapide, que c'était la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun, je vous rappelle qu'il n'y a effectivement pas d'obligation d'assignation à domicile mais que le cadre de déplacement est au moins la commune et comme on vient de le rappeler, si on veut sortir de la commune, la liberté de pouvoir passer parce que c'est une liberté. De pouvoir porter un bracelet électronique qui permet de faire en sorte que l'on puisse contrôler qu'à un moment donné, celui que l'on suspecte de commettre un attentat ne va pas tout d'un coup, comme cela s'est produit dans le passé, disparaître dans la nature j'expliquais que, par exemple, l'un des attentats qui avaient été commis à Lyon vous donc un terroriste avait exécuté son chef d'entreprise de manière horrible en le décapitant c'est parce qu'à un moment donné, les services avaient perdu qu'il était passé d'un département à l'autre et qu'il n'était plus du coup suivi par aucun service si nous ne mettons pas en place ce type de dispositif, alors nous pourrons nous dire nous avons commis des fautes, voyez, par exemple, après l'attentat qui a failli être commis sur les Champs-Élysées, nous nous sommes dits : nous avons des gens qui sont signalés sur tous les fichiers et acquis à un moment donné, on a laissé le droit de port d'arme sans même et c'était une de nos difficultés que nous avons résolu par une circulaire à tous les préfets que les préfets puissent être avertis du fait qu'ils étaient effectivement fichées dans un certain nombre de fichiers de terrorisme, nous avons d'autre part permis que nous puissions avoir donc au juge administratif et je vous rappelle qu'effectivement il n'y a pas une privation de liberté, mais une restriction de liberté et donc c'est le juge administratif, qui doit effectivement être concernés, c'est pour cela que nous n'avons pas le même dispositif entre l'article numéro 3 et l'article numéro 4 ou effective. Maintenant, nous sommes dans une privation de liberté et donc où le juge des libertés doit être effectivement mis dans le circuit et pouvoir intervenir dans ces cas, voilà pourquoi nous sommes défavorables

Je soutiendrai l'amendement de notre collègue et je voudrais vous lire les propos qu'Emmanuel Macron avait fait d'ailleurs, mais ce qu'il avait écrit dans son ouvrage révolutions en novembre 2000 et je pense oui mais d'accord mais si justement, quand on veut faire une le Nouveau Monde, c'est quand même de faire ce qu'on a dit avant, après, j'espère, j'espère en tout cas je partage ce qu'il disait à cette époque, à savoir : nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime de d'exception, il faut donc revenir au droit commun, telle qu'il a été renforcée par le législateur et agir avec les bons instruments, nous avons tout l'appareil législatif permettant de répondre dans la durée à la situation qui est la nôtre car, chers collègues, aucun d'entre nous n'hésite sur la fermeté et la nécessité pour la nation de se défendre âprement contre la menace terroriste, la question centrale, c'est l'efficacité, l'efficacité au regard des principes et ce qu'a dit le président de la République à Versailles et correct quand il explique, on ne peut pas combattre les ennemis de la liberté, en étant soi-même, porteur d'un recul sur ses libertés, c'est ce qu'il souhaite, mais la vraie question aussi c'est il y a-t-il une autre méthode pour être plus efficace, or c'est de cela dont on ne parle jamais, je prends un exemple : on nous explique qu'on va mettre en pourrait en assignation n'ont pas de résidence, mais dans la commune, une personne menacée qu'on suspecte puisque il y a pas de preuves qui tendent à penser qu'on pourrait avoir une démarche juridique, judiciaire aux suspecte de terrorisme, il peut très bien le trucider quelqu'un dans la commune. Je sais pas de de mémoire, j'ai pas regardé mais à Saint-Étienne-du-Rouvray, il me semble que le le le prêtre a été tué par quelqu'un qui était originaire de l'accord, en tout cas qui y habitaient, qui étaient sur place. Ou qui étaient tout près, en tout cas, ça peut être dans sa commune, donc on peut très bien, tout en laissant les gens soi-disant en protection dans la commune et peuvent faire des actes terroristes, ils peuvent rencontrer plein de gens, donc on voit bien que ce genre de méthode n'est pas la plus efficace, par contre renforcer tout ce qui est surveillance renforcée, l'efficacité des services et des personnes sur le terrain, se donner les moyens d'avoir des filatures efficace, pouvoir faire un jugement tout le pluraliste sur quel est celui qui, dans la dangerosité potentielle, on voit bien qu'on a des gens qui étaient fichés S dont on n'imaginait pas qu'ils allaient basculer et que d'autres peut-être, on imaginait qu'ils ont basculé, n'ont pas fait donc il y a tout un travail d'investigation de suivi de renseignements qui sait qui est indispensable et de ces sujets-là, on ne trouve pas en parler pour des raisons ça c'est que ça coûte cher, tandis que imaginer qu'on va pouvoir par des mécanismes de privation de liberté parce que même si ces restrictions de liberté au bout du compte, comme c'est durable et répétitif, ça devient de la privation de liberté, permettez-moi de vous dire que nous reculons sur les principes, nous ne gagnons pas en efficacité, on commence avec le petit doigt et vous allez voir qu'à chaque attentat, on va nous refaire le coup de la énième loi terroriste pour durcir encore plus et pour ne pas être plus puissant pour faire reculer ce fléau qui nécessite la mobilisation de toute la nation et de grands moyens. Merci, merci Monsieur Pilet. Monsieur le président je, je trouve que ce débat une nouvelle fois au nord, le Sénat puisque effectivement nous sommes dans un train débattent sur quelque chose qui est très, très délicat et en ce domaine, je voudrais tout de même qu'on qu'on oublie pas tout à l'heure, nous avons des explications du président les les membres de la commission des lois, peut-être plus apprécié à raison de leur présence pendant les débats, qui, je pense que vous vous pour vous rassurer sur ce qui a été créé par notre rapporteur et par la commission des lois pour prendre toute précaution pour autant sur sur ce texte sur le, sur l'article 3, encore une fois, je comprends les hésitations mais pour autant, on n'abandonne pas du tout, le recours au juge, on n'abandonne pas du tout, le recours au juge puisque, en ce domaine, en toute hypothèse, restera le recours au juge administratif et notre inquiétude traduiraient quelque chose d'un peu particulier : elle traduirait le fait que nous pensons que le juge administratif défend moins bien les libertés que le juge judiciaire, ce n'est historiquement pas vrai et dans la jurisprudence, ce n'est pas vrai aussi, moi je pense que nous pouvons tenter cette solution étant précisé d'ailleurs que si, à la demande d'une personne ayant été assigné trop longtemps et estimant qu'elle n'est plus dans la restriction de liberté mais dans quelque chose de beaucoup plus fort, hé bien on verra par le mécanisme de la QPC intervenir la réponse sur ce point, mais encore une fois en ce domaine ne laissons pas penser par nos propos qui aurait des sous-juges en matière de liberté, de respect des libertés, le juge du tribunal administratif et je suis un prof ont admirateur des juges de l'ordre judiciaire, le juge des tribunaux administratifs de l'ordre administratif ne mérite pas du tout qu'on lui fasse, ne serait-ce que sur un fragment de raisonnement le procès compte d'un mauvais juge en ce qui concerne le respect des libertés. Merci monsieur idée monsieur souligne. Oui, je crois qu'on touche aux 2 articles qui nécessite. Un débat et qui, franchement, que chacun au moins l'avouent qu'ils défendent, même quand il défend ses articles que nous passons à une autre conception, alors vous pouvez dire que c'est à cause de la nouveauté du terrorisme et tout, passons à une autre façon de voir la justice Delmas-Marty Madame a développer cela et je pense que ça mérite qu'on se met aussi à ce niveau, nous étions dans une société de la justice qui punit l'acte. Nous rentrons. Subrepticement dans une société où on punirait par par prévention de l'acte, c'est un changement de paradis, ce n'est pas jusqu'à présent comme cela ainsi finissent ici et c'est pas la peine non plus de faire, nous, nous savons qui vous, vous ne savez pas par certains hochements de tête, c'est un débat d'ailleurs pourquoi on l'a maintenant le terrorisme exister des menaces ont existé, nous sommes en train de, de, de, de, de dire d'autre chose que ce que nous avons toujours dit donc pas d'un revers de main ce que ici dans sa tête Micic tous bords confondus, républicain, nous avons toujours dit.

c'est que oui, nouvelle forme de terrorisme menace notre droit, il doit se parfaire, pour se défendre, a quelque chose de complètement inédit. Et nous avons légiféré pour faire que tout ce qui était nécessaire, de façon permanente, mais qui n'existait que dans l'état d'urgence soient intégrés. Dans les lois, on commence par les débats il y a eu un quinquennat avant. On a fait des lois, on a légiféré, souvent, on a même été en désaccord, mais moi j'ai soutenu ses lois. Parce que je voyais bien la nécessité d'efforts. Quelqu'un comme Monsieur voilà ce qui a été à la vente de ce combat et comme président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et ensuite comme ministre de la justice et qui a toujours défendu de façon très ferme, la nécessité de se protéger, nous dit ce n'est pas la peine, cette loi. Parce que nous avons légiférer de façon suffisante pour lever l'état d'urgence, le président, le précédent président de la République avait dit en juillet dernier, que ce n'était plus nécessaire et qu'il fallait lever l'état d'urgence, il y a eu l'attentat, l'attentat n'a pas eu lieu parce qu'on avait levé l'état d'urgence parce qu'on n'avait pas les moyens puisqu'on était en état d'urgence et donc le problème est de je, je, je, je, je finis d'ailleurs, il y aura l'article 4 on va continuer mais franchement ne galvaude pas, ne faisons pas comme si ce n'est qu'une péripétie, on change et là c'est grave pour les libertés dans cet équilibre et ce défi que nous avons lancé les terroristes qui est de nous protéger de façon sérieuse et les combats de façon sérieuse, sans jamais leur céder le fait qu'ils auront mis en danger les libertés individuelles et collectives sur lesquelles repose notre pays là avec ses articles nous cédons et nous leur donnons quelque part une victoire. Merci monsieur Assouline monsieur Leconte. Président Monsieur mise sur les thèmes chers collègues devant le Congrès, le président de la République nous a dit je rendrai leur liberté aux Français, mais dans le Nouveau Monde on change le monde alors dans le Nouveau Monde, état d'urgence se transforme en état permanent dans le nouveau monde remplace l'assignation à résidence par mesure individuelle de contrôle. Et liberté par quoi va-t-on changer. Oui, depuis quelques années, nous avons fait évoluer le le le le code pénal pour permettre justement de l'année, de, de, de l'adapter aux nouvelles formes de terrorisme pour pouvoir créer de nouvelles incriminations et depuis plusieurs années, nous avons permis d'ouvrir des informations judiciaires et de faire donc dans le respect du juge judiciaire un certain nombre de procédures qui n'était pas possible auparavant. Pour mieux protégée et mieux punir, nous avons même eu le sentiment parfois que nous avions fait tangenter le code pénal avec le principe de précaution ou intégrer le principe de précaution au code pénal parfois lorsque nous avons voté des lois en 2014 et en 2016 en particulier, et pourtant j'ai soutenu, mais là, on arrive à autre chose, il ne s'agit que du code pénal, il s'agit finalement de créer, à côté de du code pénal, à côté des mesures judiciaires qui peuvent être prises. Une seconde voie, d'une certaine manière, une voie administrative est-ce que c'est vraiment la clarté, la clarification, la responsabilité, si on veut vraiment agir efficacement, chacun doit responsable de quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi après avoir tant avancer en se disant : c'est la justice qui doit être la la solution. Maintenant, on nous répond, non ce sont des mesures administratives, hé ben je ne crois pas que nous puissions aller dans cette direction-là, il faut que les choses soient claires, c'est à la justice de

Et de la répression des actes terroristes, je crois aussi que et vous l'avez dit, Monsieur le le ministre, vous avez évoqué Victor Hugo qui disait que finalement il y avait la liberté compte on augmenté on augmentait la responsabilité, la responsabilité, elle est absolument indispensable aujourd'hui pour que chacun soit mobilisée pour défendre la sécurité de notre société, sans cette liberté, il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas opposer les 2 sont ensemble et vous l'avez dit d'ailleurs dans d'autres, dans, dans, dans, dans, d'une certaine manière, on next en faisant une extension de ce que certains auraient pu appeler le le périmètre de la violence légitime de l'État. Que nous trouverons la solution, c'est au contraire dans la justice et dans la responsabilité et enfin je je je conclus : je ne pense pas non plus.

de Saint-Étienne-du-Rouvray et il avait un bracelet. Tronic voyez-vous, donc je suis pas du tout sûr que il y a un aménagement de peine, donc si vous voulez cette cette situation évidemment et dans une guerre totalement asymétrique, évidemment il faut prendre, il faut prendre des moyens, mais moi je voudrais quand même attirer votre attention et et notre collègue Leconte je viens de le dire sur sur les les problèmes de budget parce que la loi sur le renseignement que nous avons voté, les décrets d'application sont pas encore sortis, le texte n'est pas encore en est né n'est pas encore appliquée, nous allons avoir des restrictions de budget militaire, nous avons des restrictions budgétaires de la justice, nous avons encore des des restrictions au ministère de l'Intérieur, je, je, je comprends bien, cette guerre asymétrique contre le terrorisme, mais je vois pas du tout comment en votant ce type de disposition, vous allez pouvoir les mettre en place alors que notre justice est est complètement défaillante par manque, par manque de moyens, très honnêtement, c'est c'est un texte qui est plein de bonne volonté qui est qui, finalement, réprime de plus en plus ses intentions, mais on est d'accord, on ne on on tangue avec le le le principe de, de, de précaution, c'est, c'est une évidence mais avec quoi est-ce que vous allez le mettre en application, Monsieur le Ministre, on est en train de voter des mesures qui ne sont pas financés, qui ne sont pas financés, pas plus que le texte sur le renseignement qu'on nous a fait qu'on nous a fait voter il y a à peu près un an, au motif qu'il était absolument indispensable, et je vous parle pas du PNR dont on parlera peut-être tout à l'heure mais enfin comment est-ce que vous allez mettre ces mesures en place sans gendarmerie dans l'aide sur les territoires sans moyens pour la justice et sans moyens pour nos militaires. Merci. Monsieur le président de la commission des lois. Je vous remercie, Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cet article, je voudrais vous faire part de ma propre conviction d'abord je veux vous dire que c'est inscrit cet article s'inscrit dans le cadre de notre état de droit, il faut le lire en ayant à l'esprit les contrôles qui vont s'exercer sur la décision du ministre de l'Intérieur. Cette décision est assortie de nombreuses conditions, je les ai sous les yeux, il s'agit de prévenir des actes de terrorisme quand il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'individu, constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et leur public et si, ajoute une autre condition soit il entre en relation, de manière habituelle avec des personnes ou des organisations facilitant incitant ou participant à des actes de terrorisme, ce n'est tout de même pas rien, soit il soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et c'est seulement dans ces conditions sont remplies, que le ministre de l'Intérieur peut prendre sa décision et s'il prend cette décision. Soyez certains comme ça été le cas pour les décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence que le Conseil d'État en sera saisi. Et qu'il demandera au ministre de l'Intérieur de démontrer la réalité des renseignements sur le fondement des quelle sa décision aura été prise, alors on me pose la question mais je comptais bien en parler. Pourquoi dis-je que ça s'inscrit dans le cadre de notre être, certains ont dit : il s'agit de punir et quand il s'agit de punir, c'est le juge judiciaire hé bien précisément pas, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de prévenir : nous n'en sommes pas au stade où on recherche les auteurs d'un attentat, pour les punir, nous en sommes au stade où il n'y a pas de victimes forte heureusement et on cherche à éviter qu'il y en a, en prenant des mesures préventives et ces mesures préventives sont plus importantes encore que les mesures punitives bien évidemment car à chaque fois qu'on évitera que des vies humaines soient fauchés par des terroristes, alors on aura rendu le service le plus éminent, qu'on puisse rendre aux Français, c'est-à-dire on aura assurer leur sécurité, et là aussi nous sommes dans le cadre de l'état de droit. Républicain qui distingue bien ces 2 fonctions de prévenir, d'un côté et d'obtenir de l'autre et quand il s'agit de prévenir comprend des mesures administratives qui ne sont pas privative de liberté, il ne s'agit pas d'enfermer quelqu'un. Il s'agit de réduire pour mieux surveiller sa liberté d'aller et de venir dans des conditions précisées par la loi, avec un contrôle qui est celui du Conseil d'État, dont chacun sait son exigence en matière de protection des libertés de vérification de la proportionnalité de la mesure aux finalités que le législateur autorise le ministre de l'Intérieur de poursuivre : je voudrais vous dire aussi qu'il ne s'agit nullement des assignations à résidence pourtant très utile qui ont été prononcées par le ministre pendant la durée de l'état d'urgence car ce régime qui consiste à limiter la liberté de mouvement d'un individu dangereuse, c'est un régime qui est plus souple que celui de l'assignation à résidence, laquelle peut intervenir en dehors d'ailleurs de toute menace terroriste pour un individu qui représentent une menace pour la sécurité, là, c'est seulement quand il s'agit de terroristes, c'est aussi une mesure qui est plus souple en ce qu'elle prend en compte les exigences de la vie professionnelle et familiale de l'individu qui est mis sous surveillance, elle impose qu'ils puisse se déplacer au moins sur le territoire de sa commune et sur un périmètre plus large si le ministre de l'Intérieur le décide et enfin elle elle être prononcée pour 3 mois et son renouvellement va être assorti, grâce aux initiatives de notre rapporteur de conditions extrêmement sévère avec l'intervention obligatoire du juge des référés du tribunal administratif ou du Conseil d'État plutôt. Donc vous voyez que, on a affaire à une mesure qui est une mesure beaucoup plus souple que la mesure d'assignation à résidence, enfin je veux préciser parce que la question de l'efficacité a été posée et c'est une vraie question est-ce que vraiment, monsieur le ministre de l'Intérieur, aura besoin de ce dispositif, ma conviction, c'est qu'il en aura besoin, mais c'est une profession de foi, nous devons pouvoir le vérifier, hé bien, nous avons décidé, à la commission des lois d'imposer au ministre de l'intérieur de nous rendre compte comme il l'a fait pendant l'état d'urgence, des dispositions qui seront prises en application de cet article, c'est-à-dire que chaque année nous saurons combien de cas ont été prononcées, nous serons aussi dans combien de cas, le Conseil d'État aura annulé la mesure du ministre de l'Intérieur et nous serons de la même façon, dans combien de cas, on aura réussi, car c'est un objectif utile à judiciariser la surveillance pour que s'il y a un délit qui puisse être reproché à l'individu mis sur surveillance alors ce soit le juge judiciaire qui engage des poursuites et permettent, éventuellement de condamner l'individu à une peine hé bien ce rapport annuel, servira de base au Parlement. Lorsqu'il devra éventuellement de nouveau se prononcer sur le dispositif que je vous propose de voter car ce dispositif, nous avons prévu à la commission des lois qu'il serait seulement temporaire, c'est-à-dire que ces dispositions législatives tomberont d'elles-mêmes au 31 décembre 2021, si elles ne sont pas reconduites par un nouveau vote de l'Assemblée nationale et de cette manière nous aspirons et du Sénat et de cette manière, nous nous aspirons de nouveau de ce qui existait pour l'état d'urgence, l'une des forces du régime de l'état d'urgence, pour nous ça a été non seulement le contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, mais ça a été notre propre de notre propre contrôle car nous avons mis en place une mission de suivi dans le rapporteur spécial été Michel Mercier, et cette mission de suivi a été doté par le Sénat des pouvoirs d'investigation, d'une commission d'enquête, si bien que nous savons tout de ce qui a été mis en 9 par l'État dans le cadre de l'état d'urgence et, qui plus est, quand nous appliquons l'état d'urgence s'il doit être prolongée nous revote, on est bien de la même façon, ce dispositif s'il doit être prolongée au-delà du 31 décembre 2021, nous devrons revoter c'est une clause d'auto-destruction que nous avons introduit et il faudra que le ministre de l'Intérieur nous démontre que ces mesures auront été véritablement utile comme ça les doutes que vous pouvez avoir aujourd'hui seront soit confirmer soit levé, mais de toute façon, ce dispositif ne survivra pas si les exigences de la lutte contre le terrorisme ne l'impose pas. Merci monsieur le président Monsieur Richard. Monsieur le Président, je Dray ajouter quelques réflexions dans ce débat qui touche au principe. Pour les collègues qui. S'interroge sur les rôle respectif du juge et de l'administration. Je voudrais simplement leur rappeler. Oui. Le principe de séparation des pouvoirs. Dans la séparation des pouvoirs, il y a le gouvernement, l'exécutif, la prévention, la recherche, la de protection de l'ordre public. Son la mission constitutionnelle de l'exécutif et les mesures qui visent à limiter la liberté de mouvements de personnes à l'encontre de qu'il existe des raisons sérieuses de suspicion d'aide au terrorisme relève de la prévention, c'est-à-dire de l'acte de gouverner, ce n'est pas une découverte, donc il est bien logique que cette mission revienne au représentant de l'exécutif, l'exécutif est sous le contrôle d'une justice qui est reconnu par la Constitution, qui la justice administrative. Qui a le même niveau de responsabilité et d'autorité, que l'autorité judiciaire dans son Champ de compétences et comme l'a dit le rapporteur à de multiples reprises au cours des mois qui viennent de s'écouler, les juges administratifs et en dernier ressort, le Conseil d'État ont démontré une capacité de contrôle critique des mesures éventuellement injustifiée qui représente une garantie pour tous les citoyens, enfin sur le sujet des moyens. moyens. Permet d'appeler votre attention sur le fait que la mesure dont on parle s'agissant de personnes qui ont été sous surveillance. Et dont il est vérifié qu'elles ont une dangerosité pour l'aide à des mesures de préparation d'actes terroristes, c'est précisément une économie de moyens, de ne pas avoir à mobiliser des dizaines d'inspecteurs de police pour les filets, mais au contraire de pouvoir circonscrire le mouvement donc, du point de vue de la bonne gestion des des moyens de sécurité, c'est au contraire une mesure d'aide à l'exécutif, qui est à la fois légales et nécessaire.

sur les amendements 6 23 et 28 en vous rappelant que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du gouvernement est défavorable. Et qui va être dans quelques instants au scrutin public

Le scrutin est ouvert.

Et personne ne demande à voter. Le scrutin est clos.

Bien, je vais vous donner les résultats du scrutin numéro 122 sur les amendements 6 23 rectifier et 28 Nombre de votants : 337 Nombre de suffrages exprimés 335 pour l'adoption 106 contre 229 le Sénat n'a pas adopté.

Moins long, monsieur le président, l'article 3 comme les 2 précédents, a fait l'objet d'une attention particulière de notre part, en effet, suite à la réaction de personnalités qualifiées dans la presse, après la publication du projet de loi soumis au Conseil d'État, le gouvernement a accepté de faire évoluer l'article 4 relatives aux visites domiciliaires sur l'article 3, le rapporteur a apporté des modifications substantielles un encadrant mieux le renouvellement de mesures individuelles de surveillance et en supprimant la disposition gouvernementale permettant d'obliger une personne n'a communiqué 6 identifiant et abonnement électronique nous considérons cependant que 2 points restent, monsieur le rapporteur, particulièrement problématique dans l'article 3 : d'une part, la question du contrôle des mesures individuelles des surveillants initiale qui reste, semble-t-il, dévolu au juge administratif, d'autre part, la question du port de bracelet et des chroniques MobilCom comme alternative à l'assignation à résidence, l'objectif de cet amendement et donc de poursuivre le chemin parcouru par le rapporteur et de soumettre la décision de prononcer des mesures individuelles de surveillance à l'appréciation du juge des libertés et de la détention auprès du TGI de Paris, il s'agit de restaurer la compétence du juge judiciaire en la matière, dès lors que c'est mesure ressemblent à celles prévues aux articles 142 55 42 13 du code de procédure pénale, il paraît en effet incohérent Descoutures le juge judiciaire de cette procédure qui lui est pourtant familière et donc chargé des juridictions aux administratifs qui n'applique depuis le début de l'état d'urgence seulement dès lors que cela constituerait possible dernière une charge supplémentaire de travail. Merci Monsieur Guérini, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup monsieur le président je reconnais toute la subtilité de Monsieur Guérini dans cet amendement, mais il y a pas échappé que la commission a choisi.

D'abord, Monsieur le Ministre, Monsieur le ministre d'État pour la vie du gouvernement défavorable et demande de retrait

J'espère que le rapporteur sur la vigilance, cette fois-ci et attentionné, cet amendement vise à alerter le gouvernement sur le risque d'application inégale des mesures individuelles de surveillance selon cannabique, une petite commune une métropole, nous espérons en vue de la rédaction de l'article que ces divergences territoriales seront prises en compte et que la commune constituera rarement le cas d'application de ces mesures, cependant, il s'agit de rappeler l'ensemble des configurations existantes sur notre territoire, comme on l'oublie parfois, lorsqu'on a légifère offert depuis Paris ou Lyon. Merci Monsieur Guérini, monsieur le rapporteur. J'ai bien compris que c'était un amendement de géographie. Et je remercie Madame Coster Monsieur Guérini, ceci dit, il s'agit de de périmètre minimal de la commune au département, la Commission a fait un choix différent, la commission a choisi que le périmètre dans lequel il y a obligation de demeurer était au minimum la commune, rien n'empêche que ce soit le département, ce sera à la décision de l'autorité administrative sous le contrôle du juge,

Bon, moi je vois dans l'amendement de Monsieur Guérini plutôt un attachement viscéral au département, mais le texte, comme l'a dit monsieur le rapporteur, c'est au moins le périmètre de la commune et donc cela peut être si l'autorité administrative, le juge nécessaire, le département, donc il a au moins partiellement satisfaction merci il peut retirer son amendement. Merci monsieur le ministre, donc il y a retiré Monsieur Guérini merci. Un 68 qui est présenté par le gouvernement, monsieur le ministre. L'amendement numéro 68 donc présenté par le gouvernement propose de revenir à la possibilité d'un pointage par jour en effet pouvoir avoir 3 pointages par semaine, cela veut dire que l'on reste comme je l'indiquais au début de ce débat pendant 3 jours, l'individu sans surveillance, et donc cela lui donne le temps et d'échapper à cette surveillance et éventuellement de pouvoir commettre un attentat, donc il nous semble que rester à une nécessité d'aller effectivement pointé auprès d'un commissariat d'une Briatte de gendarmerie territoriale est quelque chose de cohérent. Merci monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, c'est de l'histoire, j'ai bien compris quelle était votre position, mais si j'ai compris quelle était votre position, je comprends pas le fondement ni l'économie générale parce que nous avons un autre système qui a été établi par la loi qui fonctionne et qui concerne les personnes qui reviennent du théâtre irako-syrien qui est, qui est le carton Alain qui est le système de contrôle des gens qui reviennent et du théâtre des opérations,

alors que les personnes qui sont visées par le régime du cartes sur des personnes dont on peut penser qu'elles sont plus proches de passer à l'acte, parce qu'elles reviennent du théâtre irako- syrien en viennent probablement et on peut les surveiller, parce qu'on pense qu'elle revienne pour commettre des attentats, la demande de pointer 3 fois par semaine, là il s'agit pour la mesure qui est prévue par l'article 3 de personnes dont on a alors enseignement ou une source informée, l'administration, qu'il y avait peut-être quelque chose à surveiller chez cette personne. On accepte qu'elle soit placée dans cette obligation demeurer au minimum dans la commune et qu'elle puisse pointer 3 fois par semaine comme le quartier, vous nous dites : non, il faut qu'elle puisse prêter tous les jours, on aurait compris si vous aviez réformer l'carte mais comme vous n'avez pas m'a voulu réformer cartes qui vous a semblé bon outil pourquoi vous priver d'un bon outil que vous avez vous-même choisi donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre d'État pour l'explication de vote. la personne est assigné à domicile, ce qui n'est pas le cas ici pendant 8 heures par jour, donc ça veut dire que la mesure pour le kart et beaucoup plus contraignantes que celles que nous prévoyons ici mais peut-être avez-vous raison et peut-être devrions-nous aussi pour le cas passer effectivement à une assignation par un pointage par jour. Merci monsieur le ministre d'État, vous votez plus à tout le monde m'aurait conquis.

ou bien, comme l'ont dit certains, notamment notre collègue Alain Richard on veut permettre aux services de renseignement et ministre de de surveiller des gens alors qu'ils n'ont pas les moyens techniques et humains de le faire, effectivement, ce soit un pointage un jour tous les 3 jours, ça ne suffit pas, donc la seule solution, je comprends pas pourquoi ne pas proposer, on ne veut pas aller jusqu'au bout la logique c'est d'obliger tout le monde à être sous bracelet électronique, et de cette manière, on arrive à surveiller effectivement les allées et venues, on peut savoir où la personne elle est munie on est muni d'un GPS et on peut savoir que à telle heure à telle endroit elle se trouve là et là, il faut aller jusqu'au bout la logique, ça prouve bien que tout ça est absurde c'est incomplet, ça me confirme dans la volonté de suppressions que nous avions cet article. Monsieur Bigot il y a-t-il d'autres explications. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement 68 présenté par le gouvernement qui a reçu un avis défavorable, si j'ai bien compris l'avis du rapporteur de la commission des lois, et donc je je mets aux voix qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. Un amendement 46 rectifier Monsieur Guérini. Madame jour. Merci monsieur le président, nous avons constaté que le texte mentionne parfois les habitations parfois le domicile des personnes nous nous interrogeons sur le sens de ces variations et nous proposons une harmonisation des termes sauf si ces variations, car en fait des subtilités qui nous échappent. Monsieur le Président, c'est le la question posée par l'auteur de l'amendement est une question tout à fait pertinente qui nécessite l'avis du gouvernement. Et monsieur le rapporteur. Donc, on va demander l'avis du gouvernement. Monsieur le ministre de l'État. Eh bien tout dépend si l'on est latiniste et que l'on pense que domicilié hein de de la maison mais c'est en général aussi le lieu d'habitation, donc nous maintiendrons le lieu d'habitation. Merci monsieur le ministre monsieur Richard pour explication de vote. suis président, je crois qu'il y a une donnée pour répondre à la la question tout à fait pertinente que soulève l'amendement même Jouve il y a une donnée qu'il faut avoir l'esprit, c'est que le domicile est une notion juridique, il y a un lien de droit entre la personne et son lieu de domicile dont elle qui répond à des conditions de droit, donc si on prenait l'expression domicile ça ça ouvrirait des possibilités d'annulation de la mesure, lorsque la personne qu'il s'agit donc il s'agit de limiter les mouvements n'est pas à son domicile juridique mais dans un lieu d'habitation par exemple qui est le résultat de ces contacts de réseau, donc il me semble évident que, dans le la préoccupation de d'efficacité prévention qui motive cette mesure, il vaut mieux prendre le terme d'habitation qui lui correspond à une réalité de fait, c'est-à-dire là où la personne était en habitation en résidence au moment où la mesure est prise alors que la la notion de domicile pourrait faire obstacle à la à l'application de la mesure. Merci Monsieur Richard. Donc, vous le maintenez l'amendement madame jour. Oui, il est maintenu, je n'ai donc on voit qui est pour, non il est pas maintenu, il les retiré, je vous remercie, un 66 rectifier bis qu'il présente Monsieur Guérini. Dans tous nos débats. Relatives à l'état d'urgence et la lutte contre le terrorisme, il a été question de la répartition des compétences entre le juge administratif et du juge judiciaire en effet le fait de créer des mesures j'administratives donc succéder de recours devant le juge administratif concurrente à certaines procédures judiciaires existence conduit à brouiller la répartition des compétences par cet amendement, nous proposons une solution médiane qui consiste pour les mesures individuelles de surveillance initial à mettre en oeuvre un dialogue entre le juge administratif et le juge judiciaire dans un temps imparti, il est donc proposé de contraindre le juge administratif saisi dans ces cas précis, a posé une question préjudicielle au juge judiciaire pour obtenir son avis sur l'opportunité des mesures en cause là où ce n'est pas aujourd'hui qu'une faculté. Le juge administratif éclairé d'une part par l'avis du juge des libertés et de la détention et par la vie de l'administration, à l'origine de la mesure, d'autre part, sera alors en pleine capacité de trancher cet amendement propose donc de prôner un dialogue des juges, selon l'expression consacrée, de Bruno Genevois pour désamorcer une guerre des juges. Et Monsieur Guérini, monsieur le rapporteur. Oui merci beaucoup monsieur le Président, cet amendement propose une collaboration intéressante entre. Le juge administratif et le juge judiciaire, néanmoins, je crois qu'il faut faire un choix parce que la proposition de qui.

référés saisi d'une demande d'annulation de la prorogation éventuelle par l'autorité du stratégique de la mesure d'obligation de demeurer dans la commune doit non pas statuer mais question préjudicielle au profit du gel des de Paris et donc envoyé au gel de Paris attendent qu'se prononce avant de reprendre l'affaire son tour et si pendant tout ce temps,

c'est vrai et je reconnais que Monsieur Guérini a fait d'efforts pour essayer de faire collaborer les 2 juges ensemble et c'est intéressant de ce point de vue, mais il y a aussi, comme disait tout à l'heure, vous avez une manne la question de l'efficacité de l'action administrative par le juge et je lui demande donc de bien vouloir retirer son amendement sinon avides de favoris. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Même avis que monsieur le rapporteur, pensez de Monsieur Guérini toujours riche et complexe, mais peut-être justement trop complexe : avis défavorable. Et Monsieur le ministre d'État, Monsieur Guérini. Il est retiré, merci Monsieur Guérini 2 amendements et un sous-amendement qui font l'objet d'une discussion commune le 65 rectifier n'est pas défendu le 77 rectifier, monsieur le ministre d'État. Bien donc nous entrons avec cet amendement dans le débat que nous avons engagée avec la commission est dans un 1er temps donc proposait de faire appel au JLD et donc nous avons eu une discussion ensemble intéressante la position de la commission a évolué nous-mêmes avons accepté un certain nombre de modifications de la pensée et je crois que nous sommes aujourd'hui en train d'arriver à un équilibre qui est satisfera progressivement les uns les autres quelques nuances sur les questions de durée dont je parlais tout à l'heure et ensuite tout sera parfait. Merci monsieur mini État Monsieur Mercier. Président, je crois, je veux après le ministre d'État, saluer la qualité du dialogue que nous avons pu avoir avec le gouvernement sur cette question, pour nous, il était essentiel qu'il y a pas de renouvellement d'une mesure d'obligation de résider du commune sans intervention d'un juge juge avait pensé aux juges au JLD parce que dans l'article IV on avait utilisé le JLD, mais c'est vrai que l'article 2 il y a un système très intéressant qui a été retenu et qui consiste à ne pas exécuter la mesure de fermeture des lieux de culte pendant un délai suffisant pour qu'on saisisse le juge des référés administratifs à base de référé-liberté et que tant que le juge ne s'est pas prononcé il y a pas d'exécution de la mesure de fermeture des lieux de culte, donc on propose de de reprendre le même schéma, c'est-à-dire que lorsque l'Autorité administratif de proroger la mesure d'obligation de résider dans la commune pour une personne, la personne en cause soit averti, 5 jours avant qu'elle dispose alors de délai de 72 heures pour saisir le juge avait des référés administratifs sur la base d'un référé liberté et que tant que le juge n'a pas statué, il peut pas y avoir de prorogation de la mesure de d'obligation de résider dans la commune, alors c'est une sorte d'autorisation qui est donné à l'autorité administrative par le juge, c'est une autorisation, si la personne concernée et saisit le juge, cela est bien évident ce ministre d'État a fait allusion à une question de durée, je dois dire que que je vois pas bien où il où est le problème parce que dit exactement la même chose, moi je prends la la l'amendement du gouvernement Monsieur le Ministre d'État et je le dis parce que je suis pas bien malin, elles peuvent être renouvelé les les mesures. Or, par décision motivée pour une durée équivalente, c'est-à-dire 3 mois

Et du sous-amendements Monsieur Mercier. Non, mais moi je laisse 3 mois jusqu'à ce que Monsieur le Ministre d'État et trouver une solution en lisant le bas de la page, mais ça change pas la règle. Il faut mieux rédigé le. monsieur le ministre d'État. Monsieur le rapporteur, je pense que ce qui nous pose problème, ce n'est pas ce que vous avez cité c'est plutôt toute décision de renouvellement, prévu au 1er et au 3ème du présent article, c'est cela qui nous pose problème, et donc la difficulté c'est de pouvoir conjuguer 2 choses voilà et donc c'est de pouvoir apporter des éléments nouveaux, comme il a été demandé par le Conseil constitutionnel et en même temps, au bout de 3 mois parce que c'est assez compliqué en 3 mois de pouvoir apporter des éléments nouveaux, donc c'est pour cela que l'on veut faire intervenir nous au bout du 1er renouvellement c'est au bout de 6 mois. là. Ensemble, on est clair, il y a qui a gardé donc la version qui a été élaboré par le gouvernement. Bon alors. La Commission, monsieur le rapporteur, est d'accord avec l'amendement du gouvernement. Non Non et et donc. à ce stade, le gouvernement est défavorable, mais on est d'accord pour examiner dans la navette. le sous-amendement, le gouvernement est défavorable sous-amendement qui étaient présenté donc je fait voter le sous-avoue qui est pour. qui est pour. Il est adopté et l'amendement du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté.

le raisonnement est le même que celui qui était annoncé pour l'amendement 45 donc c'est identique donc là. Absolument. Il retirait merci Monsieur Guérini vous me devancé, monsieur le rapporteur, cette histoire ordinaire.

il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en 9 du dispositif technique permettant le contrôle à distance, prévu au 3ème alinéa pour lequel peut être mis en oeuvre un traitement autonome anisée de données à caractère personnel peut être confié à une personne de droit privé habilités. Je propose la suppression de cet alinéa, j'ai entendu avec attention tout à l'heure notre collègue Alain Richard nous expliquer que dans le cas de mesures de prévention, il y avait un rôle exclusif de l'État.

ce rôle ne peut pas, compte tenu de ce que ça représente en matière de privation de liberté, de surveillance de l'individu qui, je le répète, n'est pas dans une démarche n'est pas soumis à un contrôle judiciaire ne peut pas être transmis à une personne privée, ce n'est pas acceptable, donc je propose la suppression de cet alinéa.

l'avènement de correspond pas à ce que vous souhaitez, parce que vous êtes sûrement favorable au bracelet électronique, mais l'amendement telle que vous le déposez empêche d'avoir des bras qui renaît donc je vous demande de bien vouloir retirer sinon avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État. Pour les mêmes raisons avis défavorable, c'est ce qui est aujourd'hui pratiqué par la justice. Merci monsieur ministre c'est à monsieur Leconte pour l'explication de vote. J'aime bien de la part à la fin de la commission et de du gouvernement l'assurance que c'est un marché public pour les bracelets électroniques et pas le suivi des personnes. J'ai pas de problème pour leur tirer je souhaite avoir cette assurance. à l'assurance, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur.

Il s'agit bien uniquement de la des bracelets et donc ensuite et pouvoir alerter les policiers, les gendarmes Biya il est retiré, merci. 3 amendements et un sous-amendement à 69 rectifier qui est présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre d'État. Bien donc. Il s'agit, mesdames et messieurs les sénateurs, de rétablir la possibilité d'obliger la personne a communiqué ses numéros d'abonnement et rétablir la rédaction initiale sur les interdictions d'entrer en relation, pour ce qui concerne l'obligation à la personne de communiquer ces numéros d'abonnement, nous précisons que ce n'est pas le numéro de code et que nous allons pas écouter les conversations rivés, il s'agit uniquement de pouvoir donner les identifier enfin pour ce qui concerne donc les interdictions d'entrer en relation donc le texte issu des travaux de la commission limite ces personnes à celles pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement, les activités terroristes ces qualifications, c'est que cette qualification est trop restrictive, compte tenu de la porosité entre les activités terroristes et la délinquance ou la criminalité organisée, c'est la raison pour laquelle la référence à un comportement constituant une menace pour la sécurité publique a été préféré par le gouvernement. Merci Monsieur le Président, comme nos amendements précédent cet amendement vise à permettre au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l'opportunité de prononcer les autres mesures individuelles prévues par l'article. Merci madame joue en 78 qui est présenté par le gouvernement, monsieur le ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement numéro 77. Très bien, merci, monsieur le ministre d'État, 82 ans sous-amendements Monsieur Mercier, coordination et vous donner l'avis de la commission sur les 3 amendements, s'il vous plaît. Sur le premier amendement du gouvernement, le numéro 69 rectifier, il faut bien que 1 point désaccord entre le gouvernement et la Commission, et là il y a un vrai point de Bellac il y a 2 dispositions dans l'amendement du gouvernement et dispositions ne soulève pas des problèmes insurmontables, mais qui est inutile et et sur notre poids c'est une disposition, ce qui est également inutile mais à laquelle le gouvernement a choisi de donner un relief particulier et donc pour aller dans le sens du gouvernement, je vais donner un relief particulier à ma réponse il s'agit de l'obligation déclaration des identifiants de communications électroniques des personnes placées dans l'obligation de résider dans leur, Cette mesure a donc pour but de faciliter la surveillance des individus comme lors de l'examen. Et du projet de loi visant à renforcer la lutte contre la criminalité organisée, la loi du 3 juin 2016 ou le Parlement avait rejeté cette mesure, la commission s'est opposée à cette mesure pour 4 raisons. Premières raison aucun cadre juridique n'est prévu pour encadrer la conservation et l'utilisation de ces données, il est prévu que ces données soient communiquées aux services de renseignement pour qu'ils puissent notamment mettre en place des interceptions, or aucune durée limite de conservation de préciser le projet de loi dans le cadre ni les finalités, ni les conditions d'utilisation de se donner des les personnes qui ont accès aucune voie de recours n'est organisé pour permettre à la personne de contester cette conservation, la CNIL a formulé les plus vives réserves sur cette disposition, elle considère également que le Champ des identifiants de communications téléphonie fixe ou mobile, transmission vocale par internet, SMS, courriel, messagerie instantanée, réseaux sociaux susceptibles d'être concernées par la mesure n'est ni préciser ni limité par le projet de loi dans sa décision du donner chambre 2016 PC le Conseil constitutionnel a rappelé la nécessité pour le législateur de prévoir concernant la conservation des données des garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, voilà pour la 1ère raison qui à elle seule ne semble suffisante, mais il y en a 2, il y en a d'autres 2ème raison cette obligation serait sanctionné pénalement. Elle porte donc atteinte aux droits de la défense. En obligeant la personne concernée a facilité sa propre incrimination, or je vous rappelle que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2016 le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser dont découle le droit de se taire à valeur constitutionnelle, sur le fondement de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette mesure paraît également contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans un arrêt rendu en 2017 et sa guerre contre France. 3ème raison pour laquelle nous pouvons qu'être défavorable à cette mesure et la prison, gouvernement, être attentif à cette raison c'est que cette obligation n'était pas exigé pendant l'état d'urgence. Et il serait. Paradoxal d'imposer des obligations plus grande dans le droit commun pendant la mise en oeuvre de l'état d'urgence. 4ème raison qui elle me semble résumer toutes les autres, c'est que cette demande est complètement inutile. Cette mesure proposée par le gouvernement est de nature certes à faciliter la mise sur sous surveillance de la personne, en l'obligeant à livrer elle-même des informations qu'en temps normal, les services de renseignements doivent collecter par l'utilisation de toutes les techniques de renseignement que leur a fourni dans les dernières lois et je suis bien sûr, monsieur le ministre d'État, que pourra prendre la décision d'obliger cette personne de demeurer dans une commune, c'est que vous avez quelques informations, vous n'auriez pas pris décision comme ça, vous avez donc eu des renseignements qui a été fournie par les services de renseignement ils ont trouvé qu'il faudrait placer cette personne dans l'obligation de rester dans sa commune, ils ont sûrement trouvé aussi ses identifiants. électronique donc la commission ne s'oppose pas à ce que toutes les personnes visées par l'article 3 fasse l'objet de mesures surveillance de mise sur écoute notamment, et notamment de géolocalisation l'intégralité du droit commun du renseignement cependant s'appliquer, il appartient aux services de renseignement d'utiliser les procédures rappelé dans la loi de 2015 pour pouvoir pouvoir récupérer les identifiants technique. Connexion je me demande si à la fin de compte, la seule justification de la mesure que vous nous proposez, c'est pas d'échapper à la loi de 2015 comme je veux pas avoir une mauvaise pensée j'ai face tout de suite de elle ne cette mauvaise pensée et je pense donc que vous serez d'accord avec nous pour renoncer à cette mesure inutile qui apportent rien du tout à l'efficacité de l'administration qui va poser des problèmes contentieux difficile vous souhaitez également que supprimer une précision de la commission qui est souhaitée, qualifier les personnes avec lesquelles ne personne a signé d'aurait pas le droit d'entrer en relation par la par par rapport à l'existence d'un risque d'une menace terroriste, le texte de la commission est innocent, monsieur le ministre d'État, nous sommes bornés à reprendre le texte même de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, à savoir l'interdiction de tous les relations avec certaines personnes nommément designé dont le comportement est y à des activités à caractère terroriste, c'est la loi de 2014, que nous avons voté c'est troupes, pas la peine de ne pas l'appliquer, voilà ce que je pouvais dire sur certains mouvements noirs sur l'amendement numéro 64 de Monsieur Guérini et s'agit de supprimer les visites domiciliaires et les saisies dans les perquisitions donc un avis défavorable parce que contraire à la position de la commission. Sion sur le 78 avis favorable sous réserve de l'adoption du sous-amendements, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on sera la même position et on verra ça dans la navette mais on maintient notre sous-amendement numéro 80 2 qui est conforme aux 78. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État sur le 64 rectifier.

mais vous pouvez, Monsieur le ministre d'État. Monsieur Mercier le dit. Que la mesure que nous voulons introduire. N'était pas dans l'état d'urgence. Ce qui est tout à fait vrai. Sauf que. à l'époque de l'état d'urgence. La personne incriminée. Devait pointer 3 fois par jour. être à domicile 12 heures par jour. Donc évidemment, avait moins de risque de le perdre que hors de, état d'urgence et donc dans les mesures que nous proposons ici par rapport comme la mémoire du Sénat Éva j'ai souvenir que la commission des lois, lors de l'examen de 2007 avait peur qu'effectivement le numéro donc le code soit indiqué et donc que les conversations soient et coûté, c'est pour cela que le gouvernement pour suivre votre raisonnement de l'époque a indiqué précisément que ce numéro ne serait pas utilisé le mot de passe, ne serait pas utilisées enfin pourquoi cette mesure parce que si demain la personne achetait ce qui se passe souvent un nouveau téléphone, elle serait et qu'elle ne déclare pas, elle serait effectivement passible de 3 ans de prison ce qui évidemment est un peu dissuasif. Je vais me mettre aux voix, donc le 69 rectifier. Qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour.

Qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et un avis défavorable de la commission. Il est retiré il retiré le 78 qui a reçu. D'abord le sous-amendements 82 de Monsieur merci si et qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est pour. Qui s'abstient, il est adopté, et donc le 78 le d'amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Un amendement 20 rectifier, qui est le dernier de cet article qui est présenté par Monsieur Grand. Merci Monsieur le Président, cet amendement, le maire et de l'autorité de police administrative au nom de la commune, il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité tranquillité salubrité publique, il possède la qualité d'officier de police judiciaire, il y a donc proposé que les maires soient tenus informés des mesures individuelles de surveillance prises à l'encontre de ses administrés, ça a toujours été comme ça dans le temps, je vois pas pourquoi aujourd'hui, ça changerait.

y a 36000 maires qui pourraient être concernés, et on ne peut pas eu diffusé toutes ces mesures comme cela il y a eu plusieurs tentatives d'abonnement de ce type, je comprends pourquoi on a on a accepté ce matin, dans certains cas, qu'il y a une information du maire, c'est tout comme : c'est tout à fait normal, là je crois qu'on peut pas le faire et l'efficacité même de l'action du du strates Yves nécessite que monsieur Grand accepte de retirer son amendement et je le remercie d'avance.

donc les propositions de monsieur grand mais je partage l'avis du rapporteur, ces mesures s'inscrivent en effet dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui relèvent de la compétence des États et donc évidemment l'information doit être gardée discrète, je crois que monsieur le rapporteur, indiquer les raisons si nous partagions des informations avec l'ensemble des maires et quelques chances qu'elle se diffuse un peu.

qui, quelques semaines après, s'est retrouvée mise hors de circuit est aujourd'hui en prison, voilà donc c'est pour ça que je pense que il y a peut-être un juste milieu à voir avec les maires, parce que je me permets de rappeler que nous embauchons-les pour des contrats à durée très déterminée pour l'été, notamment

Oui, cette discussion sur certains sur cet article montre que il s'agit de ce qui est le plus contestable dans cette loi, la volonté de la loi tout à fait louer c'est que il s'agit de nous donner tous les moyens pour faire face au terrorisme, à ces horreurs et ne pas baisser la garde et tous les efforts depuis 2 ans et demi et y compris dans le 1er article était à comment ou maintien cet équilibre entre cette lutte impitoyable cette non-naïveté de la démocratie et la préservation des libertés avec cet article, je pense que nous rentrons dans l'intégration dans le droit commun de mesure typique. D'état d'urgence, c'est-à-dire de mesures exceptionnelles, on m'a rétorqué que non, et notamment en pointant le fait que ce n'est pas une assignation à résidence, mais c'est dans un périmètre, la commune où brasser électronique or Monsieur Mercier, je, je, j'entends l'argument, mais il ne change pas la nature, c'est-à-dire que il est différent d'une mesure d'état d'urgence classiques sur le fait qu'il s'agit pas de l'assignation à résidence, c'est la la dureté, c'est la gradation de la mesure qui qui changent mais pas sa nature, il s'agit bien de punir en limitant la liberté. D'un individu, au lieu d'être chez lui, il peut être dans la commune où il peut être dans le département, mais par nature sans intervention du juge, il y a une décision qui est prise, c'est bien de cela dont dont il s'agit ensuite et je veux finir là- dessus, un autre argument a été donné par le ministre d'État. Notamment concernant sa région pour montrer que, il fallait qu'il y a une traçabilité et cette question de le maintenir dans sa commune, permettez, 2, il donne l'exemple de ce terroriste qui a décapité son patron et si on avait. Tracé le moment où il était dans un autre département et repérés comme radicalisés, on aurait évité pas du tout, là ça a été dit par des collègues à ce moment-là, quand on la repère et je crois que c'était du côté de Besançon, si ma mémoire est bonne, il n'était pas du tout considéré comme pouvant passer à l'acte et relevant des mesures qui sont sanctionnés par cet article de loi, donc le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas été tracées parce qu'il a pas les moyens aujourd'hui pour la police de tracer l'ensemble de ceux qui sont fichier S dans leur parcours et leurs déplacements et leur changement de domicile et donc la question de l'efficacité et la question des moyens que nous discutons peu et j'espère que la loi de finances, on n'en discutera, c'est-à-dire comment on donne les moyens aux services terroristes et à la police de faire face à ce nouveau terrorisme qui effectivement complexe et non pas de penser que par la loi ou ce type de mesures, nous pouvons faire face donc inefficacité atteinte aux libertés, je pense que ça nécessite le rejet de cet article. Merci monsieur Assouline il n'y a pas d'autre explication de vote, je mets au voit donc l'article 3 qui est pour. Qui s'abstient, Qui s'abstient, il est adopté. Je vais suspende la séance, elle sera reprise à 21 heures 45 bien sûr pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.